La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Mes chers collègues. En votre nom. J'ai le plaisir de saluer. La présence dans la tribune d'honneur. D'une délégation du Sénat de la République de Madagascar. La délégation est conduite par son président. Composé de trois sénateurs, dont le doyen et le questeur de cette assemblée. Elle est accompagnée par notre collègue Nassimah Dindar, présidente du groupe d'amitié France-Madagascar et les pays de l'océan Indien. La délégation. Que j'ai reçu ce matin avec Roger Karoutchi avec une souris et la présidente de la délégation est en France jusqu'au 10 avril. Sa visite d'étude s'inscrit dans le cadre des relations privilégiées et que nous souhaitons renforcer. Entre nos 2 pays. En fin de journée elle rencontrera les membres de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation présidée par notre collègue Françoise Gatel ainsi que nos collègues qui composent le groupe d'amitié France-Madagascar et pays de l'océan Indien. Le sénat français. Entretient d'excellents rapports de confiance et d'amitié avec le Sénat de Madagascar et souhaitent. Nous sommes. Particulièrement attentifs. Au renforcement de la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises et bagages dans les perspectives d'assises de la décentralisation, qui se tiendront à Madagascar. Sans doute l'an prochain. Et naturellement. Renforcement avec nos territoires ultramarins. Je pense à la Réunion et à Mayotte tout particulièrement. Permettez-moi mes chers collègues, de souhaiter en votre nom à tous. À notre homologue président du Sénat malgache et à nos collègues sénateurs la plus cordiale bienvenue ainsi qu'un excellent et fructueux séjour dans notre pays.

Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et au respect du temps de parole et je donne immédiatement la parole à notre collègue Mathieu Darnaud. Pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, le président de la République a dévoilé le tant attendu plan au la semaine dernière dans les Hautes-Alpes. à certaines orientations que nous avions nous-mêmes. Pointée du doigt dans le rapport de la délégation à la prospective sur l'avenir de l'eau. Il. Certains points nous inquiète en revanche, s'agissant de la question des financements. Déjà ici au Sénat, notre collègue Rémy Pointereau avait à l'époque dans un rapport, dénoncé que l'eau ne payait plus l'eau, mais que l'eau payer l'État et de constater malheureusement qu'après avoir ponctionné près de 400 millions par an sur le budget des agences de l'eau pour financer l'Office français de la biodiversité. Vous avez souhaité restituer 475 millions d'euros aux agences de l'eau. Habile tour de passe-passe. Cet ingénieux, créatif. Mais la ficelle. Est pour nous un petit peu grosse et. Cela ne nous permettra pas de résoudre les problématiques selon nous impérieuse pour notre pays, s'agissant de la question de l'eau. Nous avons toutefois noté la volonté du président de la République de faire écho à la proposition de loi que nous avons voté ici au Sénat, s'agissant de la gouvernance différencier de l'eau et de la capacité à rendre facultative le transfert aux intercommunalités. Alors ma question est simple et Direct. Écran de fumée ou véritable volonté d'agir. Je vous remercie. La parole est à. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique la cohésion des territoires, vous avez la parole. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Monsieur le Sénateur d'Arnaud. D'abord je voudrais. Vous remercier de vous être rendu hommage à vous-même hein. Je l'avais fait par anticipation en répondant à Guillaume Chevrollier, juste avant le plan au disons que vous retrouveriez une partie de vos petits puisque nous étions appuyé sur le rapport récent de la Cour des comptes sur le rapport de la mission d'inspection après l'été, mais également sur des rapports parlementaires et en particulier sur le rapport de la délégation sénatoriale à la prospective et donc il est logique et légitime que vous saluez des propositions qui, pour un grand nombre d'entre elles ont été reprises. La question des moyens, elle est crucial et. Nous nous sommes appuyés là aussi sur la concertation avec les premiers concernés, les comités de bassin et les agences de l'eau qui avait deux attendent sur la question des moyens, vous avez peut-être été un peu vite sur l'Inde et de. Mais l'annonce de la suppression des plafonds mordant. Qui était attendu sur la totalité des territoires qui était une contrainte sur les niveaux de dépenses et de subventions qui pouvait accompagner les collectivités territoriales. Était une demande unanime des territoires qui est satisfaite dans le cadre du plan eau ensuite il y a la question des moyens. Les près de 500 millions. De supplément de crédit pour les agences de l'eau que vous évoquiez ça correspondait à la fois au chiffrage exprimée par le conseil national et par les comités de bassin partout sur le territoire. Donc on n'est pas dans l'incantation dans la réponse à ces sujets. Et vous, il faut ajouter le milliard d'euros d'Aqua près rendue possible par la Caisse des dépôts et consignations. J'ai bien conscience qu'il avait 2 volets dans votre question. Une concernant les financements une concernant la gouvernance, mais comme il m'a semblé voir que le sénateur Arnaud poser une question juste après vous sur la question de la gouvernance. Je vais commencer à vous répondre dans les 20 secondes qui me restent et je finirai dans la question qui arrive après pour vous dire que c'est tout sauf un écran de fumée. Le président de la République au cours de ses 53 mesure a répondu de manière directe aux interrogations que peuvent avoir un certain nombre d'élus communaux et je vais avoir l'occasion de vous préciser le cap dans lequel nous le faisons dans quelques instants pour ne pas dépasser le temps de parole qui met un parti. Oui, merci Monsieur le Ministre, nous serons très vigilants, compter sur la vigilance du Sénat pour. Veiller à ce que vos propos qui relève du président de la République se traduisent par des actes, mais aujourd'hui l'impérieuse nécessité, c'est d'accompagner nos territoires et au-delà des financements, faire en sorte que leur fléchage permettre à l'ensemble des communes de faire face à ce défi qui est celui de l'eau parce que celui qui vous parle vient d'un département où 26 communes vient de se voir interdire de délivrer des permis de construire et l'enjeu de l'eau, il est là aussi c'est le développement de nos territoires. territoires. Un autre collègue Jean Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste et merci monsieur le président, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, comme ça a été dit par mon collègue Arnaud, le président de la République est venu dans mon département présenté le plan au la semaine dernière. Les mesures présentées dans ce plan ont le mérite de fixer un cap alors que la politique de l'autre tanguer depuis tant d'années. Le président a notamment appelé à une tarification progressive et responsabilisante de l'eau s'autant qu'elle soit en concertation avec les élus généralisée en France. Cela signifie que les premiers mètres cubes seront facturés à un prix modeste proche du prix coûtant puis au-delà d'un certain niveau, plus on consommera plus le prix sera plus élevé. Cela paraît simple sur le papier, en pratique, cela sera beaucoup moins facile. La mesure suppose que les consommateurs soient informés de leur consommation d'eau en temps réel. Pour ce faire, ils vont être dotés de compteurs intelligents. Or, seulement 40% des foyers en possède un. Comment avez-vous prévu de généraliser ces compteurs. Par ailleurs, se posera également le problème de la tarification. Il devra prendre ce problème en compte à la fois le volume d'eau consommé mais aussi les usages qui sont faits de cette eau. Allez vous mettre en place une hiérarchie des usages si oui, comment s'articulera-t-elle avec la tarification progressive je vous invite également à préciser la gouvernance locale de l'eau puisque je n'avais pas envisagé de poser la question mais comme elle est sur toutes les lèvres éventuellement dans votre conscience. J'attends avec beaucoup d'attention votre réponse. Pour vous répondre. La parole est à bord. Monsieur Béchu Ministre de la Transition écologique. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Arnaud vous étiez aux premières loges. À Savines le lac au moment de cette présentation sur. L'ensemble de ces annonces. Le Sénat s'est fait l'écho, y compris au travers d'un vote ici. De l'inquiétude de vouloir fixer une règle qui soit unique en France et posant la question, mais pourquoi est-ce qu'on refuse. De maintenir des systèmes de gestion communaux. Quels sont les indicateurs et les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi on voudrait faire une marche forcée vers l'intercommunalité. Les indicateurs ils existent et ils expliquent le fait que le président a commencé par rappeler que préserver un système de gestion de l'eau avec des communes isolées n'était pas une option. 80% des communes privées d'eau potable. L'année dernière, gérer l'eau de manière seul. 116 des 170 communes dont les niveaux de fuite dépasse les 50% Gerlot. De façon seul mais ce que le président a dit est-ce que je reviens redire aujourd'hui. À l'ensemble du Sénat. C'est que l'enjeu c'est de sortir de la commune isolée sans nécessairement. Aller vers une intercommunalité d'autres formes de mutualisation pouvant prendre le relais. L'enjeu et c'est le point d'équilibre qui ne reste à trouver. Pas de comme seule mutualisation mais des formes qui tiennent compte de la topographie de la géographie de la réalité des territoires. Voilà. Mesdames et messieurs. Le point d'équilibre sur lequel nous pouvons aller sur lequel à l'intérieur. Un bout de mission parlementaire ne permettrait sans doute de préciser la manière dont les choses pourraient se faire. Sur la tarification sociale, voilà un chantier à partir d'un principe simple, il s'agit pas de pénaliser les familles nombreuses. Il s'agit de trouver un dispositif qui fasse en sorte que pour des usages de confort, on soit capable d'objectiver les situations et c'est la raison pour laquelle nous allons confier au CESE, dans un premier temps, une demande de préconisations pour ensuite l'évoquer avec vous, avec les associations d'élus locaux qui ont la responsabilité. De la tarification. Vous serez évidemment associés et entendu, comme vous l'avez été dans le cadre de ce plan lancé par la Première ministre conclut par le président de la République. Monsieur Arnaud. Oui, monsieur le Ministre, le président la République annoncé dans mon département vouloir un modèle pluriel et différencier. J'entends que vous nous annoncez aujourd'hui. Je vous en remercie, la possibilité de créer à nouveau des syndicats pour gérer la compétence au au plus près du territoire. Vous avez également annoncé la création d'une mission parlementaire nous ils collaboreront et je pense qu'il sera nécessaire effectivement de préciser les choses, y compris dans des situations particulières, le maintien d'une compétence communale là où c'est nécessaire, pas forcément partout parce que nous cherchons un compromis les prochaines semaines dans les prochaines semaines pour que nous soyons prêts avant le 1er janvier 2026, date butoir du transfert de la compétence dans tous les cas je salue votre ouverture et nous travaillerons ensemble pour trouver des solutions. La parole est à d'autres collègues. Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste il avait la parole. Monsieur le président. Cher collègue, madame, la Première ministre. Votre réunion avec l'intersyndicale s'est terminée par un échec. À vrai dire, c'était prévisible. Tant votre gouvernement et le président de la République s'en-tête à ne pas vouloir entendre les Français. Le Parlement et le monde du travail. Vous vous êtes engagé dans une stratégie jusqu'au-boutiste. Qui amène au désordre. Comme si vous imaginiez sortir de l'impasse politique et du rejet massif des reculs sociaux. Par la méthode du rappel à l'ordre et de la peur du chaos. Mais les Français ne sont pas dupes. Car c'est une crise démocratique qui s'ajoute à la crise sociale. C'est très grave pour notre pays. Son avenir et la confiance du peuple ont la République. Alors madame, la Première ministre. Il est temps d'atterrir qu'en retirez-vous la réforme des retraites. Pour vous répondre. La parole est au ministre du Travail du plaignant. Toi de l'insertion. Monsieur Olivier Dussopt. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs Madame la Ministre Iman ce matin effectivement avec la Première ministre et son invitation. Nous avons reçu l'intersyndicale. Toute l'incertain de l'intersyndicale puisque l'ensemble des organisations étaient présentes. C'est une étape importante qui a été franchi une réunion importante. Nous avons pu écouter. Chacun d'entre eux et l'échange entre le gouvernement, la Première ministre et les organisations syndicales a été un échange respectueux. Nous avons entendu les désaccords répétés de leur part sur le relèvement de l'âge de départ et pour certains d'entre eux sur la fermeture des régimes spéciaux. Nous avons aussi évoqué un certain nombre d'autres sujets, je pense aux carrières longues. Je pense à la prévention de l'usure professionnelle je pense à tout ce qui fait finalement l'accompagnement des des carrières et un certain nombre de mesures qui jalonnent à la fois la carrière professionnelle et les retraites. le désaccord qui persiste entre les organisations syndicales, le gouvernement et sa majorité sur la question de l'âge n'a pas permis d'approfondir plus avant les thèmes que je viens d'évoquer, nous avons entendu comme vous Madame la Ministre que. Le représentant de l'intersyndicale à la sortie de cette réunion avait indiqué que les mêmes organisations syndicales. Souhaité pouvoir ultérieurement travailler sur ces sujets là nous y sommes favorables et la Première ministre a eu l'occasion de leur dire. Que nous sommes prêts, je vois ce qu'ils seront prêts lorsqu'ils le souhaiteront à ouvrir l'ensemble de ces chantiers à l'occasion de cette réunion, nous avons pu aussi la Première ministre a pu plus singulièrement encore le rappeler, la conviction du gouvernement sur la nécessité de cette réforme nécessité face à un déficit nécessité face un système qui si nous n'agissons pas va se dégrader si vous me permettez cette expression, va aller dans le mur. Donc nous souhaitons mener cette réforme, aujourd'hui le texte et au Conseil constitutionnel. Nous attendons sa décision pour ensuite pouvoir mettre en oeuvre cette réforme. Madame Lienemann. je veux bien qu'on fasse semblant de croire que c'était important de son temps pour entendre les syndicats, mais enfin je m'excuse fallait sourd mais Arcis sourd pour ne pas avoir entendu leurs arguments. Auparavant, les sujets que vous évoquez carrières longues pénibilité. C'est au coeur des débats que nous avons eu ici et pour la réforme. Alors Monsieur le Ministre, puisque ce serait une nécessité fondamentale pour la France. Si vous ne voulez parvenir sur le retrait. Organisé à référendum. N'ayez pas peur du peuple, demandez leur leur avis et leur arbitrage c'est peut être la seule façon de sortir de cet entêtement, qui est le vôtre. Nous exigeons un référendum ou le retrait. La parole est à notre collègue. Michel Dagbert pour le groupe. Du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Il y avait là, monsieur le président. Monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur François Braun Ministre de la Santé et de la prévention. Monsieur le Ministre, ce lundi 3 avril est entré en vigueur la loi Rist et notamment son article 33 relatif au contrôle du plafond maximum pour la rémunération des praticiens intérimaires qui a fixé à 1390 euros par vacation de 24h. Le montant. J'ai eu le 28 mars dernier à la demande du directeur de l'ARS des Hauts-de-France un échange téléphonique avec le directeur adjoint en charge de mon département, ceci afin de faire le point sur les établissements hospitaliers susceptibles de rencontrer des difficultés à la faveur de la mise en oeuvre de cette loi. La surenchère à laquelle était soumis les directeurs d'établissements. Mettent en danger l'équilibre budgétaire de ceux-ci par son impact sur les dépenses de personnel mais elle fragilise aussi la stabilité des équipes médicales en place en ouvrant de façon bien légitime une question éthique. Ces nouvelles dispositions n'ont pas vocation à mettre un terme à l'intérim, dont le coût est estimé à 1,5 milliards mais plutôt a appelé tout le monde a la responsabilité en rappelant avec force les principes déontologiques liées à ces professions. J'en veux pour preuve l'accueil favorable des grandes fédérations hospitalières tant publics que privés, la réactivité de certains établissements proposant d'ores et déjà la possibilité de contrat à durée déterminée. Si ce sujet a fait l'objet de beaucoup d'inquiétude voire de réactions hostiles. La majorité de nos concitoyens attachés à notre système de santé, accueil cette disposition avec satisfaction dans ce contexte, avez-vous Monsieur le Ministre, la possibilité dans une dimension plus large que celle de mon seul la possibilité d'éclairer notre assemblée sur l'impact de celle-ci et les éventuelles remontées de terrain qui sont à votre disposition. Merci. Pour vous réponde. La parole est au ministère de la Santé de la prévention François Braun. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs, 7h, Monsieur le Sénateur Dacbert, je vous remercie de relever que ce gouvernement fait bien appliquer la loi qui a été votée par ce Parlement. Alors dans ce qui nous concerne sur l'intérim et et je reprends ce que vous avez dit c'est bien la lutte contre les dérives de cet intérim qui est importante. Ces dérives qui certes ont une incidence financière non négligeable loin de là. Pour l'hôpital, mais surtout qui aboutissent à la destruction de notre hôpital public quel médecin voudra rester dans l'hôpital public quand ils voient à côté de lui un collègue venir pour 24h et de payer une fois et demie 2 fois plus que lui en un mois. C'est donc une oeuvre essentielle pour la refonte de notre système hospitalier. Mais elle ne va pas sans la reconnaissance aussi en parallèle de la pénibilité des carrières de ces praticiens hospitaliers qui sont la colonne vertébrale de notre service public hospitalier. C'est bien des de choses que nous devons mener de concert. C'est déjà le cas depuis les mesures qui ont été prises cet été je prolonge les discussions avec les syndicats de praticiens hospitaliers pour justement améliorer les conditions de travail des praticiens à l'hôpital et faire revenir tous ces praticiens à l'hôpital alors à l'heure où je vous parle. Il n'y a pas de territoire qui est laissé sans solution. Y compris des zones qui étaient extrêmement compliqué, je pense aux maternités de Carhaix de Landerneau, par exemple, ça fait des mois voire des années, qu'il y avait des difficultés bien grâce à la mobilisation des soignants à l'échelle des territoires entre établissements et je tiens là à le souligner, grâce à l'engagement des ARS nous avons pu trouver des solutions quasiment partout jeudi quasiment parce qu'il existe des points de difficultés qui existait avant cette mise en application pour rester dans le sujet des maternités par exemple, la maternité de Sarlat ou celle de Sedan qui étaient en difficulté avant pour lesquels nous n'arrivons pas à avoir les professionnels mais pour autant, nous avons mis en place des parcours de soins pour les parturientes donc partout, il y a des solutions. Je suis cela de très près avec les ARS 2 fois par jour et nous continuerons dans cette logique territoriale à lutter inlassablement contre les inégalités territoriales d'accès à la santé. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Corinne Ferré pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Ministre. Injuste injustifiable imposer votre réforme des retraites doit être retiré. Demain pour la 11ème journée de mobilisation des centaines de milliers de Français défileront partout dans le pays pour exprimer une fois encore leur colère et leur opposition à cette réforme. Après 2 mois d'un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans très largement soutenue par la population et un parcours parlementaire s'étant achevée par un 49.3. L'absence de réponse de l'exécutif a conduit à une situation de tension extrême dans le pays alors qu'il aurait fallu jouer la carte du dialogue social et de l'apaisement. Vous avez opté pour le mépris, l'essence sans réponse pendant un mois la demande de l'intersyndicale au président de la République d'être reçus en urgence ce silence comme tout ce que vous avez fait pendant des semaines pour empêcher un vrai débat parlementaire en dit long sur votre conception de la démocratie sociale. Alors que les Français sont toujours plus nombreux à comprendre que vous avez essayé de les berner madame, la Première ministre a Denier enfin ce matin recevoir l'intersyndicale ce fut de toute évidence un échec. Alors monsieur le Monsieur le Ministre ne voyez-vous pas que le pays s'enfonce dans une grave crise démocratique quand allez-vous entendre la colère qui s'exprime. Quand allez-vous retirer cette réforme. Pour vous répondre, la parole. Est au ministre du Travail plaide emploi. Monsieur Dussopt. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Je ne reviendrai pas sur la rencontre de ce matin, j'ai dit en réponse à Madame. La sénatrice combien il était important à nos yeux combien nous sommes heureux qu'elle ait pu se tenir dans un état d'esprit respectueux et combien nous sommes prêts avec madame, la Première ministre à ce que sur tous les sujets évoqués. Au-delà de la réforme des retraites, nous puissions avoir un dialogue social le plus productif possible vous dites madame la sénatrice qu'il faudrait retirer la réforme retirer la réforme, madame la sénatrice a signifié laisser les déficits s'accumuler, il n'y a que vous qui imaginez peut être une seconde que lorsqu'on met une réforme en pause les déficits sont en pause. Il n'y a que vous qui. Imaginez que si nous ne faisons pas cette réforme, aujourd'hui les marches ce serait plus facile à gravir, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ne pas commencer. Ne pas faire cette réforme, madame la sénatrice. Ça signifie si vous vous en tenez au seul rapport du conseil d'orientation des retraites. Ça signifie un déficit qui s'accumulent et cela signifie des pensions de retraite qui décroche par rapport au niveau de vie moyen des Français. Nous ne souhaitons pas la pourvu doucement des retraités et nous ne souhaitons pas que le système puisse être engloutis assommée par les déficits, c'est la raison pour laquelle nous agissons, nous agissons et nous le faisons d'autant plus que chacune des alternatives qui nous a été proposé. Chacune des contre-. Propositions qui a été formulée, y compris celles que vous avez porté se serait traduite par une perte de pouvoir d'achat pour les actifs par une augmentation des cotisations par une dégradation de la compétitivité et par une perte d'emploi ou alors par le creusement d'un déficit qui aurait porté sur les générations ultérieures. J'ai souvenir madame la sénatrice, mesdames et messieurs les sénateurs du groupe socialiste. J'ai souvenir d'un esprit de responsabilité en 2013 lorsqu'il a été voté l'allongement de la durée de cotisation, allongement que vous osez nous reprocher aujourd'hui je l'ai voté et vous aussi je l'ai voté en responsabilité vous aussi cet esprit de responsabilité vous a désormais échapper. vous avez fait le choix d'accentuer la crise démocratique et sociale et nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous la sagesse elle aurait été d'écouter les Français, on ne peut pas mettre les gens autour de la table et dire d'emblée que l'on continue à faire comme si de rien n'était. Le dialogue social, ça ne fonctionne pas comme ça parce que, encourager les fractures les tensions dans un pays au bord de l'implosion, ne peut que mener au pire plus que jamais, il importe d'entendre et même de consulter les Français, nous avons proposé d'organiser un référendum d'initiative populaire alors donner la parole au peuple serait véritablement une voie d'apaisement. La parole est à notre collègue. Henri Cabanel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen avez la parole. Président. Madame, la Première Ministre Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues. Madame la Ministre dans un contexte de défiance exacerbée envers les élus. Il est urgent de resserrer les Liens avec les citoyens. Le dialogue en amont des projets la construction sont nécessaires mais il est également urgent de réinventer une culture citoyenne, notamment pour les jeunes qui se ne se sentent ni légitime, ni écoutés ni compris les chiffres de l'abstention en témoignent. J'ai été rapporteur d'une mission à ce sujet, présidée par mon collègue Stéphane Piednoir. Plusieurs outils existent. La journée de défense et citoyenneté la ma morale et civique, le service civique et celui dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois le service national universel. Généralisé obligatoire abandonné remis à plus tard, tout s'est dit. Le constat concernant ces outils et qu'il faut les étudier un transversalité car ils sont inter indépendants. De nombreuses informations ont été données sur le SNU certaines fausses comme à l'amitié réalisation des jeunes. Le SNU généralisée génère des questions sur la compétence des encadrants et les lieux d'accueil et il faut se poser la co-construction avec toutes les parties prenantes, notamment avec les jeunes. Le service civique et il a fait ses preuves, il doit être poursuivi sur longtemps il permet un réel engagement envers la société avec à la clé. CV et une ouverture sur le monde de professionnel. Madame la Ministre commun visés envisagez-vous l'avenir de ce dispositif. Et quid de la générale de la Un débat parlementaire a été préconisée par notre mission l'envisagez-vous et dans quel délai. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Cabanel, vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison. Le rapport qui préconisait, plus de 23 mesure et tout à fait juste. Aujourd'hui, nous manquons d'une culture citoyenne d'une culture citoyenne renforcée et elle se construit, elle se construit en toute transversalité. Monsieur le sénateur dans votre rapport effectivement la mission d'informations, présidée par le sénateur. Mais également, en réalité, complété par le rapport du Saguenay sénateur Jean Saint-tasses sur la question financière du service national universel apporte un certain nombre de réponses. La culture citoyenne, c'est d'abord une culture commune. Ce sont des repères communs, c'est une aspiration à la nation commune ça commence à l'école éducation morale et civique, ça passe par des classes découvertes, ça passe par la reconnaissance de la démocratie scolaire ça continue bien sûr avec la formation de nos enseignants la redécouverte des chantiers de Patrimoine mais ça passe aussi par la relation que nous avons avec nos élus. Monsieur le sénateur, plus que jamais, vous avez raison, nos jeunes boudent les urnes. 9 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés aux dernières élections régionales. Monsieur le sénateur, plus que jamais des conseils de jeunesse des conseils municipaux de jeunes la découverte au sein du service national universel comme genre de de de temps pivot de temps fort mais non exclusif qui vient compléter la journée défense mémoire les questions mémorielles que nous portons avec ma collègue Patricia mais l'Amiral nous permettront demain de renforcer cette force mentale cette force morale la jeunesse elle a besoin d'avoir confiance, confiance dans nos nos institutions, elle a besoin qu'on lui donne. Des temps de rencontres cette mixité, elle doit être sociale et territoriale et monsieur le sénateur, il se trouve que le SNU en ce moment et je sais que ça touchera un certain nombre de sénateurs hé bien permet aux jeunes ultramarins de venir en métropole aux jeunes métropolitains d'aller au bout d'outre-mer des jeunes des territoires ruraux de venir en zone plus urbaine de nos jeunes que demain un jeune d'une zone. Péri-urbaine retrouve je crois la beauté de nos territoires ruraux est une chance, cette chance elle mérite d'être défendue et monsieur le sénateur, je me tiens à votre disposition pour les débats parlementaires au sein des groupes et des commissions. Je vous remercie. madame. Madame la Ministre. Mais voilà, dans le rapport comme vous l'avez cité, nous préconisons un débat, un débat parlementaire. Au ne veut pas se priver de ce débat et c'est un ciel pour pour notre jeunesse. Car le SNU. Le service civique et les autres outils. Peuvent et doivent devenir un outil d'intégration sociale et d'éducation à la citoyenneté. La parole est à l'autre collègue Jacques Fernique. Pour le groupe écologiste solidarité. Victoire. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, Hervé Berville dimanche. Vous avez crânement proclamé avoir fait reculer Bruxelles sur l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées non. Non, vous n'avez pas fait plier la Commission européenne puisque dès le départ, son plan d'action n'était pas contraignant en racontant aux pêcheurs que la commission allait je vous cite condamné la pêche artisanale française dès demain. Vous avez joué un jeu dangereux. Vous avez aggraver un climat déjà électrique à l'encontre des défenseurs de l'environnement. C'est gonflé je crois Monsieur le Ministre de se prévaloir de la cause de la pêche artisanale pour soutenir en fait le chalutage industriel de fond, c'est un peu comme si on subventionnés Amazon en prétendant défendent les commerces de proximité nos pêcheurs n'ont pas besoin d'une telle du prix, ils ont besoin d'écosystème en bonne état si nous voulons pouvoir encore péché dans 20 30 ans vos aires marines protégées sont-elles des supercheries. Quand tu la Commission européenne a recommandé dit cesser le chalutage de fond ben vous avez été pris à votre propre jeu de dupes. Vous avez vu une occasion de vous érigé en héros de la pêche artisanale, fallait oser. Fallait oser. Alors que vous laissez des chalutiers géants détruire la pêche côtière alors que vous vous opposez à la demande de nos pêcheurs d'interdire la scène des maires salle près des côtes. Alors oui, les pêcheurs sont en colère, ils refusent la casse sociale sans solution durable on ne parviendra pas à un apaisement. Nous ne voulons pas qu'un incendie comme celui de l'Office français de la biodiversité à Brest se reproduise. Alors Monsieur le Ministre, plutôt que de pointer du doigt les défenseurs de l'environnement de l'stigmatisé comme certains s'y essaie à fond, et sur tous les fronts ces derniers temps. À quand une cohérence entre vos déclarations et vos actes. On vous répond, on a parlé. Au secrétaire d'État chargée de la mer. Hervé Berville, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Fernique alors désolé de vous le dire mais je ne sais pas où est-ce que vous êtes allés pêcher tout ça mais c'est purement et simplement faux. Je n'ai pas indiqué que la commission avait reculé j'ai indiqué qu'elle avait confirmé ce que je vous avez dit ici au Sénat, le 8 mars c'est que c'était un plan une une communication et qu'est-ce que vous n'avait pas vocation à être traduit en actes législatifs. Écoutez ce qu'il dit au Sénat ici ensuite 2ème élément. La Commission européenne devant les parlementaires européens, avait indiqué qu'elle avait l'intention peut être de le traduire en actes et donc, quand c'est flou, c'est parfois il y a un loup. Et donc j'ai demandé à la Commission européenne quand je me suis rendu au Conseil européen d'avoir la confirmation que oui, en effet, tout ça n'était laissé qu'à la main des États. Ensuite, vous parlez des aires marines protégées. Ça me permet de clarifier les choses. Vous étiez aux responsabilités. Vous avez vous même créer des aires marines protégées entre 2012, et de Louis XIV. Est-ce que tout y était interdit non car le code de l'environnement prévoit qu'il y a 14 type d'aires marines protégées de la réserve intégrale. On ne peut rien faire aucune activité humaine à des aires marines protégées où il peut y avoir des activités de pêche et tous les élus locaux ici littoraux le savent très bien, nous pouvons avoir des activités de pêche qui sont vertueuses qui permettent de protéger l'habitat marin et ma position et celle de l'ensemble des élus locaux des façades littorales a été une position de cohérence. Nous avons fait la démonstration depuis 20 ans en France qu'on peut avoir une pêche côtière artisanale. Est-ce que vous pensez que les pêcheurs à la coquille ravage la planète non est-ce que vous pensez que les producteurs d'huîtres ravage la planète non est-ce que vous pensez que les pêcheurs la langoustine ravage la planète non. Or s'il y avait une traduction législative. C'est ce qui aurait abouti. La fin de cette pêche artisanale. nous assumons de continuer à défendre la pêche artisanale. La pêche côtière. Et donc, nous assumons de continuer à avoir dans des zones près de nos côtes. Cette pratique d'une pêche qui est vertueuse qui a fait ses preuves et qu'il faut continuer à pousser à défendre et c'est ce qu'on a à faire avec vous. Les élus locaux.

Où sont les mesures structurelles pour nos pêcheurs artisanaux pour une pêche durable socialement vivable protéger le statu quo, ce serait à terme les couler. La parole est à notre collègue Franck Menonville. Pour le groupe les indépendants République et Thierry. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Près de 4000 élues ont démissionné depuis le début de leur mandat en 2020 le seuil de 1000 maires démissionnaire est dépassé, a annoncé ce lundi le président de l'AMF dans un entretien au Figaro. Cette vague de démissions et sans précédent et c'est très inquiétant. Pour mon département de la Meuse en des membres en dénombre. La démission de 10 maire 64 adjoint 207 conseiller un président de code comme et un vice-président les élus sont le maillon de proximité de la vaste chaîne des acteurs de l'intérêt général dans notre République. Ils sont positionnés en première ligne face aux nombreux défis actuels pourtant ils exercent leur mission dans un climat parfois délétères. Ils voient leur pouvoir se diluer progressivement notamment avec les transferts de compétences, ils subissent les complexités administratives et les lourdeurs veut bureaucratique pesante qui entravent leur action, sans oublier l'importance des responsabilités qui leur incombent. Il est de plus en plus difficile à construire de concilier l'exercice du mandat avec une vie professionnelle et personnelle. Cela implique donc de, de nombreux sacrifices. Nous pouvons ajouter les actes d'intimidation et les agressions envers les élus qui se multiplient ces derniers temps, nous observons avec inquiétude la radicalité les montée de l'individualisme et le durcissement croissant de la société post-Covid. Les causes qui déprécie l'attractivité du mandat local sont multiples. Monsieur le Ministre, à trois ans des prochaines élections municipales prévues en 2026. Il est urgent d'adresser un message de confiance à nos élus locaux et d'engager une vaste réflexion sur leur statut. Dès lors, quelles initiatives comptez-vous prendre pour restaurer l'attractivité de cet engagement. Revaloriser concrètement le mandat municipal à trois ans du renouvellement. Pour vous répondre, la parole à. Au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Ville merci. Pour cette question. 1293. C'est le nombre très exact de mer. Non pas qui ont cessé leurs fonctions parce que on intègre évidemment pas les décès mais le nombre de démissions de maire depuis le début du mandat. Il faut toujours se méfier des chiffres. Parce que sur les six entre 2014 et 2020. Ce sont 2925 maire. Qui avait démissionné. Et on est donc sur des moyennes comparables de lors de 40 par mois. Mais on est qu'à la moitié du mandat. Et on a eu beaucoup de démissions en tout début de mandat dont certainement. Qui sont liés au Covid, un contexte d'entrer dans la fonction qui a été compliqué. Je le vois dans mon département. Avec des équipes municipales ou la mayonnaise n'a pas prise parce qu'on n'a pas eu le temps et l'occasion de travailler ensemble. Mais pour autant. La conjoncture explique pas tout. Il y a la montée de la violence et je veux saluer à la fois la loi Engagement et proximité qui a permis en 2019 de renforcer la protection fonctionnelle et le texte récent défendue par Éric Dupond-Moretti et par Gérald Darmanin, porté par le RDSE et qui permet de faire en sorte de permettre de mieux tenir compte de mieux répondre avec les constitutions de parties civiles, des associations, il faut évidemment aller plus loin et de ce point de vue il y a 2 moments qui vont compter. D'abord je me tourne vers le président d'Arnaud parce qu'il y a la mission sur l'avenir de la commune et du maire que la chambre haute de l'Assemblée. Se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer essaye d'objectiver ces chiffres dont je parlais il y a quelques instants, c'est souhaitable et c'est précieux. Et puis enfin la semaine prochaine. Élisabeth Borne recevra l'ensemble des associations d'élus, dont David Lisnard avec lequel nous avons commencé déjà discuté de cette question et la question du statut de l'élu dans l'agenda territorial que nous porterons avec Dominique Faure dans la continuité de ses échanges sera évidemment un des sujets qui va rythmer dans les prochains mois la vie démocratique de notre pays. Les maires, ce sont les fantassins de la République, ils sont à portée de baffe de nos concitoyens, ils assument toutes les missions. Il porte toutes les responsabilités. Le moment est venu de regarder comment on peut mieux les accompagner. La parole est à notre collègue Stéphane Le Rudulier. Dans le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre de la justice ces dernières heures. La guerre des gangs, sur fond de trafic de drogue fait rage à Marseille avec. 3 morts, 3 morts de plus et on se dirige, malheureusement. Vers un nouveau record après les 39 morts en 2021. Ces règlements de comptes ont déjà fait plus de 300 morts en 10 ans 300 remonte 300 morts qui font du vieux port et de de Marseille. Un nouveau Medellin. Une nouvelle French Connection, Marseille est aujourd'hui l'otage des cartels et pourtant pourtant les moyens sécuritaires ont été mises en oeuvre. Plus de 300 policiers supplémentaires, 3 compagnies de CRS, 39 points de deal de démanteler. C'est une guerre d'usure et non pas une guerre éclair, certes, mais là où nos forces de l'ordre combattent au quotidien ce cartel. La justice et l'arsenal juridique semble marquer le pas. Alors Monsieur le ministre de la Justice, pensez-vous que la réponse pénale est à la hauteur de la stratégie de déstabilisation des réseaux menée par les forces de l'ordre. Pour vous répondre. Le six. La parole est à au ministre de l'Intérieur. Des outre-mer monsieur Gérald Darmanin. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le secteur de Redu liés par des par des mois de remplacer Monsieur le ministre de la justice mais j'ai pas. Évidemment au nom du du gouvernement pour saluer l'engagement d'abord de nos forces de l'ordre, vous l'avez dit, je vous remercie de le saluer, qui tous les jours à Marseille et ailleurs mais pas si à Marseille ville, à la fois magnifique mais depuis très longtemps vous le savez quand gangrénée par le trafic de drogue. Les policiers et les gendarmes, tous les jours interviennent dans tous les quartiers de Marseille tout et demi-heure font des opérations antidrogue et depuis le 1er janvier à Marseille peut sénateur mais vous connaissez bien ce territoire une tonne de cannabis en trois mois, 509 interpellations de trafiquants. Ce qui monte de l'activité des quasiment 500 policiers Perez, que nous avons mis à la demande du président de la et puis que le 1er ministre a lancé depuis 2 ans et qui agissent en effet en une guerre d'usure, il faut faire davantage et notamment vous l'avez dit il faut que la justice puisse suivre cette activité de police extrêmement important de police judiciaire mais aussi de police de sécurité publique et le garde des Sceaux hier la semaine nationale a précisé les moyens très importants qu'il met à Marseille, particulièrement auprès du parquet de Marseille qui suit particulièrement ces dossiers de trafic de stupéfiants, mais aussi de magistrats de juges du siège également de greffier c'est une centaine de magistrats tout confondu, rien que pour Marseille, qui accompagne, nous le croyons que le garde des Sceaux le travail que nous faisons en commun mais il y a évidemment le fils il y a évidemment la douane il y a évidemment aussi ce que peut faire la ville de Marseille et sa métropole pour aider la police et de gendarmerie et mieux intervenir dans un certain nombre de quartiers, et puis il y a les moyens législatifs dont nous avons besoin, j'ai eu l'occasion de dire ce matin encore devant la commission des lois et dont le président de la commission des lois et devant les sénateurs que l'une des difficultés de la police et de gendarmerie, c'est que les écoutes téléphoniques à la papa, pardon de le dire comme ça fonctionne mal, puisque aujourd'hui les gens passent par Internet par des applications cryptés et que nous n'avons pas la possibilité. Le droit ne nous le permet pas d'écouter ses conversations cryptées. Ce que nous pouvons faire en terrorisme et qui montrent une efficacité est ce que je ne pouvais pas faire pour le banditisme je soumets à votre assemblée cette sagacité cette réflexion pour aider encore la police la justice à être plus efficace. merci Monsieur le Ministre de de votre réponse. Évidemment je pense qu'il faut améliorer la chaîne chaîne pénale notamment. Les places de prison notamment. Le fait de ne pas proliférer de non lieu ou de classement sans suite, parce que ça ça procure o senti un sentiment de superpuissance. Aux narco-trafiquants qui n'hésitent plus maintenant à tuer des mineurs, je comprends votre détermination mais je suis plus inquiet par rapport au, au ministre de la justice qui déclarait il y a peu, qui n'existait pas de coupe gorge en France et je l'invite bien volontiers à Marseille car il existe bien pire encore des narcos cité qui ont fait la sécession et où la Kalachnikov à remplacer Marianne avec un usage débridé des armes à feu. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Florence. Compta. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le S-métolachlore, herbicides agricoles utilisés pour de nombreuses cultures de printemps, notamment le maïs a un impact avéré sur la qualité de l'eau et notre environnement ces produits de dégradation s'accumulent dans les nappes phréatiques pendant des dizaines d'années depuis le 1er janvier 2021. Les les métabolites du S-métolachlore font partie des molécules recherchées dans l'eau, mise en distribution et de nombreuses collectivités ont été confrontés à des dépassements réguliers de la norme un million six. De nos concitoyens sont concernés. L'un des principaux fabricants de ce produit a d'ailleurs indiqué que ces produits ne ne devait pas être utilisée dans les parcelles situées dans les aires d'alimentation de captage d'eau en juin dernier, l'Agence européenne des produits chimiques, a classé cet herbicide comme substance cancérigène et perturbateurs endocriniens suspectés saisi en 2021 par les trois direction générale de l'alimentation de la prévention des risques et de la Santé Lanxess a rendu plusieurs études inquiétantes et le 15 février dernier, lançait sa logiquement annoncé engager une procédure de retrait concernant cet herbicide. Or, à la veille de la présentation du plan eau par le président de la République. Le ministre de l'Agriculture a annoncé devant le congrès de la FNSEA, avoir demandé à Laon ne cesse de revenir sur sa volonté d'interdire les principaux usages du S-métolachlore. Monsieur le Ministre, au titre de la souveraineté alimentaire que nous appelons tous de nos voeux mais qui a parfois bon dos quand il est question de l'usage des pesticides comptez-vous réellement jouer avec la santé de nos concitoyens. En revenant sur la décision de l'Inde cesse de retirer le S-métolachlore est-ce compatible avec le plan visant à protéger la ressource en eau. Pour vous répondre. La parole est. Le ministre porte-parole du gouvernement, monsieur Olivier Véran. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Florence Beatrice, comptable. S'excuse. Le ministre de l'agriculture qui est actuellement avec le président de la République en déplacement en Chine et je vais donc tâcher de de répondre à sa place à votre question. D'abord vous dire que nous partageons. Madame la sénatrice. L'envie de nous débarrasser des pesticides qui ont un impact sur la santé des gens. Vous l'avez dit vous-même. Il est suspecté il est pas avéré mais il est suspecté. Donc le principe de précaution doit l'emporter comme c'est le cas avec toutes les substances qui peuvent avoir un impact sur la santé. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire et c'est le sens de travail que conduit la France et que conduit l'Europe. Ce que je crois comprendre en matière s'agissant de ce de ce pesticide de sa substance. En particulier, c'est que vous l'avez cité, l'enjeu de souveraineté alimentaire mais il y a aussi l'enjeu qui consiste à être capable d'avancer en européen sur ces questions. La France n'est pas une île et que si la France était le seul pays de l'Union européenne à interdire une substance on se retrouverait dans la situation abracadabrantesque où la France hein porterait d'autres pays européens, des produits alimentaires parce qu'elle serait plus capable de produire elles-mêmes ces aliments parce qu'elle n'aurait pu les substances pour pour la cultiver notre bonnes conditions et donc un porterait à grands frais les mêmes produits qui eux auraient été subis soumis aux mêmes substances chez les pays voisins, donc on veut y arriver, il y a les l'Europe je crois donne un je vais pas vous dire de bêtises, mais de, de, ça doit être de 2 ou 3 ans pour pouvoir y parvenir et c'est bien la volonté française de manière générale que de se passer de toutes les substances qui peuvent avoir un impact, je vous le redis sur la santé, c'est un objectif partagé. Monsieur le Ministre, rien ne sert de reporter. C'est une question de santé publique et il est urgent de travailler aux alternatives pour les agriculteurs et donc à leur résilience et je crois que nous avons finalement une occasion de prendre de l'avance sur nos partenaires européens. La parole est à notre collègue Anne Chain Larché pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur Monsieur Gérald Darmanin. En septembre, la France accueille la Coupe du monde de rugby et en août 2024 les JO. 10 millions de passagers supplémentaires sont attendus dans nos aéroports, surtout à Roissy Charles de Gaulle, vaisseau amiral du groupe ADP. Rappelez-vous le groupe ADP. C'est cette entreprise que Bruno Le Maire, voulait à tout prix privatisée en 2019 pour payer la facture des gilets jaunes. Hé bien elle devrait rapporter plus de 150 millions d'euros de dividendes à l'État actionnaire pour 2022. Nous avons bien fait de nous opposer à sa privatisation. Mais revenons à l'avenir proche. Ma question concerne l'organisation des contrôles aux frontières à Roissy Charles de Gaulle où arrivent les vols long-courriers, vous en avez la responsabilité. On nous parle d'embauche à venir mais 355 postes de policiers aux frontières ont été supprimés. On nous parle d'automatisation mais les sas paraphent ces bornes qui lisent les passeports biométriques ne sont pas assez nombreux et sont souvent fermés faute de personnel pour les surveiller. Résultat, il y a parfois jusqu'à 2h d'attente oui 2h pour passer la frontière belle première image de la France face à décède désorganisation ces voyageurs étrangers au fort pouvoir d'achat préféreront atterrir à Bruxelles ou Francfort et regagner Paris en train. L'attractivité de la France est menacée car elle n'est pas prête à faire face. On se dirige vers une pagaille qui risque de ternir encore plus l'image de notre pays. Monsieur le Ministre que comptez-vous faire pour améliorer l'accueil des visiteurs étrangers dans nos aéroports. Pour vous répondre, la parole. Au ministre de matériel. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, je partage avec vous le souci de bien accueillir les personnes étrangères qui arrivent notamment de longs courriers donc notamment tout le matin, c'est le cas de vol, qui viennent de l'Asie où qu'qui viennent. Des Amériques. Lorsqu'ils arrivent dans les aéroports et notamment parisiens et singulièrement à Roissy Charles de Gaulle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accueil est parfait. Non il ne l'est pas et cette responsabilité est partagée entre le groupe aéroports de Paris et la police aux frontières, comme vous l'avez évoqué. La difficulté que nous avons c'est qu'en effet la mise en place d'un certain nombre de traitement automatisé des passeports qu'on appelle le système paraphes et tu en nombre insuffisant et la première décision prise par ADP que nous soutenons, c'est 40%. De paraphes en plus, c'est-à-dire une cinquantaine qui seront installés d'ici cet été, ce qui est une très bonne chose, notamment pour la Coupe du monde de rugby. Deuxièmement, il y a-t-il assez de personnes qui, pour le ministère de l'Intérieur contrôle l'arrivée des personnes pour le point de vue de sécurité non il n'y en a pas assez. 510 personnes sont en cours de recrutement, 300 d'ailleurs d'ici la fin du mois d'avril. Et si le mois d'avril est un mois encore compliqué à passer bien évidemment et nous le renforçons par des policiers venus de l'extérieur cet été j'en prends l'engagement, les choses se passeront au mieux et la publication désormais a été initiée avec ADP chaque semaine de connaître le temps d'attente. Terminal par terminal pour que chacun puisse vérifier des choses. Troisièmement, madame, je pense que la réponse n'est pas le renforcement forcément de policiers aux frontières la police aux frontières, ce sont des femmes et des hommes de la police nationale formé qui porte une arme, et qui mérite d'être de faire des choses parfois plus importante pour le territoire national comme la reconduite des personnes dans leur pays d'origine en revanche qu'il y ait du personnel civil du ministère de l'Intérieur. Formé à la fraude documentaire aux consultation des fichiers contractuelle qui permet de les embaucher plus rapidement encore et notamment c'est le cas en en Seine-Saint-Denis dans l'ensemble de l'Île-de-France. Oui c'est ce que nous faisons ces transformations très forte. Donc, vous l'aurez compris, je partage votre souci votre constat et avec ADP avec la police aux frontières de faisons tout pour être prêt non pas pour la Coupe du monde, mais dès le mois de mai de cette année.

Je pense qu'il faut prendre conscience de la terrible vitrine que nous offrons au monde entier, ça ne Soline les émeutes, les grèves, les mairies et les CRS en flammes, les manifestations, les Black blocs s'elle est bien loin notre douce France. La parole est à notre collègue Nadia sur le groove pour le groupe de l'Union centriste. Son prédécesseur, déclarait le 27 mars 2020. On est dans de telles circonstances exceptionnelles que les fermetures de classes qui se prévoit en ce moment nous les revoyons il ne doit pas y avoir de querelles entre quiconque sur ces sujets actuellement les circonstances exceptionnelles dont parlait Jean Michel Blanquer, c'était la crise sanitaire. En avril 2023. Nous vivons une autre crise profonde tout aussi exceptionnelle qui est aussi celle des territoires et de la ruralité et il faut y apporter des réponses exceptionnelles. Dans ce contexte ce vendredi à Nevers où j'ai eu le plaisir de vous accueillir madame, la Première ministre, vous avez fait des annonces. Les fermetures seront désormais je vous cite prévu trois ans à l'avance afin de laisser aux maires le temps de s'organiser. Je ne vous cache pas ma déception car ce n'est pas ce que j'espérais aussi je veux renouvelle publiquement ma question. Quel message adressez-vous aux maires qui, en avril 2023 désemparés déçu pour certains tenté par la démission dans un contexte local et national particulièrement compliquée espère encore que vous ne fermerait pas leur 1500 classes. Je vous remercie. On vous répond la parole et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement et la formation professionnelle Madame Grandjean. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs à madame la sénatrice Sollogoub. ne tiens déjà à présenter les excuses de monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui est retenue à l'Assemblée nationale pour un débat. Madame la sénatrice. Je voudrais rappeler au préalable de chiffres, moins 300.000 élèves c'est le le nombre d'élèves en moins sur ces 5 dernières années et moins 500.000 élèves prêts à prévoir entre 2022 et 2027. Cette réalité. Madame la Ministre, là évidemment, exprimé vendredi dernier dans votre département qui. Accompagné par les ministres Pap Ndiaye et Dominique Faure a justement pu échanger avec les enseignants, les élèves et les élus sur la question de l'école et notamment l'école en ruralité une fermeture de classe, évidemment, a un impact particulièrement prononcé dans les et communes rurales et c'est ce que la Première ministre a souhaité. Échanger avec vos acteurs. La Première ministre a annoncé effectivement la méthode, une méthode permettant une anticipation sur 3 années, permettant un dialogue avec les élus pour organiser. Cette démographie en baisse qui partout en France. A évidemment un impact sur l'organisation de l'école sur le territoire. Je voudrais dire que cette anticipation bien sûr elle. Elle elle et. Avec une conséquence qui est tout à fait favorable sur le taux d'encadrement, je permets de le rappeler ces 5 46 élèves enseignants pour 100 élèves en 2017 alors qu'on est à 5 98 en 2023. Hé bien que les élus du département et vous-même avez effectivement interpellé Ministre de l'Éducation nationale. Je me permets de rappeler que vous n'avez aucune classe à moins de 24 élèves dans votre département et que nous avons décidé de maintenir 3 classes. Sur ce département, c'est. Bien sûr. Une volonté que nous souhaitons étendre à tout le territoire. Une méthode qui permet l'anticipation et encore une fois, un dialogue avec les élus du département. Nous prenons évidemment en compte la question des écoles en milieu rural et tenons à effectivement la qualité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire. Oui merci beaucoup madame la Ministre, alors moi j'arrive toujours pas à comprendre quand il y a moins d'enfants et le même nombre de professeurs en quoi ça oblige à fermer des classes. Au contraire, on pourrait avoir moins d'enfants par classe dans. S'il y avait moins de professeurs encore ce serait dans l'autre sens mais dans ce sens là. Je ne comprends pas. en ce qui concerne le taux d'encadrement. Je vous rappelle que nous sommes les plus mauvais élèves d'Europe puisque avec 24 élèves par classe, ce sont les pires taux qui puisse exister, la moyenne étant plutôt autour de 22 quant à cette organisation qui ressent plus à une forme de programmation triennale de fermeture. Je vous assure qu'elle ne vient absolument pas en aide des élus d'ailleurs regroupé des classes dans tous les sens, ça veut dire maître des enfants sur la route, organiser des transports scolaires. C'est un coût supplémentaire c'est beaucoup d'organisation beaucoup de fatigue pour les enfants, donc vraiment donné n'ajoutait pas des manifestations, manifestations, ni de la colère à la colère. Donner une année de respiration donner un geste d'apaisement. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Véronique Del Favero pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président Madame le Ministre, mes chers collègues. Pour être très précise ces 4751 élus qui ont raccroché leur écharpe tricolore depuis le début du mandat de 2020. Les chiffres sont ce qu'ils sont. N'empêche que 275 913 adjoints, 3563 élus municipaux ont estimé qu'il y avait trop d'ennuis trop de complexité, trop de violence physique et morales pour continuer sereinement à exercer leur mandat. Trois quarts de ces démissions ont ont eu lieu dans des communes de moins de 1500 habitants. L'engagement public Madame le Ministre attire de moins en moins et ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre démocratie. De plus en plus d'élus locaux expriment leurs difficultés au quotidien pour exercer leur fonction à la fois animateur d'une équipe municipale employeur du personnel communal garant des deniers publics. J'ai souvenir de crise médiateur comptable de fermetures de classes. Ils s'interrogent sur leur avenir. Ces élus locaux jette l'éponge face à l'inflation réglementaire et législative le code général des collectivités territoriales a trippé en 20 ans. Certains élus parlent de harcèlement textuel. Ces élus locaux jette l'éponge face à la baisse des dotations face à l'affaiblissement. Organisé de leurs ressources or aux réformes successives. C'est les ces élus locaux jette l'éponge face au manque de considération du plus haut niveau de l'État pour le mandat le paternalisme d'État exaspérant les maires aspirent à un peu plus de liberté, un petit peu moins de contraintes inutiles Madame le Ministre je suis sûr que vous êtes consciente de ces difficultés. Mais comment allez-vous y remédier. On vous la parole est à la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Madame Dominique Faure. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Del Fabbro. Alors comme mes collègues. Ministres Gérald Darmanin et Christophe Béchu. J'ai eu la chance et vous le savez d'exercer le mandat de maire pendant près de 10 ans et c'est pour moi un des plus beaux mandats de notre République. Dans ce contexte social agité je veux tout d'abord réaffirmer mon soutien notre soutien sans faille à tous les parlementaires et à tous les élus locaux qui ont subi des agressions ces dernières semaines, chaque jour, la liste s'allonge et c'est inacceptable. En ce qui concerne la démission des maires depuis juillet j'ai rencontré personnellement et depuis début juillet, plus de 1000 élus locaux qui me aussi leur bonheur d'être maire mais il ne faut pas le nier. Il y a un malaise, une lassitude dans l'exercice de leurs fonctions ce sentiment a récemment été très bien décrit par le président de l'AMF David Lisnard que je tiens ici à saluer dans sa mobilisation pour ce sujet je sais mesdames et messieurs les sénateurs, que vous êtes également très impliqué sur ce sujet au travers de la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire, présidée par la sénatrice Maryse Carrère. Le gouvernement l'est aussi. La loi Engagement et proximité par exemple le permis en 2019, la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, des plus petites communes, vous l'avez cité, j'ai bien conscience qu'une nouvelle évolution est plus que nécessaire et qu'elle doit dépasser le cadre statutaire à ce mal profond auquel je ne peux me résoudre, nous devons apporter une réponse forte, je reçois et j'échange avec des maires démissionnaires pour en comprendre les causes de la façon la plus précise possible au-delà de celles que vous avez cités et que je partage. Dans les prochaines semaines. Je ferai une proposition pour engager avec les élus locaux, les associations d'élus. L'AMF l'AMRF vous aussi parlementaire dans une démarche large et concertée pour bâtir une feuille de route commune sur la place de l'élu local au sein de notre République et au sein de notre société. Je crois fermement que l'avenir de notre démocratie repose sur les mères, ils sont le visage, ils sont le ciment conclure sont le pilier de notre république. Je vous remercie. Madame le Ministre, je vous remercie beaucoup pour votre réponse sincère ou par laquelle vous dites que vous allez soutenir les maires et j'en suis ravi, puisqu'il il y a à peine 3 mois j'étais encore maire d'une commune de moins de 350 habitants le statut c'est important mais ce n'est pas suffisant. Les maires aspirent à plus d'autonomie à plus de liberté dans ce cas-là, on comprend pas très bien pourquoi étatiser la tarification de l'eau comme le président de la République l'a annoncé. On ne comprend pas très bien la multiplication de tous ces schémas directeurs alors Madame la conclusion je l'espère fait confiance à tous ces élus. La parole est à notre collègue Michel Meunier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Mesdames, et messieurs les ministres, ma question s'adresse au ministre des solidarités. Monsieur le Ministre, je ne vous parlerai pas de fin de vie, ni de fin de carrière professionnelle, même si ce sujet préoccupe les Françaises et les Français, je parlerais de la fin du mois des plus précaires d'entre eux RSA allocation adulte handicapé. Minimum vieillesse, les minima sociaux ont été revalorisées de 1,6%. Le premier avril dernier après une hausse de 4% l'année dernière en juillet en comparaison à la hausse du coût de la vie, c'est loin d'être suffisant. Les plus modestes subissent une inflation de plus de 7% en un an et le budget alimentaire c'est même supérieur à plus de 14%. Les dépenses du budget de d'un ménage d'une femme seule avec 2 enfants augmente de 170 euros par mois et ses prestations et allocations, elles augmentent de 17 euros par mois, 10 fois moins. La sonnette d'alarme a été tirée par le collectif Alerte qui comme vous le savez, fédère 34 organisations de lutte contre les exclusions, elle souhaite l'indexation des minima sociaux sur les Budgets de référence des ménages modestes comme les calculs est fait pour le SMIC, elles exigent dans l'immédiat Pour vous répondent. La parole est au ministre des solidarités, de l'autonomie des personnes handicapées. Monsieur Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice Michèle Meunier. Je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de rappeler que depuis le depuis 18 mois le gouvernement agissant relâche pour lutter contre l'inflation et en particulier contre l'inflation à la racine, avec le bouclier tarifaire sur l'énergie. Avec l'ensemble des mesures qui ont été prises pour maîtriser. L'inflation vis-à-vis des Français. Les prix ont accéléré au cours de l'été 2022. Il vous l'avez dit, nous avons pris la décision de revaloriser de façon anticipée les minima sociaux de 4% parce que les les plus modestes ont été les plus exposés à l'augmentation des prix à la rentrée scolaire 2022. Nous avons distribué une aide exceptionnelle de solidarité de 160 euros en moyenne par ménage à la rentrée et nous avons continué les prix, les prix pétroliers ont été les plus dynamiques a augmenté en cette fin d'année nous avons mis en place un chèque énergie de 100 à 200 euros par ménage et vous l'avez dit, à partir d'avril. Depuis le premier avril, les prestations sociales ont été revalorisées de plus de 5,6%. Sur 12 mois, c'est le niveau d'inflation calculée strictement par l'Insee au cours de ces 12 derniers mois et donc jusqu'à présent notre réponse face face à l'inflation a été à la hauteur et a permis de protéger les Français face à la hausse des prix, en particulier les plus modestes en 2023. On a un défi majeur, c'est celle de la poursuite de cette inflation, en particulier sur les prix de l'alimentation, c'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités et lancé le trimestre anti-inflation pour permettre un accès aux produits de première nécessité dans les supermarchés. C'est pour ça également que nous avons mis en place le programme mieux manger pour tous pour permettre un accès aux ménages les plus modestes à des produits de qualité puisqu'on sait que ce sont les produits qui sont arbitrées en 1er par ces ménages les plus modestes. Je pense aux fruits et légumes à la viande au poisson, bref à tous les produits de qualité dont les Français ont besoin. J'ai réuni il y a quelques jours, l'ensemble des associations de solidarité pour faire le point avec exclure et nous nous reverrons dans deux mois pour faire un point sur la situation et prendre les mesures nécessaires si la situation perdure. Monsieur le Ministre, nous sommes loin du compte et pour répondre à cette crise, il faut des politiques publiques de redistribution et de sortie de la précarité c'est incompatible avec la politique fiscale de votre gouvernement qui concentre les baisses d'impôts sur les entreprises et les plus aisés des Français on savait cette politique dangereuse pour le climat et on la c'est maintenant aussi alarmante pour le climat social. La parole est à d'autres collègues, elle se Joseph pour le groupe Les Républicains. Ce le président. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre pays subit en matière de santé hein, véritables des aménagement du territoire avec une fracture territoriale qui ne cesse de s'accroître. Ce problème existe depuis plus de 20 ans et concerne de manière dramatique toutes les formes de l'exercice médical en France. Mais ce sujet n'a pas fait l'objet d'un moindre programme du président de la République pendant sa campagne. Si nous sommes sensibles aux excès produit par les fonctions intérimaires à l'hôpital. La loi Rist risquent d'augmenter et d'aggraver la problématique des déserts médicaux dans certaines régions. Nous manquons cruellement de médecins d'anesthésistes de gynécologues de psychiatres et bien au-delà. Certains habitants en France sont en grand danger de perte de chances et de manque de soins et surtout dans notre ruralité. Un récent rapport, remis à l'Académie de médecine envisage la suppression d'une centaine de maternités pour tout établissement pratiquant, moins de 1000 accouchements. La maternité de Sedan dans les Ardennes est ainsi visé et il a été annoncé la suspension provisoire d'activité des accouchements par manque de professionnels. Cette invitation fermetures de maternités repose sur un critère arbitraire. Elle se nourrit d'une vision purement comptable de la médecine et d'une approche réductrice de ce qui est une naissance. Certes, vous avez augmenté le numerus clausus, mais le nombre de places dans les facultés n'augmente pas comme il le faudrait et dans certaines spécialités, les choix que vous faites en matière de répartition des places d'internat ne sont pas toujours judicieux et aggrave le phénomène. La situation est l'avenir de la maternité de Sedan ne nous rassure pas. Les appels à la réserve sanitaire sont aujourd'hui infructueux Net ne doit pas devenir un soin difficiles et un parcours du combattant, mais rester un apport un moment important et Secure, Monsieur le Ministre comptez qu'entendez-vous faire pour que la santé des femmes et de leurs enfants ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la comptabilité au nom de conception technocratique qui ont déjà tant fragiliser notre pays. Qu'envisagez-vous pour que nous ne passions pas d'une suspension provisoire à une suspension définitive et n'avoir plus ainsi qu'une seule maternité dans le département des Ardennes. La situation est extrêmement grave et je peux vous dire que les Français la ressentent. Merci pour moi et pour la parole est au ministre de la Santé de la prévention. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Joseph. Effectivement, lutter contre les inégalités territoriales d'accès à la santé est une de mes priorités, vous le savez très bien. Pour autant, il faut dire la vérité et dire continuellement la vérité aux Français, nous n'aurons pas 10.000 médecins de plus demain en claquant des doigts, heureusement lors du mandat précédent le numerus clausus a été déverrouiller. Ce qui a permis déjà aujourd'hui d'avoir 15% de médecins de plus qui rentre en deuxième année de médecine. Pour autant, vous le savez comme moi il faut 10 ans pour faire un médecin, donc nous n'aurons pas de résultats en terme d'effectifs demain même si même si nous travaillons en permanence pour augmenter cette disponibilité de temps médical en s'appuyant entre autres sur les autres professionnels de santé et particulièrement les sages-femmes en ce qui concerne les maternités Le rapport du professeur Yves Ville est un rapport scientifique fait pour l'Académie de médecine, ils n'engagent bien sûr en rien le gouvernement c'est un des éléments de la discussion mais concernant précisément les les maternités, vous savez parfaitement que la complexité et d'associer proximité mais surtout sécurité des soins et il est de ma responsabilité comme ministre de la Santé de la prévention d'assurer cette sécurité partout sur le territoire ce extrêmement complexe au niveau de cette équation parce que nous manquons de professionnels. Les établissements les services les maternités ne ferme pas parce que pour des raisons financières ça c'était avant, aujourd'hui c'est pour des problèmes simplement d'effectifs médicaux. l'engagement que j'ai pris et que je continue à à tenir, c'est de trouver des solutions sur chaque territoire d'organiser des parcours de santé pour les parturientes partout y compris à Sedan la maternité de Sedan qui est. Relayée par la maternité de de Charleville-Mézières à proximité nous mettent en place des solutions innovantes au niveau local, que ce soit les Centres de périnatalité, mais que ce soit aussi des exemples comme depuis quelques jours à Autun sur décembre de maternité qui permet à la femme de rester jusqu'à l'accouchement près de chez elle et dans les 12h suivantes revenir au même endroit, c'est là-dessus que nous devons travailler collectivement avec les élus dès maintenant je vous remercie. Madame, la parole et l'autre collègue Annick Jacquemet. Pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'action et des Comptes publics monsieur Gabriel Attal. Elle porte sur la compensation pour l'année 2023 de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE dont la suppression progressive sur 2 ans, a été acté par la dernière loi de finance en compensation de cette perte de ressources fiscales, les collectivités territoriales se voir affecter une fraction de la TVA. De manière pérenne et dynamique. Toutefois, depuis l'annonce des montants individuelle de compensation de la CVAE notifié aux collectivités avec 3 mois de retard. Les élus locaux concernés ont publiquement fait part de leur incompréhension. Selon l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. L'AMF. Les chiffres transmis montrent que dans certaines collectivités le montant de la compensation théorique est nettement inférieur à celui de la CVAE qui aurait été perçu en 2023. L'engagement pris par le gouvernement de compenser à l'euro près la CVAE n'est donc pas tenu cette année ce sont près de 650 millions d'euros qui manquent à l'appel. Le choix du gouvernement de calculer la fraction socle de la compensation sur la moyenne des années 2022 1023 est également contestée. Sans remettre en cause la nécessité de calculer la répartition de la compensation sur plusieurs années afin de lisser les écarts, les élus demandaient à juste titre l'exclusion de l'année 2021 qui a enregistré une baisse exceptionnelle de la CVAE. En raison de la crise sanitaire. Ainsi, Monsieur le Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement pour compenser la suppression de la CVAE sans porter atteinte aux finances des collectivités territoriales, je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Annick Jacquemet. S'il est un point sur lequel nous nous retrouvons je crois à toutes et tous, ici, sur les bancs. C'est la volonté de restaurer notre industrie et de retrouver une situation où nous créons des emplois industriels où nous ouvrons des usines en France, on est tous d'accord là-dessus. Ensuite il y a un débat sur les modalités d'y parvenir. Effectivement nous considérons qu'il faut baisser les impôts de production, comme nous l'avons fait et on voit de premiers résultats même s'il faut évidemment poursuivre et amplifier notre action, il y a eu ce débat et nous avons effectivement assumé de supprimer la CVAE. Et je suis absolument persuadé même que dans le choix de la majorité sénatoriale à l'époque de vouloir annuler la suppression de la CVAE. Il n'y avait pas le rejet de la baisse des impôts de production, mais des doutes, des inquiétudes sur la manière dont nous allions la compensée pour les collectivités locales effectivement la Première ministre a pris des engagements très clairs devant les associations d'élus et ses engagements ont été tenus par un euro de CVAE pour l'année 2023 n'gardé par l'État. Vous avez parlé d'une différence d'un Delta de 650 millions d'euros. Ils sont précisément versées aux fameux fonds Vert porté par Christophe Béchu et au SDIS 500 millions d'euros sur le pont va font verse 150 millions sur les SDIS. Au global, l'écrasante majorité des collectivités voir leur CVAE en 2023 progressé par rapport à 2022. C'est notamment le cas chez vous dans le Doubs. J'ai regardé j'avais regardé la proposition faite par l'AMF de retraités. L'année 2021 du calcul de la moyenne, mais il y aura eu 45% des EPCI et 40% des communes qui auraient été perdante. La réalité c'est que prendre une moyenne sur plusieurs années. Ça permet de lisser une grande volatilité comme vous l'avez dit, avec des communes qui peuvent se retrouver sur une année avec un trou, sans évidemment avoir aucune responsabilité. Je crois que le choix que nous avons fait et protecteur pour les collectivités, les engagements de la Première ministre permettent d'assurer que l'État ne garde rien de la CVAE collecter et que tout est reversée aux collectivités locales évidemment dans le travail qui va se poursuivre avec elle sur la poursuite de la définition des modalités de compensation, on continuera à avancer avec vous. avec les questions au gouvernement, prochaine. Question d'actualité, le 12 avril à 15h, la séance va être suspendu. Elle sera reprise à 16h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à favoriser l'accès de tous les étudiants, une offre de restauration. Tarif modéré. La séance est suspendue.

La séance est reprise. Madame la Ministre. Mes chers collègues. J'ai le plaisir de saluer dans la tribune d'honneur, une délégation de parlementaires canadiens conduite par Madame Marie-France Lalonde, présidente de l'Association interparlementaire Canada-France. Ils sont accompagnés par notre collègue Monsieur Yan Chantrel. Président du groupe d'amitié France-Canada. La délégation est arrivée en France, le premier avril pour une visite d'étude consacrée aux politiques environnementales et culturelles. Ces travaux porteront particulier sur l'action de la France pour le développement des énergies renouvelables. Après avoir visité ce matin le chantier du village olympique à Saint-Ouen. La délégation va poursuivre sa mission en Normandie. Le sénat français entretient d'excellentes relations avec le Parlement du Canada. Ces rapports de confiance et d'amitié sont à l'image du partenariat d'exception qui unit nos 2 pays. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du Parlement du Canada la plus cordiale bienvenue ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est parvenu à l'adoption d'un texte commun. J'informe également le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et en fonctionnement des installations existantes ont été publiés. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion en 2ème lecture de la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarifs modérés. Et dans la discussion générale. La parole est à madame Sylvie Retailleau Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est à vous, madame la Ministre. Merci Merci madame la présidente. Monsieur le président, la font. Monsieur le rapporteur agréer. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs. Alors nous sommes réunis cet après-midi pour l'examen de la proposition de loi du sénateur Pierre-Antoine Levi visant à favoriser l'accès à tous les étudiants à cette offre à une offre de restauration à tarif modéré. Dans plus de la moitié des communes dites en zone blanche, le nombre d'étudiants n'excède pas la centaine. Le modèle des Crous et donc difficilement mobilisables dans ces conditions et il nous faut donc effectivement nous appuyer sur des acteurs déjà en présence, c'est le sens de la restauration agréé par les Crous, plus de 170 acteurs publics comme privés ont pris, ont pris part à une convention pour étendre leurs services pour un public étudiant. Pour les facilités. J'ai souhaité renforcer les moyens consacrés et la loi de finances initiale pour 2023, a relevé de 33% les crédits prévus pour permettre le développement de ces conventions. C'est aussi en ce sens que j'avais porté lors de l'examen du projet de loi de finances 2023. Votre proposition visant à permettre au Crous d'ouvrir leurs centrales d'achat à d'autres acteurs et que le Sénat a adopté une contrepartie à cette ouverture était bien sûr de contribuer à l'accès à la restauration pour des étudiants à tarification sociale. Cela peut constituer un bon levier pour engager des acteurs à renforcer leur activité tout en faisant des économies d'échelle, à la fois dans leur intérêt comme dans celui du réseau social des heures des Oeuvres universitaires et bien sûr toujours au bénéfice des étudiants pour autant dans certaines communes ciblées. Il apparaît qu'aucun acteur ne souhaite s'engager dans une démarche de conventionnement de ce type, il nous faut donc encore trouver d'autres leviers. Et c'est là que je mesure l'intérêt de la proposition si de loi du sénateur Lévy après les évolutions du travail parlementaire en première lecture. Vous proposer aux étudiants un dispositif spécifique leur permettant de régler l'achat d'un repas à tarification. Auprès d'un acteur faisant l'objet d'une forme de conventions de partenariat, c'est une autre logique qui contribuent à renforcer les outils à notre disposition. Je suis attaché comme vous à ce que nous trouvions des solutions collectives plutôt que des solutions individuelles pour répondre à une ambition que nous partageons, permettre à chaque étudiant de déjeuner d'un repas complet à proximité de son lieu d'études et à tarification. Pour autant, votre proposition de loi soulève des questions concernant sa mise en oeuvre sur lesquels mes services sont actuellement pleinement mobilisés afin de la rendre opérationnelle. Si elle devait être adoptée aujourd'hui et pour qu'elle rentre en vigueur le plus rapidement possible et si possible à la rentrée. C'est absolument essentiel pour éviter par exemple une inflation des prix de la restauration étudiante à proximité des lieux d'études concernées, soit par effet d'aubaine qui serait préjudiciable, tant pour les étudiants que pour les finances publiques. Vous le savez, le gouvernement est pleinement engagé aux côtés des étudiants. Cette mesure viendrait utilement compléter les nombreuses autres mesures mises en oeuvre depuis ma prise de fonction. Permettez-moi de rappeler quelques éléments concourant à l'amélioration des conditions de vie étudiantes, auquel on tient tous l'été dernier j'ai annoncé des mesures d'urgence visant à préserver leur pouvoir d'achat le 7 octobre dernier jeu lancé à la demande de la Première ministre. Une large concertation sur la vie étudiante dans toutes ses composantes, les bourses bien sûr mais aussi la restauration sujet qui nous réunit aujourd'hui ou encore le logement, l'accès au sport, à la santé ou bien encore à la culture. Sur le sujet spécifique des bourses. Le constat était clair et partagé notre système sur critères sociaux qui est efficace et distributive présenté aujourd'hui certaines limites. Conformément aux orientations du président de la République qui avait inscrit ce chantier dans la feuille de route de son second quinquennat. Une attention particulière devait lui être accordée afin que le coût de la vie ne soit jamais une barrière aux études, des études J'avais donc dressé à la fois une méthode mais aussi un calendrier clair et j'ai eu l'occasion de présenter devant la commission de la culture avec une première étape présentant des annonces pour la rentrée prochaine et une seconde étape à l'été pour donner les contours d'un modèle cibles. La semaine dernière, j'ai donc annoncé cette première étape de la réforme des bourses qui représente un engagement d'un demi-milliard d'euros. Ces annonces sont également une réponse aux préoccupations liées au pouvoir d'achat étudiant et aussi à leur accès à la restauration pour la prochaine rentrée. Cette première étape de la réforme cibles 3 objectifs principaux et des plus d'étudiants. Et des mieux tous les étudiants en revalorisant toutes les bourses et neutraliser ces fameux effet de seuil. 35.000 étudiants vont donc devenir boursier nouveaux boursiers alors qu'il n'aurait pas bénéficié de cet accompagnement si les paramètres demeuré inchangé le montant des bourses augmenteront d'un montant de 37 et et euros pardon pour tous les échelons et cela correspond à environ une augmentation de 34% pour le premier échelon et une augmentation à hauteur de l'inflation pour l'échelon le plus élevé. C'est la plus forte revalorisation depuis 10 ans et elle concerne cette fois tous les étudiants boursiers nous permettons aussi à 140.000 boursiers actuels, soit environ 20% du nombre total de boursiers de basculer à un échelon de bourse supérieure en tenant mieux compte de leur situation familiale. Cela représente une augmentation entre 66 euros par mois jusqu'à 127 euros par mois, c'est plus de boursiers reclasser que lors de toutes les précédentes réformes enfin nous neutralisant dès cette année ses effets de seuil. En attendant de les supprimer de manière pérenne ainsi à la rentrée 2023 aucun étudiant ne verra sa bourse diminué d'un montant supérieur à l'augmentation des revenus de ses parents. En complément, j'ai aussi annoncé la pérennisation d'une tarification très social des repas pour les boursiers et pour les étudiants précaires. Cela dit, pour tous les étudiants c'est tarification de la restauration seront gelés pour la rentrée prochaine, à 3 euros 30 et aussi à un euro pour le tarif très social. De même que les loyers pour les résidences Crous mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. Nous sommes tous donc mobilisés pour accompagner les étudiants pour leur garantir de bonnes conditions à la fois de vie et d'études. Nous savons que les ces dernières années n'ont pas été facile particulièrement pour notre jeunesse. Nous avons besoin de tous les outils et de toutes les bonnes volontés, ainsi que de toute la souplesse possible pour pouvoir apporter des réponses à tous les étudiants sur tous les territoires pour ces raisons et parce que nous poursuivons ce même objectif je serai amené à émettre un avis favorable à l'adoption de votre proposition de loi, sous réserve bien sûr que sa mesure principale ne soit pas des des des dénaturé et croyez bien que nous ferons tous les efforts pour la mettre en oeuvre au plus tôt. Je vous remercie. remercie. Mais. La. La parole est à monsieur Jean Angry rapporteur de la commission de la culture de l'éducation et de la communication pour 10 minutes.

mon binôme Pierre-Antoine Levi, qui est à l'initiative de ce texte. Une initiative que nous portons avec le le groupe centriste, et le Sénat depuis mars 2021 qui a été et l'objet d'une grande pugnace cité d'un combat de chaque instant de ce que nous faisons aussi suite à l'excellent rapport du président là font hein de notre ami. Pierre Ouzoulias ce qu'ils. Faisaient dans leurs recommandations. Aussi. Qui allait dans le sens des recommandations. Du sénateur Lafont et de Pierre Ouzoulias pour mettre en place ce repas à tarif modéré sur l'ensemble du territoire et c'est ce que nous voulons. Mettre en place aujourd'hui Madame la Ministre faire voter conforme ce texte. Qui est passé à l'Assemblée nationale, certes avec quelques modifications parce que nous étions partis sur l'idée. D'un ticket restaurant étudiant dans laquelle. L'État rajouter 3 euros 30 ou 3 euros 30, que les étudiants non boursiers devaient verser pour s'alimenter, puisque nous avons. Toutes et toutes été marquée par ces files d'attente des étudiants au moment de la crise sanitaire. Des files d'attente de parfois de plusieurs centaines de mètres, voire de kilomètres et qui nous ont qui est clairement heurté. Alors nous avons. Au cours de la crise Covid. Nous vous avions interpellée pour le repas, 1 euros pour les boursiers, vous l'avez mis en place. Avec le gouvernement. Vous venez de de le redire, contrairement à ce que nous pouvons lire ici ou là dans la presse, il sera toujours. Maintenue aujourd'hui, nous vous proposons l'élargissement d'un conventionnement déconventionnement qui peuvent exister ici ou là dans à peu près. De 100 lieu et c'est la généralisation de ces conventionnement qui vont permettre aux étudiants de pouvoir soit déjeuner à un euro pour les étudiants boursiers. 3 euros 30 pour les étudiants non boursiers et cela dans des institutions publiques Par exemple le cas pour les hôpitaux, nos mairies ou encore des épiceries sociales et solidaires et aussi et nous le. Tenons particulièrement cela à des restaurants privés que dans certains territoires, vous l'avez dit, c'est l'objet de notre de notre PPL aujourd'hui il n'y a pas de restauration universitaire et donc les étudiants ne sont pas sur un, un pied d'égalité. Quand vous êtes jeune. Étudiant ou apprenti dans un territoire. Rural. Vous n'avez pas forcément accès. À cette restauration qui vous permet de vous nourrir dans de bonnes conditions. Nous l'avions de nous l'avions dit avec Pierre-Antoine lors de la première lecture de ce texte nous tenons particulièrement à l'action des Crous, l'autre objet n'était pas de remettre en cause l'action des coups d'écrous, ce qui fait vraiment. Du bon, du bon travail, il y a encore pas si longtemps que ça, que j'étais étudiant et que je pouvais aller. Déjeuner. Au restaurant universitaire et nous saluons naturellement toutes les personnes qui sont engagés dans la restauration universitaire et qui permettent à nos étudiants de déjeuner dignement. Chaque jour il y a aussi une hypothèse de travail qui est mis en place dans cette, dans cette PPL et qui je pense Va intéresser. Plus particulièrement certains de nos collègues, le fait que l'État finance directement. Les repas avec une aide sociale directe. Je pense que c'était une hypothèse de travail qui complète les autres hypothèses et c'est le décret d'application et les débats qui continueront après le vote conforme de cette loi aujourd'hui au Sénat qui permettra de voir si les différentes hypothèses. Sont maintenus ou pas dans le décret d'application. Nous continuerons entre guillemets le combat avec notre collègue Pierre-Antoine Laurent Lafon pour que les différentes hypothèses soit approfondi et mis en place naturellement avec votre accord et avec l'accord madame, la Première ministre et du président de de la République. Concernant aussi les améliorations qui avait été apportée par l'Assemblée nationale il y a un rapport annuel qui permettra aux parlementaires, que ça soit l'Assemblée nationale ou au Sénat, de pouvoir avoir accès aux différents conventionnement qui seront mis en place en partenariat avec les Crous et cela. Par la même nous mettons en exergue donc l'action des Crous, mais aussi avec. Un échelon elle nous tenons particulièrement est l'échelon territorial puisque l'action publique doit aussi se dérouler de manière concrète à l'échelle de nos territoires. Nous sommes. Particulièrement fiers et heureux de porter cette loi, les groupes votent de la même manière, avec nos collègues, nos collègues votent de la même manière qu'en commission il trouvera un écho favorable de la part des différents groupes. Au Sénat et nous espérons même que certains puissent passer d'une abstention bienveillante à un vote pour, parce que nous pensons que ce texte ces Oeuvres d'une justice sociale pour l'ensemble des étudiants de notre territoire, en tout cas Madame la Ministre nous tenions à vous remercier, avec l'ensemble des des collègues pour cette avancée majeure que constitue ce texte pour les étudiants dans les différents dans les différents territoires et c'est bien au Sénat que nous défendons les territoires parce que notre chambre en est issu. En tout cas merci et j'attends. Nous attendons de pied ferme les avis des différents. Personnes qui vont intervenir pour pouvoir voter ce texte de manière conforme malgré 2 amendements qui ont pu être déposée. Je vous remercie. Merci cher collègue. Alors dans la suite de la discussion générale là. Parole est à monsieur Julien Bargeton pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la Ministre, en effet, notre groupe avait en première lecture il y a 2 ans émis. Une abstention bienveillante. Nous craignons en effet que le texte remettent en cause un service public qui est celui des Crous et auquel nous sommes très attachés parce que aujourd'hui c'est le CROUS qui assure ce service et qui repère d'ailleurs dans les zones blanches. ce qu'il faut pour que on puisse conventionnée ou donner un agrément et c'est comme ça qu'il y a 180 structure à peu près la musique vous l'avez dit, qui ont reçu un agrément donc nous sommes très attachés au Crous d'autant plus que pendant la période du Covid. Ils ont joué un rôle fondamental, lorsque

à un euro d'abord aux boursiers et puis ensuite ça a été étendue à tous les étudiants, y compris étrangers. Donc on voit la force de frappe aussi des Crous, à ce moment-là. Et enfin je rappelle qu'ils ont beaucoup évolué, puisqu'ils ont mis en oeuvre. Le click and collect la livraison la commande. Enfin voilà il y a eu une modernisation des des cross donc. Pour cette raison là notre volonté de défendre ce service public. Nous nous étions. Attentifs à ce qu'qui pouvaient être les conséquences de ce texte, il se trouve qu'il a beaucoup évolué depuis cette première lecture, d'abord parce que notre commission a territorialisée le dispositif en disant que c'était là où il y avait un manque on pouvait et finalement trouver une autre solution telle que vous la proposiez. Ensuite parce que à l'Assemblée il y a eu. Beaucoup de changements. Le rappel de l'universalité de l'accès des étudiants à la restauration universitaire ensuite le rappelle qu'il y a une priorité à la restauration collective, avec les Crous mais qui sont avec une possibilité d'agrément et de conventionnement. En en complément mais bien en complément et puis. L'idée de remplacer le ticket restaurant enfin le ticket telle qui avait été créé par une aide financière qui permet de mieux cibler selon nous le dispositif. de cette territorialisation qui avait été apportée dans un 1er temps par notre commission ici au Sénat, par les trois évolutions apportées par l'Assemblée nationale, hé bien notre groupe votera favorablement à ce texte, tel qu'il est issu de ce débat constructif entre. Nos deux chambres parce qu'il permet d'assurer un certain dispositifs qui nous paraît clair et cohérent, cependant il y a, il reste quelques questions quand même qui sont pendantes. Première question, vous l'avez cité Madame la Ministre c'est celle de l'effet prix on sait que parfois quand il inversement vous savez que c'est le débat qu'on a aussi avec les APL dans d'autres dans d'autres discussions au moment de la la débat budgétaire ou dans d'autres commissions. Est-ce que ça a un effet prix, c'est-à-dire que, au fond, il ne faut pas que ça crée finalement ensuite la deuxième question c'est la condition. De. Ce versement hein comment sous quelles. Conditions il va être versé et puis la 3ème question c'est l'appréciation de la proximité. Quand est-ce qu'il y a vraiment un besoin comment on va identifier et caetera, bon il y a un certain nombre de questions qui reste posée mais pour autant, si des interrogations subsistent. Il nous semble que désormais le texte va dans le bon sens et nous nous félicitons de l'accord ainsi trouver et c'est pourquoi notre groupe votera en sa faveur. Je vous remercie. Merci la parole est à madame Sabine Vanek pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes. Madame la présidente. Madame la Ministre, Monsieur le président de commission. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en 2ème lecture la proposition de loi visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarifs modérés et je tiens à remercier notre rapporteur pour la qualité de son travail. L'idée initiale de cette PPL lors de sa première lecture au Sénat en juin à 21 et de créer un ticket-restaurant étudiant. Sur le modèle de ce que les entreprises propose aux salariés. Outre le questionnement sur son financement, sur le risque d'un repli sur soi et d'une alimentation déséquilibrée, nous avions insisté sur les dangers que ça tpl faisait courir au Crous en les affaiblissant dans leur mission de restauration qui rentre, qui représente 30% de leur chiffre d'affaires, ainsi que dans leurs autres missions à caractère social. L'Assemblée nationale dans sa réécriture a proposé un 2ème système de conventionnement l'avec les Crous pour les structures proposant directement une offre à tarif modéré similaire à celle des restos U. Et l'autre de conventionnement avec les Crous les établissements ou les collectivités pour les structures dans lesquelles les étudiants pourront s'acheter un repas grâce à l'aide financière octroyée lorsque l'offre de restauration à tarifs modérés sera défaillante dans le territoire. La réécriture par l'Assemblée nationale, opère un changement total de raisonnement. Nous ne parlons plus de tickets restaurant. Mais cette solution n'est pour nous pas encore tout à fait satisfaisante complexifie le système en l'encadrant de façon insuffisante selon qu'une offre de restauration à tarifs dits modérés existe ou non localement. Le dispositif du premier alinéa de l'article impose le postulat de départ que dans chaque territoire existe une possibilité pour les étudiants de bénéficier d'une offre de restauration à tarifs modérés et à proximité du lieu d'études. Il s'agit d'abord d'une simple possibilité et il faudra un meilleur encadrement des notions de territoires de tarif modéré et de proximité du lieu d'études. Le dispositif du 3ème alinéa de l'article 1 prévoit que lorsque l'offre n'existe pas une aide financière et proposer aux étudiants concernés pour permettre l'acquisition de tout ou partie du prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'un organisme conventionné. Il n'est donc plus fait allusion en tickets restaurant, on l'a dit, mais cette fois on ne connaît ni la forme ni le montant de l'aide accordée aux étudiants éloignés de territoires avec sa réécriture. L'assemblée nationale donne au service public de l'enseignement supérieur, un rôle prépondérant dans le service d'être mais le flou entoure encore la rédaction du dispositif par ailleurs non contraignant accès à une restauration à tarif modéré pour des étudiants sur des territoires non défini le double système de conventionnement, selon que cette offre à tarif modéré existe ou non n'apporte donc aucune véritable garantie supplémentaire par rapport au texte adopté en première lecture au Sénat. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale peuvent générer un petit plus pour les étudiants. Même si le nouveau dispositif ne nous rassure pas tout à fait il est complexe, avec la crainte de son inefficacité pour apporter une aide concrète pourtant impérative à notre jeunesse étudiante en proie à des difficultés pour seulement satisfaire le besoin vital de se nourrir. C'est pourquoi les sénateurs socialistes, écologistes et républicains soutiennent le ticket resto U à un euro pour tous les étudiants dispositif simple et efficace. Débattu à l'Assemblée nationale le mois dernier grâce à une proposition de loi des députés socialistes et apparentés. Cette mesure de bon sens a hélas été rejetée par les députés de la majorité de droite sous prétexte que les fils de millionnaire pourrait profiter des repas à un euro. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'de de millionnaires dans les sites d'attente. De distribution alimentaire. Notre pays ne doit pas sacrifier sa jeunesse éprouvée par 2 ans de Covid de Covid pardon et attention à ne pas provoquer la colère ou le désespoir des jeunes qui se verraient priver d'études et d'avenir du fait de conditions d'existence trop précaire. En tout état de cause, aucune avancée même minime ne pouvant être négligé. Le groupe des sénateurs socialistes écologistes républicains. Maintiendront leur positionnement sur une une abstention bienveillante sur cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Les universités françaises souffrent depuis trop longtemps d'un manque chronique d'investissements. Elles ont dû accueillir toujours plus d'étudiants avec des moyens budgétaires limitées, les disparités entre les établissements, les mieux dotés situé dans les métropoles et ce moins bien financé des villes moyennes n'ont cessé de s'accroître notre pays ne pourra pas affronter les défis majeurs de notre temps, comme ceux de la décarbonation de la réindustrialisation ou de la restauration de la confiance en la science si nous ne faisons pas de la connaissance une priorité de nos politiques publiques. Les universités doivent devenir les outils essentiels au service de la nation prenantes afin de rendre la raison populaire pour reprendre les expressions de Condorcet. Ce large dessins impose entre autres choses, de favoriser la Russie des étudiants, mais aussi de soutenir l'accès à l'université des publics qui en sont les plus éloignés, pour des raisons sociales ou géographiques. Ainsi le récent rapport de la Cour des comptes examinés par notre commission la semaine dernière a montré que le taux de diplomation décroît. En fonction de l'éloignement aux universités. À la suite du rapport du président là font sur la vie étudiante, je me félicite que nous partagions aujourd'hui l'idée que l'université doit redevenir un instrument indispensable de l'aménagement du territoire. Pour des raisons budgétaires mais aussi fonctionnel les politiques en faveur de l'université ne peuvent être conçu et mis en oeuvre sans une collaboration active avec les collectivités. Le logement, la restauration, la santé, les transports, l'emploi sont des domaines pour lesquels les interactions avec les collectivités seront décisives pour offrir aux étudiants un environnement favorable à leur réussite pédagogique.

en permettant à ces dernières d'accéder à sa centrale d'achat et en relançant la politique de conventionnement entre ses partenaires. Un amendement du gouvernement, la loi de finances pour 2023, a satisfait le premier objectif en introduisant l'Arctique L du code de l'éducation. Une disposition qui permet au Cnous d'exercer les missions d'une centrale d'achat au bénéfice des collectivités et des établissement publics. La présente, proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale et après la levée du gage financier par le gouvernement complète cet article du code de l'éducation est inscrit dans la loi la possibilité d'un conventionnement entre le que nous et les collectivités pour permettre aux étudiants l'accès à une offre de restauration publique alternatif. Il faudra Madame la Ministre donner au Cnous les moyens budgétaires de satisfaire ce nouveau service. Notre ambition collective et maintenant que tous les étudiants puissent avoir accès la restauration publique dès la rentrée de septembre prochain. Il faut redire ici combien les actions du que nous c'est des Crous ont été décisive pour aider les étudiants lors de la pandémie, la capacité d'innovation de ce réseau et la façon dont il a pu mobiliser des ressources supplémentaires et les décliner en fonction des particularités locales ont montré toute l'utilité d'un organisme national travaillant en bonne Intelligence avec toutes les universités. Un nouvel élan aujourd'hui doit lui être donnée par une politique ambitieuse et nouvelle de collaboration avec les collectivités. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre-Antoine Levi. Pour le groupe Union centriste pour six minutes. Madame Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur chargé en Hongrie. Monsieur le président de la commission de la culture. Cher Laurent Lafon, mes chers collègues. Le 3 mars 2021. Il y a déjà 2 ans, j'ai déposé une proposition de loi visant à créer un ticket-restaurant étudiant. Je dispositif répondait à une attente importante de nombreux des étudiants, notamment ceux qui se trouvaient dans les zones blanches moins bien ou pas du tout desservies par les dispositifs du Crous. Les zones blanches désigne des régions où il n'y a pas de structure de restauration universitaire à proximité, obligeant les étudiants à parcourir des distances souvent longue pour se restaurer un tarif abordable. Face à la crise de la Covid 19 qui a aggravé la précarité étudiante, avec des images bouleversantes de jeunes faisant la queue lors de distributions alimentaires caritative. Cette proposition de loi, cosignée par 82 sénateur de 3 groupes politiques différents. Visait à apporter une solution concrète et rapide. Un problème réel. La pandémie a accentué les inégalités sociales et a rendu les conditions de vie des étudiants encore plus difficile notamment en terme de logement. D'accès à l'éducation et de santé mentale. Je tiens à remercier mes collègues du union centriste qui ont accepté d'inscrire cette proposition de loi dans notre niche parlementaire de ce jour. Oui, mes chers collègues, nous avons progressé il nous sommes proches de notre objectif, créer un dispositif permettant à près de 500.000 étudiants d'avoir accès à une restauration à tarif modérés, comme c'est le cas dans les grands centres universitaires. L'accès à une alimentation saine et abordable est essentiel pour le bien-être et la réussite académique des étudiants. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce principe. Lors de l'examen par l'Assemblée nationale, le texte a évolué. L'ancienne majorité et le gouvernement n'ont pas souhaité conserver le dispositif initial, préférant miser sur l'Europe à un euro. Une mesure louable en soi. Cette mesure bien que bénéfique pour les étudiants ayant accès à un restaurant universitaire ne répondait pas à la problématique des zones blanches. Les étudiants sans accès un restaurant du Crous ne pouvait de toute façon pas profiter des repas à un euro, les laissant dans une situation extrêmement précaire. J'ai interpellé à plusieurs reprises, l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ce sujet en lui demandant de trouver des solutions, malheureusement sans succès. Je salue. Par contre l'action volontaire de Sylvie Retailleau sa successeure et notre dialogue commun pour chercher et trouver des solutions. La collaboration entre les différentes instances politiques est essentielle pour résoudre les dit problèmes auxquels sont confrontés les étudiants. Aujourd'hui le texte que nous examinons est différent. Au fil de nos travaux en commission et de la navette parlementaire cette proposition de loi évoluer. Certains pourraient penser qu'elle ne va pas assez loin, ou que le dispositif initial et dénaturé. Je trouvais un titre personnel assez simple et facile à mettre en oeuvre une proposition de création d'un ticket-restaurant étudiant. Mais mes chers collègues, je crois qu'il faut savoir penser à l'intérêt de nos étudiants. Et d'éviter une nouvelle navette vers l'Assemblée nationale si nous votions pas ce texte conforme. Il faut se satisfaire de victoire, quelle qu'elle soit lorsque nous en avons l'occasion. Le compromis atteint apportera des améliorations significatives à la situation des étudiants en difficulté. Notre objectif est bien n'est-ce pas, d'améliorer la vie des étudiants qui s'est compliqué depuis la crise de la Covid 19. Et maintenant la crise de l'inflation. La hausse des prix affectent tous les aspects de la vie quotidienne, y compris le coût de la nourriture, rendant encore plus difficile l'accès à une alimentation équilibrée pour les étudiants en situation de précarité. Une partie des critiques émises par certaines de collecte de nos groupes, des groupes politiques résider dans le risque qu'il percevait d'affaiblissement des Crous, avec la mise en place du ticket-restaurant étudiant il craignait que l'instauration de ce dispositif ne détourne les étudiants des structures existantes et n'entraîne à terme une diminution des ressources pour les Crous. Bien que je ne partirai chauffage cette inquiétude qu'ils soient rassurés. Le dispositif actuel sera organisé autour des Crous. Via des conventions avec des structures de restauration qu'elle soit publiques comme les cuisines centrales de mairie d'hôpital par exemple ou privés comme des restaurants ou des restaurants d'entreprise. Ce partenariat permettra de soutenir les Crous tout en offrant des alternatives pour les étudiants dans les zones blanches et s'il n'y a pas de possibilité de conventionner hé bien les étudiants pourront éventuellement se voir verser une aide financière pour se restaurer. C'est un des dispositifs prévus par cette proposition de loi. Cette mesure permettra jusqu'à 500.000 étudiants de paix bénéficier d'un tarif modéré pour pouvoir manger. L'essentiel c'est bien cela. Nous ne pouvons pas dire que cette mesure coûte cher car il s'agit ni plus ni moins que du rétablissement d'une égalité sur un droit existant mais simplement non exercer en raison de l'absence de restaurant universitaire. J'espère que le Sénat votera très largement en faveur de cette proposition de loi il adoptera conforme. La prochaine étape sera sa promulgation rapide et l'écriture des décrets d'application. J'ai bien noté Madame la Ministre votre volonté de nous associer à cette écriture je vous en remercie très sincèrement. Avant de conclure, je tiens à remercier tout particulièrement mon collègue et mis en Hongrie pour son implication sur cette proposition de loi. Et bien évidemment Laurent Lafon, président de la commission culture pour son aide et ses précieux conseils et en fait un soleil Rieffel administratrice pour la qualité de son travail. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe de l'Union centriste voterait unanimement en faveur de cette proposition de loi, il était temps d'agir pour soutenir nos étudiants et leur offrir enfin des conditions de vie plus décente. Ce texte, c'est une première étape, il y a encore beaucoup à faire pour que nos chers étudiants n'est qu'un seul objectif, se concentrer et réussir leurs études, ils peuvent compter sur mon engagement le plus total. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame. Esther Benbassa pour 3 minutes.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs l'erreur les rapporteurs, mes chers collègues, le 29 mars dernier, le gouvernement a annoncé les premières mesures de sa réforme des bourses qui promet une revalide revalorisation générale historique 35.000 étudiants issus de la classe moyenne rejoignent le système des bourses et 37 euros supplémentaires pour tous les échelons. tout cela paraît bien beau mais suffisant pour corriger les inégalités et pallier les mauvaises conditions de vie des étudiants. Nous nous étions promis de ne pas nous habitués aux files d'attente interminables d'étudiants devant les points de distribution d'aide alimentaire. Payer son loyer ou manger télé souvent la question. Pour certains, selon l'Observatoire du SAMU social, un quart des étudiants présents à l'aide alimentaire, déclare un état de enfin modérée à sévère. Un état dépressif majeur pour pour un tiers d'entre eux Madame la Ministre comment réussir ses études quand on arrive même plus à se nourrir correctement. Aujourd'hui, nous discutons en seconde lecture d'un texte qui permet l'accès à tous les étudiants du nord de restauration à tarifs modérés ainsi s'il n'y a pas de restaurant Cruz une aide financière. Compensera ce manque certes il y a de réelles disparités selon les régions. Toutefois cette PPL ne précise pas les modalités de mise en place de cette contribution financière et on ignore également le montant de cette somme. Le texte connaît des limites et aurait pu être plus ambitieux. Dans un pays où il attend du milliardaire. Pourtant, le 9 février dernier, le Parti socialiste avait proposé à l'Assemblée nationale. Le repas à un euro pour tous les étudiants. La droite et la majorité présidentielle avait fait le choix de voter contre en prétextant préféré réserver ce dispositif à ceux qui en ont le plus besoin, nous, y a-t-il pas une contradiction flagrante et incompréhensible en cette PPL qui souhaite favoriser l'accès à tous les étudiants à une offre de restauration à tarifs modérés et votre rejet du repas Cruz à un euro pour tous. Difficile de voter contre un tel texte, je m'abstiendrai avec le souhait qu'un projet de loi plus complet, plus en 2. Ambitieux, voit le jour. Nos étudiants le mérite pour finir j'aimerais citer le communard Eugène Varlin, qui disait, tant que l'homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorgent. Il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. Merci. Je passe la parole à Monsieur Bernard s'il a l'air pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes. madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Le mérite de cette proposition de loi, c'est de mettre le doigt sur un véritable problème, celui de la précarité étudiante. Plus qu'une nécessité, c'est un devoir et je salue les annonces que vous venez de nous faire en direction des étudiants. Parce que si la crise sanitaire a aggravé cette précarité et accentuer les inégalités au sein d'une population étudiante très hétérogène. Elle a aussi révélé les failles structurelles de la restauration universitaire. Maillage territorial de l'offre insuffisant excluant les étudiants effectuant leurs études sur des sites. Délai d'attente décourageant et plages d'ouverture inadaptée modèle économique intrinsèquement. Autant de raisons légitimes en au débat de ce jour qui doit servir de 1er pas vers un système français de restauration étudiante plus égalitaire, plus juste et plus vertueux. Notre chambre en première lecture a permis de centrer le débat sur un problème identifié comme essentielle. L'inégalité d'accès des étudiants au service public de la restauration universitaire selon où ils se trouvent sur le territoire de la République. Cette anomalie rappel des rappellent celles déjà mises en lumière par le rapport d'information que nous avions rendu avec Céline Boulay-Espéronnier sur la CV c'est. Cette dernière finançant chaque année des Crous à hauteur de 40 millions d'euros ne permet pas à certains étudiants pourtant assujettis à sa contribution de bénéficier des services et actions finance. La territorialisation du dispositif Fabius et les modalités de sa mise en oeuvre modifié par l'Assemblée nationale. Il n'est plus question de tickets restaurant mais d'une aide financière ainsi que donc conventionnement. L'objectif étant de soutenir l'action des Crous en confortant et encourageant la possibilité qu'ils ont de conventionnés avec des acteurs publics tels que les collectivités territoriales, des acteurs privés et des acteurs sociaux. Parallèlement, l'aide financière versée aux étudiants n'ayant pas accès aux structures de restauration universitaire pourra prendre plusieurs formes et s'adapter aux besoins du terrain et aux solutions déjà existantes. Le groupe RDSE comprend la volonté de la Commission de voter un texte conformément à la rédaction issue des travaux de la chambre basse afin de ne pas repartir vers une navette à l'issue incertaine. Mais il ne peut occulter que sa réécriture par l'Assemblée nationale a opéré un changement de raisonnement et introduit une complexité inquiétante. Il ne faudrait pas que ce nouveau dispositif soit source d'inefficacité de manque de clarté et souffrent d'une insuffisance d'encadrement dans sa mise en oeuvre, notamment parce que l'aide financière. Et la politique de conventionnement du réseau des Oeuvres universitaires et scolaires reste à instruire à organiser et administrée par des services supplémentaires. N'hésitez pas Madame la Ministre a privilégié l'échelon local pour la mise en oeuvre de cette nouvelle aide financière en déléguant cette compétences aux métropoles ou aux régions déjà en charge d'une partie de l'enseignement supérieur avec les BTS ou les classes préparatoires. Les conventionnement existants avec les Crous sont encore insuffisants et il pourrait s'agir ici d'une chance de créer de recréer un lien multirisques rejet multi-générationnel entre les étudiants en zone blanche Crous et des établissements tels que des lycées ou des Ehpads. Par ailleurs ce dispositif territorialisée ne permet pas de résoudre certains problèmes structurels, liés aux délais d'attente décourageant les étudiants. Et aux plages d'ouverture journalière hebdomadaire et annuel inadaptés aux besoins des étudiants. Bon nombre d'étudiants pourtant présent sur des sites disposant de restaurant universitaire se retrouvent sans la possibilité de consommer une restauration à tarif modéré. Si l'uniformisation du repas à un euro n'est pas forcément synonyme d'égalité des droits. Faut compter il bien. Je. Territorialisée, le dispositif ne permet pas de résoudre toutes les sources d'innocuité face à l'accès et au droit à tous les étudiants et restauration à tarifs modérés en tout cas le groupe RDSE votera cette proposition de loi. Cependant ce vote sera même bilan. Si. Ça va vite. La parole est à monsieur Bruno Belin pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Madame la présidente Madame la Ministre, Monsieur le Président la font. Monsieur le rapporteur. Chers collègues d'abord dur d'entrée le soutien. De notre groupe à la proposition qui est présentée cet après-midi et remercié le président là font le rapporteur Jean engrais et Pierre-Antoine Levi pour le le travail qui vient d'être présenté. Mais même là la ministre notre collègue. L'éminent Pierre Ouzoulias. Ça a commencé son propos par ça par un état des universités. Et c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu se situer. Dans le cadre le contexte le quotidien et la réalité. D'abord les étudiants arrivent à l'université essoré par Parcoursup. Il faut déjà quand même pour l'avoir vécu certains comme parents. Exprimé la difficulté que ça représente. Et puis ils arrivent dans un cadre où là effectivement.

Il était grand temps de raser la faculté de Châtenay Malabry. Si vous voulez avoir un, un contexte où vous avez des étudiants qui ont envie d'étudier. Il faut quand même leur donner et le cadre nécessaire et les moyens parce que les moyens des universités, là encore, ça mériterait un grand débat. Avec notre collègue Yves Bouloux. On pourrait vous parler de la faculté de médecine de Poitiers si elle a été reconstruite. C'est uniquement par la volonté politique du président Monory et les fonds du Conseil général à l'époque, donc il faut absolument qu'on se préoccupe de l'avenir des universités parce que c'est quand même l'endroit où les étudiants étudient. Il faut que je vous ai dit le cadre il y a le contexte le contexte c'est une sortie de Covid qui a eu comme première conséquence d'isolement de tout le monde étudiant. Et puis effectivement cette inflation qui pèse à tous les étages de la vie étudiante pas que sur l'alimentation. Parce que le quotidien, il est là. Le quotidien c'est cette précarité. Alimentaire mais c'est aussi la question du logement du déplacement. C'est la nécessité pour. Une grosse moitié des étudiants, vous connaissez les chiffre comme moi de devoir travailler pour se payer leurs études. Et donc bien évidemment tout ça ne favorise pas actuellement. À cause de ce contexte et ce quotidien et puis il y a une autre réalité. Et pardon de prendre quelques secondes pour insister là-dessus, c'est la disparité là. Le mot effort fort discrimination territoriale. Parce que vous n'avez pas les mêmes chances et les mêmes accès aux services que vous avez présentée Madame la Ministre, que vous soyez. Milieu. Métropolitain urbain voir dans et ça. Certains établissements qui sont en milieux ruraux. Et donc ce dispositif, il faut aller y penser pour ça que soutien total à la proposition qui est faite, mais il faut peut-être l'élargir à d'autres volets. Moi je pense aux transports, à un moment donné on parle décarbonation mobilité. Je peux vous assurer que quand encore là vous êtes dans des territoires ruraux isolés on pénalise et évidemment on porte un poids un peu plus lourd sur les étudiants issus de ces territoires. Parce que en fait l'avenir de ce pays et c'est vrai depuis évidemment déjà quelques siècles et ça restera valable longtemps dépend évidemment du traitement que l'on portera nos étudiants parce qu'il porte l'avenir de la France, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à madame. Colette Mélot pour le groupe les indépendants pour 4 minutes. Madame le président. Madame la ministre, monsieur le président de la commission culture éducation monsieur le rapporteur cherche en engrais. Lors de la crise sanitaire relatives au Covid-19. Nous avions tous été. Par les images de longues files d'étudiants venus chercher un colis alimentaire. Aujourd'hui, l'édifice fait culté existe toujours en raison de l'inflation généralisée de la hausse du coût de l'alimentation avec l'impérieuse nécessité de soutenir les élèves de l'enseignement supérieur. nombreux sont les étudiants qui ne peuvent plus se permettre le même panier quotidien qu'auparavant. L'alimentation est devenue la première variable d'ajustement pour boucler les fins de mois. Dans ce contexte, toute aide destinée à leur permettre de poursuivre sereinement leurs études est la bienvenue. La hausse des bourses d'études. Annoncé la semaine dernière est également une excellente nouvelle. Antelme Bria Savarin écrivez dans sa célèbre Physiologie du goût que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. De la même manière la réussite universitaire de nos étudiants dépend aussi de la manière dont ils s'alimentent quoi de plus essentiel que de permettre à notre jeunesse de manger à sa faim. Voilà tout l'objet du texte que nous examinons aujourd'hui destiné à garantir à tous les étudiants l'accès à une offre de restauration abordable. En première lecture au Sénat, nous avions proposé la création d'une aide de territorialiser. Destiné aux étudiants qui réside à distance de restaurant universitaire. Je pense en particulier aux zones rurales et de montagne. Ces jeunes sont défavorisés puisqu'ils ne bénéficient pas de tarifs avantageux et des repas équilibrés fournis par ces fameux resto U. Depuis son dépôt au Sénat par notre collègue Pierre-Antoine Levi. Le texte a bien évolué et c'est peu de le dire. Permettez-moi d'un profit d'en profiter pour saluer son travail ainsi que celui de son rapporteur Jean Grey. Le projet de création d'un ticket-restaurant étudiant a été abandonné. Je ne peux que regretter la complexification du dispositif à l'issue de son examen à l'Assemblée nationale pour autant la philosophie du texte reste la bonne et cette nouvelle écriture va dans le bon sens. Cela explique son adoption conforme en commission. De son côté le gouvernement sera engagée à remettre chaque année au Parlement un bilan de la mise en oeuvre du dispositif, c'est une bonne chose. Nous serons particulièrement attentifs au retour d'expérience. En conclusion, le groupe les indépendants votera ce texte et se félicite du déploiement de dispositifs destiné à pallier les difficultés financières des étudiants. Merci, cher collègue, la parole est à madame Monique de Marco. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour quatre minutes. Madame la présidente, madame le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous elle. Amina aujourd'hui poursuit un objectif louable, celui de répondre à la précarité étudiante et à l'accès d'une offre de restauration et tarif modéré. Depuis le mois de mars 2021, au moment où notre collègue Pierre-Antoine Levi la rédiger. La situation n'a malheureusement pas évoluer. Je voudrais donc commencer par le remercier, ainsi que de groupe Union centriste pour l'inscription de cette proposition de loi dans leur niche. Mais la première version de tickets restaurant avait le mérite de plus de précisions. Aujourd'hui encore, 48% des étudiants sont contraints de travailler pour financer leurs études. L'inflation, l'inflation les oblige à recourir aux banques alimentaires pour se nourrir et les moins de 25 ans représentent un quart des bénéficiaires. Sur le campus de l'université de Bordeaux Montaigne 91% des étudiants vivent avec un budget inférieur. Au seuil de pauvreté, établi à 940 euros par mois. Face à situation Madame la Ministre la réponse du gouvernement, nous ne sommes pas à la hauteur. La revalorisation de 4% du montant des bourses à la rentrée 2022, soit 10,5 points en dessous de l'inflation des produits alimentaires s'est révélé insuffisante. Très rapidement, le gouvernement. Contraint de se rendre à l'évidence en prévoyant d'abord une aide exceptionnelle de 10 millions d'euros au mois de novembre dernier. Pour des colis alimentaires. Puis en ouvrant l'accessibilité à la mesure du repas à un euro aux étudiants non boursiers des plus précaires qui en feraient la demande. Le 23 mars dernier après la forte mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites. Vous avez Madame la Ministre débloquer une nouvelle enveloppe de 10 millions au type de l'aide alimentaire. 10 millions ce n'est pas grand chose quand on sait que 258 millions minimum serait nécessaire pour financer cette proposition de loi. De la même manière, l'annonce d'une enveloppe de 500 millions d'euros supplémentaires dévolus aux bourses pour la rentrée 2023 n'offre aucune garantie à long terme de sortir les étudiants de considérations financières qui les éloigne de leurs études. Il n'est donc pas acceptable que cette précarité soit gravée dans des territoires dépourvus de restaurants et de cafétérias universitaires à proximité des lieux d'études. Je voudrais particulièrement insisté sur la situation des étudiants ultramarins. Une récente note de l'UNEF a montré que le coût de la vie est supérieure de 26% pour les étudiants d'outre- mer comparé à ceux de la métropole. Il me semble incompréhensible également que pour ces derniers, des frais additionnels de 70 centimes leur soit appliqué au titre de frais d'emballage de transport. Cela double presque le reste à charge dans le cas dispositif à un euro. Comment justifier cette rupture d'égalité institutionnalisé. En première lecture nous avions souligné des limites du ticket restaurant, étudiants. Réduction de temps de sociabilité coût trop importante pour l'achat d'un ticket de pour les étudiants les plus précaires. Nous ne pouvons pas, se montre cependant nous enthousiasmer de la réécriture totale du texte de l'Assemblée nationale. L'instauration d'une aide financière non chiffrée à dossier un réseau d'organismes conventionnés est extrêmement vague. Nous amendement de précision. Qui visaient simplement à prévoir un reste à charge. Pour l'étudiant identique sur tout le territoire en resto U comme dans un organisme conventionné il à prévoir l'existence d'une offre dans la même commune que le lieu d'études ont été rejetées rejet pour. Irrecevabilité financière relève la faille d'd'une ambition budgétaire derrière des belles intentions affichées. Il n'est pas trop tard. Madame la ministre, monsieur le rapporteur de vous approprier ses propositions en cours de séance afin de répondre réellement aux difficultés des étudiants. Je me tiens à votre disposition. Sans cela, nous considérons qu'il s'agit plus que la avec la jeunesse, nous nous abstiendrons sous ce texte avec bienveillance pour saluer la bonne volonté de son auteur. Merci. La parole est à monsieur François Bonhomme. Pour le groupe. Les républicains pour cinq minutes.

Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Alors que notre pays c'est en fait une sortie de crise sanitaire. Et que les petits boulots faisaient leur retour. Nous espérions alors que la situation des étudiants quelque peu s'améliorer. Malheureusement, l'inflation est venue fragiliser la situation des jeunes. En effet, nombre d'étudiants rencontre de grandes difficultés à payer conjointement leurs loyers et leurs dépenses alimentaires. C'est le cas notamment des quelque 700.000 boursiers qui, pour l'année universitaire 2020. T1 2022 touché rappelons-le une aide allant de 103 euros mensuels et ce sur 10 mois à 573 euros par mois pour l'échelon le plus élevé, sans parler de la situation des jeunes issus de la classe moyenne qui sont juste au-dessus du seuil ouvrant au bénéfice d'une bourse bien souvent. Ces jeunes doivent renoncer à acheter de la nourriture et parfois même à se soigner. Ce qu'ont confirmé l'Observatoire de la vie étudiante en 2021, puisque 38% des étudiants déclaré s'être restreint sur leurs dépenses alimentaires foire hein venait à supprimer serait un repas. J'ajoute que l'aide auprès d'associations afin d'obtenir des paniers alimentaires gratuit ne suffit pas toujours. Et même si le gouvernement le RAC Torino leur a octroyé une rallonge budgétaire. Ponctuel de 10 millions d'euros ces associations n'arrive plus à répondre à la hausse continue de demandes. De même, l'augmentation des APL de 3,5% pour la rentrée 2023, celle de 35.000 boursiers supplémentaires ainsi qu'une revalorisation, programmée de 37 euros. Des bourses pour la rentrée prochaine ne suffit pas. C'est pourquoi un nouveau dispositif d'aide plus efficace et permanent. Permettant aux étudiants de pouvoir se nourrir correctement et dans des conditions financières acceptables et nécessaire. Je veux saluer ici le travail de notre collègue Pierre-Antoine Levi, qui a permis au Sénat puis à l'Assemblée nationale de se saisir de cette importante question de la précarité alimentaire étudiante. Il est parti du constat que l'actuel service public de la restauration universitaire été inégalement accessible inaccessible accessible sur notre territoire en effet selon l'endroit où ils font leurs études tous les étudiants n'ont pas accès. De la même manière un restaurant universitaire. C'est le cas notamment. Dans beaucoup de vie, de taille intermédiaire ou en zone rurale celle finalement de la France périphérique puisque les étudiants ne sont pas tous dans les universités il y a aussi tous ceux qui suivent des enseignements. Dans de nombreuses écoles de l'enseignement supérieur où il n'existe pas pour l'offre de restauration adaptée. Il s'agit donc de permettre aux étudiants de ces zones blanches de bénéficier d'un tarif préférentiel. Pour un repas comme ce serait le cas dans un restaurant dépendant d'un Crous ces propositions. Corrige cette inégalité et doit rétablir dans les faits le principe d'universalité pour tous les étudiants D'avoir droit à une offre de restauration de proximité un tarif social, c'est pour cela que le Sénat avait fort opportunément adopté ce texte qui ont constitué une véritable avancée. Le deuxième le débat en deuxième lecture porte essentiellement sur les modalités de de mise en place de ce nouveau dispositif. Pierre rentre le devis proposé la création d'un ticket-restaurant étudiant, pour tous ceux qui, suivant un enseignement supérieur dans les zones blanches en avait besoin. Ce chèque permettait à chacun de régler totalement ou partiellement le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'organismes, y compris des restaurants ayant noué une convention. Avec des acteurs territoriaux de la vie étudiante en particulier le réseau des Oeuvres universitaires et scolaires dans le rôle. Prépondérant pour sa part, l'Assemblée nationale a fait le choix en première lecture de remplacer le ticket restaurant par la création de par une aide alimentaire dans les critères d'attribution demeurent les mêmes que ceux votés par le Sénat. Le dispositif adopté par l'Assemblée permettait aussi d'avoir recours à de bons à des bons alimentaires qui seraient utilisable notamment dans les lieux conventionnés. En fait, il a été prévu chaque année la remise d'un rapport d'évaluation sur l'accès des étudiants à une offre de restauration à tarif modéré et de qualité cette évidemment une bonne disposition qu'il convient de soutenir. J'ajoute que le chèque restaurant étudiants paraissait novateur est plutôt simple d'utilisation pour sa part, l'Assemblée nationale a modifié sa disposition au profit d'une aide. Même si elle a conservé l'esprit initial diversité de la proportion de la proposition de loi de notre collègue Olivier qui malgré tout laisse quelques réserves entre ces 2 options. La commission de la culture au Sénat a donc tranché en adoptant conforme la rédaction issue des travaux de l'Assemblée. Le dispositif initial avait été positivement enrichi je me range donc à cet avis de la. Lors des débats, car il existe malgré tout je crois un point. De consensus sur l'agence de la situation ainsi que sur la nécessité d'obtenir rapidement un dispositif à la fois rapide et opérationnelle pour l'ensemble des étudiants. Il y a une urgence, je crois. Ainsi à répondre à une attente très forte de ceux-ci, nous espérons bien sûr Madame la Ministre que le gouvernement garantira le financement nécessaire. À la réalisation du projet. Nous espérons parce que la nation je crois doit faire n'effort d'investissement pour soutenir notre jeunesse étudiante. Toutes ces raisons pour lesquelles je voterai bien entendu ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors la discussion générale. Close. Nous passons à la discussion du texte de la commission et je vous avertis qu'il y aura un scrutin public sur l'ensemble du texte. Alors à l'article 1er oui un rappel au règlement. Oui, je voulais faire un rappel au règlement. Je vous remercie madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues. Mon rappel vise l'article 44 terre du règlement qui vous autorise Madame la Ministre monsieur le rapporteur, a proposé des amendements jusqu'en séance. Je vous appelle à faire application de ce droit afin de préciser le texte pour le rendre réellement applicable dans l'intérêt des étudiants 2 amendements que j'avais déposé ont été. Déclarés recevables je contexte ces irrégularités. Le texte retenu revenu de l'Assemblée nationale ne comporte aucun engagement précis se demandent, as de l'aide financière allouée aux étudiants vivant hors de la zone de restauration universitaire. Il faut une égalité stricte entre étudiants, quel que soit leur positionnement géographique sur le territoire, ils doivent tous pouvoir accéder au prix subventionné d'un euros ou trois euros 30 sur leur leurs moyens. Si le reste à charge un organisme conventionné. Est supérieur au prix d'un sandwich en boulangerie. Alors la proposition de loi me semble inutile. Qu'en pensez-vous. Dans le texte de l'Assemblée l'est également écrit que l'organisme conventionné devra se trouver à proximité du lieu des. Chers collègues

Alors à l'article. 1er je suis saisi d'un amendement numéro 4 de Madame de Marco. Et donc vous avez la parole, chers collègues. Donc voici un amendement qui est resté. Madame la présidente madame la mise mais sa collègue excusez-moi d'être ponctue pointilleuse mais je crois que la situation des étudiants dans le pays le nécessite. L'objet de cet amendement. Et de préciser le texte ou de le rapprocher de l'intention exprimée dans l'exposé des motifs. Et je le cite ici les restaurants universitaires et leurs horaires d'ouverture semble de moins en moins répondent aux attentes étudiants aujourd'hui est de moins en moins adaptées à leurs emplois du temps. Nous proposons donc de compléter l'article 1er en prévoyant que les horaires de restauration dans les réseaux du Crous et des organismes conventionnés soit soumis à la consultation des syndicats étudiants en fin de les adapter à leurs besoins. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. madame la présidente. Mes chers collègues. Madame la Ministre c'est un avis. Défavorable chers collègues de Marco, vous nous invitez. À déposer des amendements au cours de ce débat, nous nous l'avons dit avec Pierre-Antoine Levi que nous ne déposeront pas d'amendement pour voter conforme. Ce texte et nous émettons donc un avis défavorable. Ce que vous appelez à travers votre amendement et cette modification à un consensus au niveau des syndicats étudiants pour intervenir dans les choix d'horaires d'ouverture des Crous, mais c'est bien là l'objet d'un conventionnement c'est. Grâce à ce texte, c'est que le conventionnement se fasse en local directement et non pas par la loi et le changement de la loi. Ne permettrait pas de voter conforme ce texte donc c'est un avis défavorable bienveillant. Si l'avis du gouvernement. Madame la Ministre. Merci madame la présidente. Même avis que monsieur le rapporteur, que même si si. Alors je vais mettre aux voix donc l'amendement numéro 4 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté, je Mist ou voir l'article 1er qui est pour un contrat qui s'abstient. Il est donc adopté. À l'article 1er bis l'amendement numéro 3 même de Marco. Je vous remercie madame la présidente de madame la ministre, mes chers collègues, après son passable. À l'Assemblée nationale. L'article 1 bis de la proposition de loi prévoit un bilan gouvernemental annuel de l'accès à l'offre de restauration à tarifs modérés. Je propose d'étendre ce bilan au suivi de l'évolution de la précarité alimentaire en France pour les étudiants. Je connais la position du Sénat sur la multiplication des demandes de rapport. Mais dans ce cas précis cela est réellement justifiée. Cet amendement vise particulièrement annualisé ce suivi alors que la crise alimentaire étudiante a atteint son paroxysme en 2022. La dernière étude de l'Observatoire de la vie étudiante date de 2021. Il a fallu attendre la forte mobilisation des étudiants contre les retraites pour qu'une nouvelle étude soit lancée au mois de mars. En l'absence de données objectives. Les syndicats étudiants les universités établissent leurs propres chiffres qui ne sont pas toujours pris au sérieux par le gouvernement et c'est un problème car il faut d'abord être en mesure des balles tu une situation pour y répondre. C'est pourquoi nous proposons cet amendement. Merci la vue de la commission. Monsieur le rapporteur. Il y. Merci madame la présidente, madame la Ministre, Monsieur le président de la commission chers. Collègues de Marco. C'est un avis. on vous l'a on l'a dit en commission parce que le but de ce texte et du conventionnement qui sera proposé dans sa généralisation est justement de lutter contre la précarité étudiante et je me permets de le dire parce que je n'ai pas je ne l'ai pas dit dans mon propos introductif que l'ensemble des syndicats étudiants que nous avons reçues avec. Pierre-Antoine Levi ont émis aussi hein. Un avis positif sur notre texte et je pense que c'est important de de le dire, mais c'est un avis donc sur cet amendement de modification un avis défavorable avec toujours autant de bienveillance. L'avis du gouvernement. Madame la Ministre un bout de réponse parce que je partage global vraiment avec vous. Ce besoin de bilan ce besoin et je voudrais vous apportez comme information que nous attendons un bilan sur les 10 millions dont vous avez parlé, dont nous avons parlé tout à l'heure d'aide sur les associations et les banques alimentaires pour essayer de mieux identifier les besoins de précarité et les besoins de ces étudiants. Premièrement, donc nous attendons ce bilan et cette identification et puis il y a l'enquête de l'Observatoire vie étudiants qui arrive en général en fin d'année et et donc sur lequel nous aurons une attention particulière bien sûr cette année encore plus en fin d'année 2023, nous pourrons le faire un rapport donc nous avons des outils pour évaluer et je voulais vous en faire part et nous y serons très attentifs. Je vous remercie. Merci. Alors je mets aux voix de Raymond mon numéro 3 qui a reçu un avis défavorable bienveillant de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté, je me vois l'article 1er bisquer pour Contre qui s'abstient et donc adopté l'article 3 reste supprimer les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe de l'Union centriste. Sur l'ensemble de cette proposition de loi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande pas à voter. Le scrutin est clos. Un résultat du scrutin. Nombre de votants 344 exprimés, 267 pour, 267 contre. Il en a pas donc. Le texte a été adopté. Unanimité. Je vais je vais. Suspendre la séance pour quelques instants, le temps que chacun soit à sa place pour le prochain texte hein. La séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi. Visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Présentée par Madame Billon filleul variant et plusieurs de leurs collègues. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte et dans la discussion générale. La parole est à madame la présidente Annick Billon, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois qui va nous rejoindre madame la rapporteure chers Françoise chers collègues, je me réjouis de l'examen aujourd'hui d'une proposition de loi corédigé avec mes collègues de la délégation aux droits des femmes. Dominique Vérien et Martine Filleul cette proposition de loi issu des travaux de notre délégation consacrée à la parité dans la haute fonction publique et au bilan d'application de 10 ans de la loi dite Sauvadet du 12 mars 2020, Elle fait suite au rapport que mes collègues ont publié en juin 2022, intitulé parité dans la haute fonction publique. Changer de braquet. 10 ans après la loi Sauvadet. La loi Sauvadet impose aux employeurs publics de respecter une proportion minimale de chaque sexe pour les primo-nominations dans près de 6000 emplois d'encadrement supérieur et de direction. Depuis 2017, ce quota est de 40% et être assorti de pénalités financières s'élevant à 90.000 euros par unité manquante progressivement ses obligations paritaire ont été atteintes dans les 3 fonctions publiques ainsi le taux de Primo nominations féminines dans les emplois d'encadrement supérieur et de direction a progressé de 10 points entre 2013 et 2020. En 2020 le quota a même été atteint pour la première fois simultanément dans les trois versants de la fonction publique. Nous avons toutefois identifions 3 principaux points de vigilance premièrement déclinée par fonction publique et par le ministère. Les résultats sont instables d'une année sur l'autre avec une progression en dents de scie. Deuxièmement les quotas Sauvadet qui sont des quotas de flux n'ont pas conduit à une accélération notable du stock c'est-à-dire de la proportion de femmes dans les feux emplois de direction et d'encadrement. Les femmes n'occupent aujourd'hui encore qu'un tiers des emplois d'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique. Pourtant l'objectif final des quotas Sauvadet et précisément d'agir sur le stock. Au-delà du flux. Troisièmement, la proportion de femmes reste plus faible dans les ministères historiquement masculin et dans les emplois considérés comme plus prestigieux ou plus technique au sein de la fonction publique d'État, la proportion de femmes occupant un emploi supérieur était de 33% en 2020 au niveau global, avec des variations notables entre ministères. 46% pour le ministère des Affaires sociales, 32% pour le ministère de l'Intérieur, 31 pour celui de la culture et 27% pour celui de l'Économie et des Finances cependant dans la fonction publique d'État, la proportion de femmes augmente au sein de tous les postes, y compris à plus haut niveau de responsabilité. Au sein de la fonction publique territoriale, la proportion de femmes nommées à des postes à responsabilité a nettement augmenté mais les nominations ont concerné essentiellement des postes de directeur adjoint des services déjà occupé à 41% par des femmes en 2020 tandis que seuls 20% des postes de directeur général des services DGS et 15% des postes de directeur général des services techniques sont occupés par des femmes. Enfin dans la fonction publique hospitalière une féminisation historiquement élevé cache une situation contrastée. En 2020 42 % des emplois d'encadrement supérieur et dirigeants ils sont occupés par des femmes. Pour autant, les femmes sont davantage à la tête d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 53% des femmes et de direction de soins 74% de femmes dans les hôpitaux et CHU considéré comme plus prestigieux. La proportion de femmes à la tête d'établissement et respectivement de 27 et 39%. Par effet de miroir, les disparités dans les Poste se retrouve également au niveau des salaires. Forte de ces constats. Notre délégation avait formulé 12 recommandations visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la haute fonction publique. Elle recommandait notamment d'élargir les obligations paritaire et de renforcer la mobilisation des employeurs publics autour d'une politique d'égalité professionnelle et salariale ambitieuse. Ces recommandations ont abouti à la rédaction de cette proposition de loi. Je tiens à remercier la rapporteure Françoise Dumont qui a été à l'écoute des préoccupations de notre délégation et avec qui nous avons pu collaborer afin d'améliorer encore ce texte. Je remercie également le ministre de la transformation et de la fonction publique Stanislas Guerini, qui s'est montré très attentif et s'est engagé à avancer sur certaines de nos recommandations d'ordre réglementaire. Je pense notamment à des sujets techniques mais essentielles telles que la transparence des données celles-ci sont aujourd'hui publiés avec un décalage de 2 ans, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant. C'est un véritable travail de co-construction législative auquel nous nous sommes attelés ensemble. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui présente 3 grandes avancées par rapport à la législation actuelle.

elle introduit un quota de stocks à compter de 2029, un taux minimal de 40% de personnes de chaque sexe s'appliquera dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique. Enfin elle instaure la publication d'indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et de représentation dans les emplois supérieurs et de direction entre femmes et hommes. L'index de l'égalité professionnelle a prouvé son intérêt dans le secteur privé et je me félicite que les employeurs publics puissent être également astreint à la publication de telles statistiques genre Nous ne pouvons convaincre de la nécessité de faire progresser la parité que si nous disposons de. Statistiques objectives vend les inégalités qui persistent entre femmes et hommes comme nous le répétons souvent au sein de notre délégation. Il faut compter les femmes pour que les femmes compte. Si les quotas font souvent débat lors de leur instauration ils font toujours preuve de leur efficacité. Nous en sommes convaincus au sein de cette délégation tout comme nous sommes persuadés de la nécessaire exemplarité des employeurs publics en matière de parité. Les employeurs publics, emploie aujourd'hui près de 6 millions d'agents, soit 20% de l'emploi en France et 62% des femmes parmi ses agents toutes catégories confondues. Ils peuvent et doivent donc jouer un rôle moteur dans la progression de l'égalité et de la parité dans notre pays. L'égalité ne progresse que sous la contrainte. Je pourrais même dire hélas depuis le 8 juillet 1999 différents quoi se sont succédé pour favoriser l'accès des femmes aux responsabilités politiques, professionnelles, sociales. Ce texte marque donc une nouvelle étape pour plus de mixité dans la haute fonction publique. C'est un signal fort d'exemplarité pour l'ensemble de notre société. Une nouvelle étape qui en appellera forcément d'autres sur la longue route escarpée vers l'égalité. Une société plus égalitaire pour l'intérêt de tous les hommes et les femmes. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Françoise Dumont, qu'à partir de la commission des lois pour 10 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues, nous examinons la proposition de loi déposée par madame Annick Billon Martine Filleul et Dominique Vérien visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, comme l'a rappelé la présidente Annick Billon, cette proposition de loi découle des travaux menés par la délégation aux droits des femmes en 2022 sur le bilan des 10 ans d'application de la loi dite Sauvadet dans sa version initiale, la proposition de loi visait à traduire IV des 12 recommandations formulées. Alors dans le but d'accélérer la féminisation des postes à responsabilité dans la fonction publique, à savoir le relèvement à 50% du taux de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants l'élargissement du Champ d'application de la loi Sauvadet la systématisation des pénalités financières à l'encontre des employeurs publics ne respectant pas l'obligation de nominations équilibrées, ainsi que l'instauration d'un index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Commission partagent là où l'objectif général de la proposition de loi. 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi Sauvadet la présence des femmes aux postes à responsabilité est encore minoritaire et il convient donc d'y remédier. La commission a toutefois considéré que cet objectif louable devait se concilier avec des impératifs des d'efficacité d'opérationnalité et de proportionnalité. S'agissant des articles 1 2 et 3 de la proposition de loi, elle a ainsi estimé que le texte déposé ne respectait pas tout à fait ses exigences et a donc apporté un certain nombre de modifications afin de rendre les dispositions applicables par les employeurs publics et bénéfique pour pour l'ensemble des agents publics. S'agissant de l'article 4 à la, au contraire, considérer que la disposition initiale visant à instaurer des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et de représentation entre les hommes et les femmes devaient être consolidée afin d'en renforcer sa portée si nous examinons le texte dans le détail la con. La commission a considéré. Que l'augmentation du taux à 50% de personnes de chaque sexe dans les nominations qui était proposée par l'article 2 du texte initial se heurterait à des difficultés d'application, voire aurait des effets contre-productifs pour les hommes comme pour les femmes en effet une telle disposition reviendrait à nommer rigoureusement 50% de femmes et 50% d'hommes. Si bien qu'elle serait inapplicable en cas de nomination en nombre impair de manière générale, elle ne laisserait aucune marge de manoeuvre aux employeurs publics. Il est d'ailleurs fort à parier qu'une telle obligation ne serait en pratique jamais respectées et que l'ensemble des administrations se trouverait contrainte de payer la pénalité financière prévue pour non respect de l'obligation des nominations équilibrées. L'instauration d'un taux de 50% serait également contraire à l'intérêt des femmes en ce qu'elle empêcherait des nominations selon un ratio autre que 50 50, y compris dans un sens favorable aux femmes en rigidifier les recrutements. Elle pourrait également se révéler contraires à l'intérêt des fonctionnaires dont les chances de progression de carrière, pourrait être amoindrie. S'ils ne sont pas du bon sexe c'est-à-dire celui permettant de satisfaire un taux strict de 50% je pense que le risque de voir les considérations liées au sexe, l'emporter sur celles liées à la compétence ne doit pas être sous-estimé. C'est pourquoi la Commission a préféré porter le taux de Primo nominations à 45% au moins deux personnes de chaque sexe. Par ailleurs, il convient de laisser le champ le temps aux administrations de s'adapter à cette obligation renforcée et il faut en particulier veiller à ne pas produire d'effet sur les cycles de nomination en cours dans le versant territorial c'est pour soi. C'est pour cela que la Commission a souhaité que le taux de 45% entre en vigueur au 1er janvier 2025 dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière et à l'issue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes de la fonction publique territoriale. La commission ensuite estimé que l'élargissement du Champ des emplois soumis à l'obligation des nominations équilibrées telle qu'il était proposé par l'article 3 dans la version initiale de la proposition de loi n'était pas opportun d'une part, il lui a semblé qu'étendre ce choix aux emplois dits d'encadrement supérieur risquerait de générer un risque d'insécurité juridique dans la mesure où une telle notion n'est pas définie dans la loi. D'autre part baisser à 20.000 habitants. Le seuil de population pour les communes et les EPCI concernés par l'obligation de nominations équilibrées n'a pas non plus semblé opportun dans la mesure où cela risquerait d'Accenture et les difficultés de recrutement des collectivités comptant entre 20.000 et 40.000 habitants. La commission a en revanche précisé la définition des employes assujettis à l'obligation de nominations équilibrées, s'agissant des des établissements publics de l'État et de la fonction publique hospitalière dans un but de clarification et de cohérence. La commission a salué l'instauration par l'article IV de la proposition de loi d'indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et de représentation. Cette initiative est bienvenu. D'autant qu'un tel index existe index existe déjà dans le secteur privé depuis 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et depuis 2020 pour les entreprises de plus de 50 salariés. Elle a souhaité renforcer la portée de cette disposition en reprenant et adaptant les mesures prévues pour le secteur privé. Elle a ainsi crée une nouvelle section au sein du code général de la fonction publique consacrée à la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. D'une part et à la mesure des écarts de représentation au sein des employes supérieurs de direction. La commission a veillé à ce que les employeurs publics dispose d'un volume de données permettant des statistiques significatives. C'est pourquoi elle a décidé que seuls les administrations publiques disposant d'au moins 50 agents en gestion se verraient appliquer de nouvelles obligations relatives aux indicateurs de rémunération pour les collectivités territoriales ce critère serait. Avec le seuil de 40.000 habitants de plus, afin de garantir le respect de ses obligations. La Commission a prévu des sanctions financières en cas de non-, publication des écarts de rémunération ou de non-, publication des écarts de représentation. Elle pourrait également être prononcée. Si les écarts de rémunération constatés sont supérieurs à un niveau défini par décret. Un tel index se fondera sur les données du rapport social unique élaboré au printemps par les administrations publiques en conséquence il ne pourra lui-même pas être disponible avant le printemps de chaque année. Nous proposons donc une entrée en vigueur au 1er juin 2024 dans la fonction publique d'État. Au 1er juin 2025 dans les versants territorial et hospitalier pour finir, la commission a jugé nécessaire d'aller plus loin que l'obligation de publication des écarts de représentation entre les hommes et les femmes dans les emplois soumis à l'obligation de nominations équilibrées que prévoit l'article comme l'a rappelé la présidente de la délégation aux droits des femmes le taux obligatoire sur les premiers primo nomination n'apporte qu'une réponse partielle à la question de la féminisation des emplois à responsabilité dans la fonction publique pour garantir le maintien des femmes en fonction. La commission a souhaité instaurer un taux minimal de 40% de personnes de chaque sexe dans les emplois supérieurs de direction à l'article 3 bis cette disposition recommandé l'an dernier par la délégation aux droits des femmes. Mais non présentes dans le texte initial de la proposition de loi est d'autant plus justifiée qu'une obligation analogue est prévu dans le secteur privé depuis la loi Rixain de décembre 2021, les entreprises qui emploient plus de 1000 salariés devront à partir du 1er mars 2029. Respecter le taux de 40% de personnes de chaque sexe au sein des cadres dirigeants et et des membres des instances dirigeantes. Sur le modèle également du privé, la Commission a décidé de sanctionner le non-respect de cette obligation par une pénalité financière d'un montant maximal de 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. C'est donc, mes chers collègues, un texte alliant ambition alliant ambition et opérationnalité que la commission des lois vous propose d'adopter. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stanislas Guerini Ministre de la Transformation et de la fonction publique. Madame la vice-présidente de la commission des lois. Madame la rapporteure Françoise Dumont. Madame la présidente de la délégation du droit des femmes du Sénat cher Annick Billon mesdames les sénatrices Dominique Vérien et Martine Filleul. Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Je le dis. Sans détour. Nous nous apprêtons aujourd'hui si votre. Votre le confirme à franchir une étape importante pour l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Le débat parlementaire que nous entamons aujourd'hui en examinant autre proposition de loi. Est un moment décisif pour la fonction publique et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Grâce à l'engagement de la délégation des droits des femmes du Sénat. Au travail que je veux saluer de sa présidente des auteurs du texte de la rapporteur de la commission des lois, nous examinons je crois un texte d'utilité publique qui a vocation, dans ce convaincu à rassembler au-delà des clivages partisans. Et je l'espère, dans les deux chambres. Je veux vous dire aujourd'hui, l'honneur qui est le mien en tant que ministre de la fonction publique de travailler avec la chambre haute à cette noble cause. Et j'ajouterais qu'il est bon dans les temps que nous vivons de débats agités où la démocratie est parfois bousculé. De pouvoir mener ensemble un travail. Sérieux dans la sérénité. Cette marche que nous franchissons, nous permet d'avancer de façon décisive sur vous le rappeliez, madame la rapporteure et madame la présidente, un chemin qui a été engagé toutes majorités confondues depuis de nombreuses années déjà. C'est la loi Sauvadet de 2012. Qui a crée le dispositif de domination équilibrée dans la fonction publique, c'est l'accord de novembre 2018 qui a rendu obligatoire la nomination de référent pour l'égalité professionnelle dans chaque versant de la fonction publique, c'est la loi de transformation de 2019 qui a rendu obligatoire pour les employeurs publics de publier et de négocier des plans d'action sur l'égalité professionnelle. Et cela a déjà porté des fruits. En disant nous avons réduit de 10% les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique en 10 ans, vous le rappeliez, nous avons réussi à atteindre 40% de prime aux nominations dans les emplois supérieurs dans les trois versants là aussi de la fonction publique. Et pourtant, mesdames et messieurs les sénateurs, regardons la réalité en face. Le salaire moyen des femmes reste encore inférieur de 12% à celui des hommes dans la fonction publique, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable quand on est le premier employeur du pays, qui plus est avec 62% de femmes dans la fonction publique, nous avons je crois un devoir d'exemplarité. Mais je veux le dire clairement. C'est aujourd'hui aussi et peut-être même surtout un enjeu d'attractivité et tout simplement d'efficacité pour la fonction publique. C'est sur cette conviction partagée mesdames les sénatrices que nous avons initié nos échanges. Quelques semaines après ma prise de fonction. Nous avons travaillé ensemble récemment encore avec la présidente de la délégation du droit des femmes de l'Assemblée nationale, c'est important et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'examiner cette proposition de loi ambitieuse et réaliste. Les échanges que j'ai eue avec vous, avec les réseaux féminins, avec les associations, avec les employeurs ont renforcé ma conviction qu'il fallait poursuivre 2 objectifs. D'abord briser le plafond de verre définitivement mais aussi réduire les inégalités de rémunérations dans l'ensemble de la fonction publique, c'est le sens des annonces que j'ai pu porter à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes et je me réjouis que cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui incarne ces 2 priorités je le disais fracturer définitivement une bonne fois pour toutes le plafond de verre je veux garantir que chaque femme puisse accéder aux plus hauts postes des trois versants de la fonction publique. Je ne cesserai de le dire, ce sont les compétences et les talents qui fonde les promotions. Mais pour mettre fin aux pesanteurs parfois, y compris culturel, sociologique. Nous avons la responsabilité de fixer un cap, y compris par la norme et quand cela est nécessaire en assumant des sanctions. C'est pour cela que nous voulons rendre plus ambitieux. Le dispositif de nominations équilibrées, vous l'avez dit d'abord en élargissant les employeurs publics concernés ensuite en fixant une nouvelle ambition pour porter à 45% les primo-nominations dans ce quinquennat. Mais je crois que nous ne devons pas nous arrêter là en portant uniquement le regard sur les flux de nomination. On sait que la réalité c'est que aujourd'hui trop souvent le turn-over concerne davantage les femmes que les hommes aux postes d'encadrement supérieur et dirigeants et c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé la volonté du gouvernement d'intégrer une ambition en termes de stock d'emplois également. Nous avons le film. Il nous faut aussi la photographie c'est une obligation de résultat que nous avons et vous l'avez intérêt dès la commission je voulais vous en remercier. Mais je le disais, briser le plafond de verre ne suffit pas. Entre plus ambitieux, c'est porter une vision de l'égalité salariale pour l'ensemble de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un index d'égalité professionnelle dans la fonction publique, il n'existait que pour le privé, vous le savez, j'ai considéré que ce n'était pas normal et que cet outil serait tout aussi utile en tant qu'employeur public. Je le dis régulièrement un index c'est fait pour pointer. Pointer les inégalités et les efforts qu'il nous reste à déployer. Demain, grâce à cette proposition de loi. Les employeurs publics auront l'obligation de publier leurs résultats sur les indicateurs de l'index. Nous les définiront pour les trois versants précisément par décret en dire un mot ici à la tribune. Évidemment, nous aurons à mener un travail d'adaptation par rapport à l'index Pénicaud qui existe dans le privé. Et je souhaite qui nous permettent de mesurer à la fois les écarts de rémunération. Pour les fonctionnaires comme pour les agents contractuels. Je crois que c'est très important. ne me permettent de mesurer aussi l'égalité en matière de promotion que les promotions soient équilibrées et sur l'égalité des postes les plus influents et les mieux rémunérés dans la fonction publique et si ces informations ne sont pas publiés. Il y aura des sanctions. Et si ces résultats ne progresse pas. Il y aura également des sanctions. La publication, je veux le dire aussi de cet index ne remplace évidemment pas et naturellement pas les plans d'action que les que les administrations, que les collectivités que les hôpitaux doivent mettre en oeuvre et je souhaite, je voulais aussi vous l'indiquer que nous puissions avec les organisations syndicales négocier un nouvel accord ambitieux pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour les prochaines années. Vous le voyez. Mesdames sénatrices messieurs les sénateurs, ce texte nous rassemble autant qui nous engage vis à vis du pays. Je souhaite que nous puissions le promulguer. À l'été et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a choisi d'engager la procédure accélérée. Je termine en vous indiquant que je proposerai à votre, votre 4, évolution à travers 5 amendements du gouvernement. La première évolution, c'est la nécessité d'accompagner les administrations parfois les collectivités. Qui partent de plus loin, pour leur permettre d'atteindre réellement les cibles exigé. En introduisant une première obligation de progression par rapport à leur situation de départ. La 2ème évolution touchera aux sanctions sur les stocks que je vous proposerai d'harmoniser avec le mécanisme de sanction forfaitaire qui existent pour les primo-nominations. La 3ème évolution c'est exigence accrue que je souhaite porter pour les emplois qui sont à décision du gouvernement et dans les cabinets ministériels. Je vous proposerai de viser 50% sur le quinquennat. Je m'étais engagé le 8 mars devant vous. je vous propose de l'inscrire dans la loi aujourd'hui enfin je porterai un amendement sur la rédaction de l'index, notamment pour qu'ils puissent rentrer en vigueur le plus rapidement possible. Mesdames et sénatrices, messieurs les sénateurs. Franchissons ensemble cette nouvelle étape. Attendue par beaucoup d'agents et je crois par beaucoup de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. Alors dans la suite de la discussion générale. La parole est à madame Martine Filleul pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes.

Madame la présidente. Madame la rapporteur Monsieur le Ministre. À l'issue de notre rapport de la délégation aux droits des femmes sur le bilan de l'application de la loi Sauvadet. Nous avons souhaité porter avec mes collègues Annick Billon et Dominique Vérien que je salue cette proposition de loi car nous avons chevillée au corps, à la fois l'égalité entre les hommes et les femmes et la fonction publique. La fonction publique qui est un des piliers de notre démocratie. Depuis 1945, elle participe à sceller le pacte républicain. Ce ne sont pas moins de 5 millions et demi d'agents engagés au quotidien au service de la population sur tout le territoire français. Guidé par le sens du devoir. Force est cependant de constater que cette fonction publique est en perte de sens et en perte d'attractivité manifestement elle n'attire plus. Confère le peu de candidats aux différents concours la diminution progressive mais drastique des moyens alloués aux services publics ainsi que celle du pouvoir d'achat des agents. Il y est pour beaucoup. Le choix du recours important aux contractuels, a de son côté affaibli le sens de cet outil au service de la République. Le revitaliser le renforcer le valoriser le moderniser le rendre exemplaire est un impératif dans une société fracturée exemplaire. On est loin du compte en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et en particulier en matière de salaire. Les hommes, vous le disiez, Monsieur le Ministre reste rémunérés en moyenne 12% de plus que les femmes en matière de parité alors que 60% des agents publics sont des femmes. Les postes de direction sont encore très majoritairement occupés par des hommes. La loi Sauvadet de 2012 a certes permis d'impulser un réel changement en imposant aux employeurs publics un quota pour les primo-nomination qui a atteint l'objectif fixé de 40% de femmes en 2017. Mais il faut, comme le dit le rapport de la délégation aux droits des femmes résolument changé de braquet car le compte n'y est toujours pas la cible des primo-nominations ne permet pas d'alimenter le nombre de femmes réellement en fonction dans des postes de direction. On observe que les sanctions mises en place sont contournées en utilisant les statistiques ou différents stratagèmes. Au final, le nombre de postes soumis à la loi Sauvadet reste réduit. Il n'y a pas eu de ruissellement. Cette proposition de loi progressive parie sur le long terme et repose sur 4 principes directeurs cher preuve d'intransigeance, en prévoyant la suppression de toute dispense de pénalités financières pour qu'aucun employeur public ne puisse se soustraire aux quotas des primo-nominations, faire preuve d'ambition en relevant le quota de Primo nomination du sexe sous-représenté pour atteindre 45%, avec un élargissement des employes concernés. Faire preuve de cohérence pour corriger la cible d'origine en instaurant un quota de 40% du sexe sous-représenté dans le stade des employes concernés et finalement faire preuve de rigueur pour que l'exigence soit au moins aussi important dans la fonction publique que dans le secteur privé. Cette proposition de loi comporte la mise en place d'un index qui doit être réalisée et rendue publique, tous les ans. Cependant. Le groupe socialiste avec en particulier mon collègue Didier Marie vous proposera de consolider ses principes. Les conclusions du rapport sont sans équivoque. Nous devons aller plus vite et nous devons faire preuve de plus d'ambition. C'est tout le sens des amendements que nous défendrons avec mon groupe, la parité ce n'est pas 45% c'est 50% et nous devons inscrire cet objectif dans le marbre de notre législation et nous ne pouvons pas attendre jusque 2029 pour l'entrée en vigueur du quota à 40% sur le stock. Mettons-nous d'accord aujourd'hui sur 2027. Pour élargir le nombre d'emplois concernés par les quotas. Nous proposons de dépasser le débat relatif à l'abaissement ou non du seuil démographique 40.000 ou 20.000. Il suffit de généraliser l'obligation de nominations équilibrées dès lors que la collectivité dispose d'un nombre d'emplois fonctionnels supérieure ou égale à Enfin nous portons la volonté que les communes les plus ambitieuses les plus volontariste qui se donne les moyens d'aller plus loin, ne soient pas pénalisées pour leurs efforts que Paris Lille ou d'autres villes se voient appliquer des sanctions financières pour avoir trop de femmes à des postes de responsabilité est incompréhensible. À l'heure d'un déséquilibre majeur au niveau national. En conclusion, cette proposition de loi n'est pas un aboutissement final dans l'évolution de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, mais c'est tout le sens de l'histoire et du progrès, ainsi que du féminisme, comme l'a très justement dit Gisèle Halimi. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang alors j'ai l'espoir que d'autres après, après nous reprendrons le flambeau pour poursuivre ce combat.

donc à 20h 35. Il y a quand même pas mal d'amendements, donc je suis désolé. Merci beaucoup. La parole est à madame Marie-Claude variable pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 4 minutes. Monsieur le Ministre, madame la rapporteur Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans leur vie professionnelle les femmes subissent de nombreuses contraintes, qui peuvent les pénaliser pour construire une carrière dans de bonnes conditions mais qui, de surcroît prive le monde du travail, de talent et de force considérable. L'égalité des sexes et plus qu'un objectif en soi, c'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté de la promotion du développement durable et de la goût de la bonne gouvernance c'est Kofi Annan qui disait cela. Nous savons aussi tout ce que si le taux d'emploi des femmes et leur rémunération étaient égaux à ceux des hommes. Le produit intérieur brut de la France bon direz de 6,9% contribuant. C'est l'actualité par là même alimenté le financement de nos caisses vieillesse. Le travail qui a été menée par nos collègues Annick Billon Martine Filleul et Dominique Vérien. Au sein de la délégation aux droits des femmes du Sénat révèle que 10 ans après la loi Sauvadet effectivement qui imposé des obligations paritaire dans la haute fonction publique, les résultats restent en demi-teinte. Car non seulement un tiers des emplois à responsabilité dans l'autre fonction publique est occupé par des femmes. Le Haut Conseil d'État, l'égalité entre les hommes et les femmes évoquée dans un rapport de 2021 une politique de petits pas et des difficultés des résistances dans la mise en oeuvre de cette loi. Le quota de 40% de Primo nominations féminines en vigueur depuis 2017 n'a été atteint en fait qu'en 2019 et 2020. Alors oui, la situation a évolué mais pas aussi rapidement qu'il eut été souhaitable dans la fonction publique d'État, la proportion de femmes occupant un emploi supérieur était de 33% en 2020. IV ministère je le rappelle, Affaires étrangères, les armées l'économie, les finances et les services du Premier Ministre ont dû s'acquitter d'ailleurs de pénalité à hauteur de 1.080.000 euros. Dans la fonction publique hospitalière très féminisée, elle n'occupe que 27% des emplois fonctionnels de directeur d'hôpital et 39% des postes de directeurs de CHU et si dans la fonction publique que j'ai particulièrement bien connu, on note une nette augmentation ces 15 dernières années, ce progrès ne saurait occulter que si les femmes occupent 41%. Comme l'a dit Annick Billon, des postes de directrice générale adjointe des services, seulement 20% sont directrice générale et 15% directrice des services techniques, les employeurs publics ont un rôle d'exemplaires d'exemplarité plat ces principes d'égalité et de parité au sein de leurs amis de leur administration. L'organisation du travail ne doit plus être limité à des logiques genre et et l'égalité salariale et professionnelle doit être réalité dans une, dans nos administrations comme dans nos entreprises. Ce texte proposé par nos collègues et de nature à aider en ce sens. Le taux de nominations aux emplois supérieurs pour chaque sexe passerait de 40 à 45%, même si je concède aussi que la parité c'est 50%. La portée de l'annexe de l'égalité professionnelle se trouvent renforcés avec des sanctions financières et un stock d'emplois et mis en place pour assurer une féminisation effective C'est la raison pour laquelle avec mon groupe, je voterai ce texte non sans souligner et j'y tiens, que nous devons nous ne devons pas oublier toutes celles en première ligne qui ont porté le service public. Quand le pays était à l'arrêt. Celle pas suffisamment. Reconnus à leur juste valeur. Avec des salaires qui ne sont pas en adéquation avec leur mission. Nous retrouverons cette question d'ailleurs demain dans la PPL proposition de loi proposée par notre groupe CRCE s'agissant des secrétaires de mairie dans les petites communes et la situation est bien réel les concernant. Merci, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame, Dominique Vérien pour le groupe Union centriste pour six minutes. Madame la présidente. Monsieur le ministre, hein. Madame la vice-, président de la commission des lois. Madame la rapporteure chers Françoise mesdames les coauteurs cher Annick et chère Martine mes chers collègues. Si vous le voulez bien, commençons tout de suite par aborder le sujet qui fâche les quotas. Je vais vous faire une confidence, je ne les aime pas. J'aimerais moi aussi que l'on puisse s'en passer et que les compétences des femmes soit naturellement reconnue et leur permettent d'accéder aux plus hautes responsabilités. Vous pourrez me rétorquer que c'est déjà le cas et vous auriez raison. Oui des femmes sont bel et bien aux plus hautes fonctions de notre pays et plusieurs d'entre vous ici présentes en sont l'exemple. Cependant, pour paraphraser Audiard. Il existe aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. Car le problème des femmes. C'est qu'elles n'osent pas revendiquer leurs capacités souvent parce qu'elles en doute elles-mêmes. Il semblerait que pour candidater à un poste un homme ose le faire dès qu'il coche 60% des compétences requises. Une femme 80%. On trouve audacieux, un homme qui vient réclamer une augmentation de salaire. Arriviste. Une femme qui le ferait. Heureusement. Nous en sommes de plus en plus consciente et pas plus tard que la semaine dernière, une association d'ingénieur au féminin organisé un séminaire pour apprendre à parler d'argent. Des femmes qui achètent qui compte qui vendent, qui compte combien coûte qu'elles construisent, qui ont fait 5 ans d'études après le bac ont besoin d'apprendre à parler d'argent. Apprendre à osé demander ce qu'elle pense mériter en 2023 mais il est vrai que l'on ne dispose de notre liberté de gérer que depuis le 13 juillet 1965, date à laquelle le Parlement votait l'autorisation pour les femmes d'ouvrir un compte en banque à leur nom et à travailler sans le consentement de leur mari. En attendant. 10 ans après l'adoption de la loi dite Sauvadet. Le compte n'y est toujours pas. Malgré l'instauration d'un quota de 40% de prime aux nominations et c'est probablement là que le bât blesse. Les seuls primo-nomination on compte plus hein. Quand une femme est nommé pas moins hein quand elle s'en va. Et quand les femmes sont présentes, bien souvent, elles ne se sont pas aux postes les plus prestigieux. Ce phénomène se vérifie dans les trois versants de la fonction publique, cela a été dit mais c'est plus d'un million d'euros de pénalités qui ont été réglés par les ministères pour ne pas avoir respecté les obligations paritaire dans nos territoires, on ne compte que 20% de femmes occupant des postes de directeur général des services et seulement 15% des postes de directeur général des services techniques dans nos hôpitaux enfin c'est 75% de femmes mais seulement 27% directrice d'hôpital là encore le quantitatif ne doit pas occulter la réalité du qualitatif. Pourtant, il est impératif que les employeurs publics fassent preuve d'exemplarité car ils emploient aujourd'hui environ 6 millions d'agents, soit 20% de l'emploi en France comme cela a été dit aussi, et 62% des femmes parmi ses agents toutes catégories confondues. En rehaussant à 45% de quotas sur les primo-nomination mais surtout en instaurant une obligation cumulative de 40% sur les emplois occupés. Je suis convaincu que nous aurons un virer table impact à moyen terme. En outre, la publication d'un index de l'égalité professionnelle permettra d'objectiver les écarts de rémunération et de représentation. Afin de garantir l'effectivité de cette obligation. Une sanction financière d'un montant maximal de 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels est prévue dans le texte. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous voulez revenir sur ce sujet en calant cette pénalité par décret. Pourquoi pas, mais je souhaite préciser qu'une sanction se doit de rester dissuasive, sinon, elle devient totalement inefficace. Mais peut-être pourrez-vous préciser mais d'ailleurs c'est fait partie des amendements qui ont été proposées et acceptées par la commission ce matin. Donc préciser dans ce décret que les sanctions seront rendus publics. Ce qui permettra de mieux connaître les administrations ayant des difficultés à appliquer la parité soit pour les aider si cela devait être par manque de viviers soit pour les contraindre, si aucune raison valable n'apparaissait. Bien sûr, le texte que nous examinons aujourd'hui aurait pu être un peu plus ambitieux et je m'adresse à ma collègue Martine Filleul, nous aurions pu voir un peu plus grand. Un peu plus vite mais je tiens ici à saluer le travail de notre rapporteure chers Françoise avec qui nous avons su trouver un compromis pour un texte équilibré et sans doute plus opérationnel. C'est là le principal car l'important reste que la situation professionnelle des femmes s'améliore et que notre fonction publique se dote d'une politique de ressources humaines à la hauteur de cet enjeu. J'en profite également pour vous remercier, monsieur le ministre a pour votre engagement sincère sur le sujet ainsi que pour votre volontarisme dans la construction de ce texte et naturellement le groupe Union centriste votera ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à madame la présidente Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la fonction publique, premier employeur de France se doit d'être exemplaire, notamment en ce qui concerne l'égalité ou l'égal accès des femmes aux responsabilités. Son action a d'autant plus de signification que les femmes managers travaillent plus fréquemment dans le secteur public que dans le secteur privé. Or, si 65% des femmes occupent des postes de catégorie A, elles ne sont plus que 42% à occuper des postes de catégorie A A plus avec un écart de rémunération moyen de 13%, selon les chiffres du rapport de la délégation aux droits des femmes de 2022, dont la proposition de loi reprend 4 recommandations. Le vivier donc là mais au XXIe siècle, il demeure encore des réticences à nommer des femmes à de tels postes notamment pour les plus prestigieux d'entre eux. Malheureusement seuls la contrainte semble permettre de renverser un statu quo et d'aboutir à un résultat plus rapide et visible. La loi Sauvadet a permis de faire un bond de 10 en matière de Primo nomination avec une progression atteint de 42% en l'espace de 10 ans. Cependant, cette évolution est loin d'être linéaire, ce qui prouve que cette revendication est encore loin d'être obsolète malheureusement cela nous oblige. Et puis ce qu'il subsiste encore des freins à l'accession des femmes aux responsabilités, il incombe au législateur de renforcer le droit en vigueur. Même si nous savons qu'il existe encore des opposants politiques des quotas. Ces derniers ont été l'un des moyens les plus efficaces pour infléchir la tendance aussi l'introduction par la commission d'un quota de 40% de perte. Sein de chaque sexe au sein des employes supérieurs et de direction constitue une réelle avancée qui faisait défaut. De ne s'appliquer qu'en 2029 laissera un temps d'adaptation qui peut s'avérer nécessaire. Par contre je serai pour ma part plus favorable à un relèvement des quotas de Primo nominations de 40% à 50% le taux de 45% retenu par la commission n'est pas suffisant car conjugué à la règle de l'arrondi à l'unité inférieure, il aboutit à un effet pratiquement nul en effet pour 4 nominations une seule nomination féminine serait suffisante pour remplir cette obligation. Rien ne changerait donc finalement par rapport à l'existant. Si ce n'est un effet d'annonce. L'argument avancé d'ailleurs dans le rapport, pour ne pas relever ce taux à 50% me laisse quelque peu perplexe. Il serait contraire à l'intérêt des fonctionnaires dont les chances de progression de carrière, pourrait être amoindrie. S'ils ne sont pas je cite du bon sexe. C'est pourtant exactement la situation dans laquelle se trouvent les femmes compétentes dont l'ascension professionnelle est entravée en raison de stéréotypes de genre. Mes chers collègues, la compétence comme l'incompétence n'ont pas de genre. Il n'y a pas plus de femmes incompétentes que d'hommes incompétents. Pour ce qui est de la fonction publique territoriale, l'application d'un taux de Primo nomination ne devrait pas dépendre de la démographie des communes ou des. Intercommunalités mais plutôt du nombre d'emplois fonctionnels, comme je le proposerai par amendement. Enfin je salue la mise en place de l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sur une partie des catégories à plus avec l'introduction par la commission des lois de pénalités financières. Certes, la loi ne réglera pas tout. L'organisation du travail doit se moderniser afin d'assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et nous pourrions à ce type de nous inspirer des pays nordiques, la crise sanitaire avait amorcé un changement de mentalité vers plus de souplesse, il faut poursuivre et la fonction publique a la capacité de le faire, notamment pour les postes à responsabilité. Je voudrais ici saluer le travail des auteurs de cette proposition de loi notre présidente Annick Billon. Martine. Présidente, je ne vais pas dire toute la délégation, parce que je n'ai plus le temps Martine Filleul et Dominique Vérien comme vous l'aurez compris, le groupe RDSE votera en faveur de la proposition de loi, bien qu'elle ne puisse pas faire disparaître à elle seule toutes les inégalités. Elle constitue néanmoins une Pierre à l'édifice pour atteindre une jeunesse. Reconnaissance du travail. Oui mais vous ne serez pas contente si je, si j'arrête et que le texte n'est pas fini hein. Je vous le rappelle encore une fois je vous rappellerai plusieurs fois la parole est à madame Laure Darcos pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Sa collègue. Monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi présentée par nos collègues Annick Billon Martine Filleul et Dominique Vérien que je salue spécialement cette proposition de loi est l'aboutissement d'un travail d'analyse approfondie menée par notre délégation sur la place des femmes dans la haute fonction publique. 10 ans après l'adoption de la loi Sauvadet. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus et que le bilan de celle-ci est assez contrasté. Assurément, il faut se réjouir de la progression du nombre de femmes occupant des postes à responsabilité. Le quota de 40% de prime aux nominations féminines a été atteint en 2020 dans les 3 fonctions publiques État territoriale et hospitalière. Pour autant, les femmes ne sont qu'un peu plus d'un tiers à occuper des emplois hautement qualifiés. Ces statistiques singulière résulte d'un billet de la loi Sauvadet qui a consisté à agir sur le flux plutôt que sur le stock. En outre, le nombre d'emplois concernés par le dispositif de prime aux nominations équilibrées est restreint aux seules fonctions supérieures et de direction, ce qui représente un gisement de moins de 6000 postes auxquels elles peuvent prétendre. La conséquence des choix opérés en 2012 est palpable. Aujourd'hui, le nombre de femmes occupant des emplois responsabilité progresse lentement, trop lentement et nous ne pouvons pas arguer le manque de candidates, le vivier existe, les femmes sont de plus en plus nombreux à accéder aux grandes écoles formant aux métiers de la fonction publique. Certes, plusieurs secteurs de la haute administration sont pourvoyeur d'emplois historiquement occupés par des femmes aux faiblement attractif pour les femmes. Devons-nous cependant nous résoudre à ce qu'elle soit réduite à la portion congrue dans ces secteurs là, qui se caractérise par une culture professionnelle et une organisation du travail particulière. Devons-nous nous résoudre à ce qu'elle soit écartée des employes jugés les plus prestigieux ou les plus techniques des trois versants de la fonction publique. Des résistances à la nomination des femmes existe, c'est une réalité. Il faut en connaître les ressorts pour mieux les combattre. Parce que nous sommes très lucide sur la situation et que nous mesurons bien que la politique des petits pas ne nous permettra pas de satisfaire l'objectif du de la stricte parité dans la haute fonction publique, dans un délai raisonnable. Il fallait agir de manière plus contraignante. La mesure la plus emblématique de la proposition de loi de nos collègues amendé par la commission des lois, consiste en l'élargissement progressif des obligations paritaires des employeurs publics. L'autre grande mesure du texte vise à inciter les organisations à s'engager en faveur d'une politique d'égalité salariale et professionnelle nettement plus ambitieuse. gens du renforcement des obligations paritaire. La proposition de loi prévoit de relever à 45% le taux de Primo nominations dans les emplois supérieurs et de direction à compter de 2025 pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière et à compter du prochain renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale. À la date du 1er janvier 2029 s'imposera par ailleurs un taux d'au moins 40% de personnes de chaque sexe sur le stock d'emplois concernés. Je me réjouis de ces avancées même si je ne méconnais pas les contraintes nouvelles qu'elles impliquent pour les collectivités territoriales qui pourrait être confronté à certaines difficultés de recrutement. Néanmoins, ces dispositions sont particulièrement bienvenues pour accéder pour accélérer pardon, l'accès des femmes aux postes à responsabilité mais également pour s'assurer de leur présence effective et continue dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique. S'agissant de la politique de rémunération et d'égalité professionnelle. Il faut souligner la décision judicieuse d'assujettir les employeurs publics comptant au moins 50 agents en gestion à la publication annuelle d'une part d'indicateurs portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et d'autre part de la mesure des écarts de représentation entre les 2 sexes. Le défaut de publications de résultats satisfaisants sera sanctionné financièrement. Ce sont des mesures pragmatiques et de bon sens qui vont permet de progresser vers une égalité réelle effective depuis un peu plus de 10 ans. L'égalité professionnelle est devenue un enjeu majeur des politiques publiques dans le champs des entreprises et la loi Copé Zimmermann et la loi du 24 décembre 2021, visant à accélérer égalité économique et professionnelle vont avoir un impact décisif sur la parité dans les conseils d'administration et les instances dirigeantes dans la fonction publique, la loi Sauvadet de 2012 à enclencher une dynamique vertueuse que parachève la proposition de loi examiné aujourd'hui. Je voudrais que chacun d'entre vous. Mesure bien ce qui vient d'être accompli en un temps relativement court. Le plafond de verre disparaît peu à peu pour les femmes qui pourront désormais montrer que leur talent et leurs compétences sont indispensables à la bonne marche de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. C'est pourquoi notre groupe Les Républicains votera sans réserve en faveur du texte qui nous est soumis, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre mais de vielles pour le groupe les indépendants pour 4 minutes.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure. Mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Elle découle des travaux menés en 2022 par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat sur le bilan de 10 ans d'application de la loi dite Sauvadet. Aujourd'hui codifié au sein du code général de la fonction publique. La loi Sauvadet impose aux employeurs publics de respecter une proportion minimale de chaque sexe pour les primo-. Nomination dans près de 6000 emplois d'encadrement supérieur et de direction. Les trois versants de la fonction publique d'État territoriale et hospitalière, sont concernés. Le calendrier d'application prévue par la loi Sauvadet étaient échelonnés d'abord fixée à 20% en 2013. Le quota de primes ont nominations féminines doit être de 40% depuis 2017. Ces obligations paritaire. Sont accompagnés de pénalités financières pour les employeurs publics. Ne respectant pas les objectifs fixés par la loi depuis 2017 le montant. Et de 90.000 euros par unité manquante. Néanmoins, le taux de féminisation des emplois supérieurs et de direction au sein de la fonction publique. Reste relatif. des différences notables ont été constatés selon les versants et selon le type et les cas d'emploi à l'intérieur de chacun d'entre eux. Afin d'accélérer la féminisation des postes à responsabilité dans la fonction publique. La proposition de loi de nos collègues Annick Billon Martine Filleul et Dominique Vérien initiative que je tiens à saluer reprend 4 mesures qui découle des recommandations élaborées en juin dernier par la délégation aux droits de la femme du Sénat. Ainsi l'article 1er de la proposition de loi rend. Les pénalités financières en cas de non respect par les employeurs publics de l'obligation de nominations équilibrées. L'article de relève à 50% le quota de nomination du sexe sous-représenté. Aux emplois supérieurs de dirigeants. L'article 3, quant à lui élargi de périmètre des employes concernés par les quotas. Enfin le dernier article instaure dans le secteur public. Un index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. afin de Rome de la proposition de loi plus efficiente vont dans le bon sens et je me félicite que les amendements proposés par le rapporteur et reçu l'accord des auteurs de la proposition de loi. Avant de conclure, je tiens à remercier la délégation aux droits des femmes. Qui nous a montré le chemin parcouru et le progrès qu'il nous reste à réaliser. Madame la Ministre, chers collègues. Bien que des disparités demeurent. La loi Sauvadet a largement contribué, en disant. À favoriser l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique les nouvelles mesures proposées dans le texte discuté aujourd'hui y participeront également. Et nous permettront de franchir, comme l'avait dit. Monsieur le Ministre, une nouvelle étape. On le groupe les indépendants votera cette proposition de loi. Merci, cher collègue, la parole est à madame Mélanie Vogel. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour 4 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues pour on peut prendre dans tous les sens l'égalité entre les genres est loin d'être atteinte en France les postes à responsabilité demeure souvent et qu'on est occupé par des hommes, y compris dans la fonction publique, ne compte seulement 3 femmes à la tête des entreprises du CAC 40, contre 65 hommes. Les secteurs à prédominance féminine en grande partie ceux du soin et du lien sont sous-valorisées et donc sous-payés et alors que la fonction publique devrait jouer un rôle d'exemplarité, puisque l'État peut décider d'être égalitaire, seulement un tiers des postes à responsabilité sont occupés par des femmes. Un tiers c'est c'est comme au Sénat fin aujourd'hui, j'ai l'impression que l'équilibre est un peu renversé mais en général c'est comme ça. Or la parité est un impératif pour l'égalité des droits pour la justice pour l'amélioration de nos politiques publiques. Et aussi ça a été dit pour notre richesse nationale, notamment celles qui contribuent à financer nos retraites, j'entends que la situation s'améliore, qu'en 2015, seulement 26% de ces postes étaient occupés par des femmes et je dois dire, c'est la logique même de ce raisonnement qui est vicié, si on se félicite d'une situation inégalitaire, mais un peu un peu moins que la veille, on n'atteindra jamais l'égalité des droits en matière de discrimination et d'inégalité. La question à se poser en tant que législateur jamais est ce qu'il est urgent d'y remédier. Mais est-ce qu'il est juste de faire perdurer cette inégalité cette discrimination alors qu'on peut y mettre fin, et la réponse pour toutes les inégalités pour toutes les discriminations. C'est toujours non. Or 10 ans après la loi Sauvadet, il apparaît clairement que cette loi n'était pas suffisante puisque la parité n'est toujours pas atteinte. Donc il faut changer la loi et la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui contribuera à combattre les inégalités. Et c'est la raison pour laquelle le groupe écologiste évidemment la vôtre. Madame la rapporteur je voudrais saluer votre travail qui a permis d'élargir certaines dispositions du texte. En revanche, je voudrais revenir sur certains points, vous voulez revenir sur l'ambition initiale du texte à certains endroits hein si vous proposer d'abaisser le taux pour les primo- domination de 50 à 45% pour chaque genre et nous appelons évidemment à maintenir l'objectif de 50% si nous voulons une loi juste et paritaire. Le seul objectif envisageable. C'est l'objectif paritaire et donc 50% pourquoi choisir délibérément de ne pas demander l'égalité mais juste un peu moins et l'argument du nombre impair. Je vous assure madame la rapporteure chez les écologistes. Nous avons beaucoup de systèmes internes pour faire la parité, même quand il y a des nombres impairs et ça marche très bien. Nous souhaitons également que les dispositions de cette loi entre en vigueur le plus rapidement possible. Si nous voulons vraiment que les choses changent. Nous ne pouvons pas nous contenter de règles qui entrent en vigueur dans 5 ans. C'est pourquoi nous opposons à tout délai supplémentaire. Un dernier mot enfin sur la nécessité d'aborder la question des inégalités de salaires et de représentation dans la société, d'un point de vue beaucoup plus holistique aujourd'hui ce qui compte au fond dans la société, c'est pas seulement les différences de salaire à poste égal entre par exemple de chef de service, un homme et une femme, c'est la distribution des postes au sein d'une entité entre les postes de direction et ce qui ne sont pas mais c'est aussi beaucoup les différences de salaires entre travail de même valeur entre les secteurs à prédominance masculine et féminine. C'est ce à quoi s'est attaqué par exemple, le Canada et l'Islande. Plus récemment, avec des résultats évidents On a établi des grilles pour déterminer la valeur de chaque travail en fonction des années d'études, responsabilité et etc et des grilles pour déterminer la prédominance d'un genre ou de l'autre dans les secteurs et on s'est aperçu qu'à travail de valeur égale les métiers dans les secteurs à prédominance féminine était sous-payés par rapport au métier dans les secteurs à prédominance masculine et vous savez ce qu'a fait l'État canadien. Avec les fonctionnaires. Dans ce cas, notamment les infirmières et ben il les a remboursés. Il leur a rendu l'argent. L'État a une dette envers les femmes de ce pays et si vous n'agissez pas plus vite, je peux vous dire que bientôt, elles viendront peut-être vous clamé son remboursement. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Nicole Duranton. Comme pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour 4 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Attaché au respect du principe constitutionnel de parité qui doit irriguer toutes les sphères d'activités qu'elle soit politique professionnelle ou sociale, j'ai cosigné cette PPL aujourd'hui nous voulons changer ce qu'il y a de plus anciens. Durable et profond dans l'état, le caractère très masculin de la haute fonction publique déposée par ma collègue, la présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Annick Billon, que je salue et cosignée par une vaste partie de collègues de tous les groupes. Cette proposition de loi vise d'une part à élargir les obligations des employeurs publics ainsi qu'à renforcer les sanctions et d'autre part à à renforcer la mobilisation autour d'une politique d'égalité ambitieuse. Beaucoup de chemin reste à parcourir. En effet, sur les 5,7 millions d'agents publics, 63% sont des femmes, mais seulement 43% pour la catégorie A, plus la proportion des femmes en. Responsabilités reste au dessus de 35% dans les ministères historiquement

Leur rémunération et de 11% moins élevés que celles de leurs homologues masculins. Depuis l'élection du président de la République sur l'égalité hommes-femmes grande cause des 2 quinquennats beaucoup de mesures ont déjà été prises, par exemple en 2019, la loi a créé un plan d'action pluri-annuelles obligatoire pour l'égalité et supprimer le jour de pour les congés maladie des femmes enceintes comme souligné dans le rapport remis par le Sénat en juin 2022, les quotas de femmes dans les postes à responsabilité ont été atteints dans les 3 fonctions publiques dès 2020. Continuons les efforts dans ce sens, c'est une autre rôle de législateur. Conformément à la Constitution de 1958 au statut général de la fonction publique, modifié en 2001 et à la loi sauva le 8 mars dernier, la Première ministre a présenté un nouveau plan pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je tiens à féliciter le gouvernement d'avoir maintenu un haut niveau d'ambition le déploiement de ce plan, contribuera aussi à faciliter la vie quotidienne des femmes fonctionnaires en particulier celles qui sont confrontées à un aléa de la vie par des mesures très concrètes. Le groupe RDPI accueille très favorablement les modifications que la commission des lois à apporter au texte initial qui sont cohérentes avec le nouveau plan inter-ministériel la suppression de dispense est reportée au 1er janvier 2029 le quota de Primo nomination et relever à 45% le chant des établissements publics concernés étaient. Un tour de 40 pour est appliquée aux stocks et les 2 versants de l'index sont distingués. Rappelons qu'en octobre 2021 à l'occasion de la discussion de la proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, notre groupe RDPI avait proposé la mise en place d'indicateurs annuels propositions restées lettre morte, les collègues de la commission des affaires sociales. Il en y étant défavorables. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de voir cette mesure reprise aujourd'hui notre groupe RDPI portera trois amendements pour pour compléter le texte issu de la commission. Le premier amendement, a pour objet de prévoir que le taux de 45% applicable aux primo-nomination entre en vigueur aussi pour des régions et départements oublié par la commission, le 2ème rédactionnel a pour objet de faire figurer dans un article dédié le disposition de publication des écarts dans la section relative relative aux nominations équilibré entre les hommes et les femmes, et enfin le 3ème a pour objet d'aligner le seuil de population à partir desquels les collectivités sont tenues de publier la somme des 10 rémunérations les plus élevées sur celui applicable à l'index d'égalité professionnelle soit 40.000 habitants. Je remercie Monsieur le Ministre d'avoir cette volontairement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, l'égalité femme-homme est un enjeu majeur et collectif qui doit être une priorité dans nos politiques publiques. C'est un enjeu qui doit être au coeur de notre société car il renvoie aux valeurs de notre devise républicaine bien évidemment l'égalité mais également la liberté et la fraternité en tant que législateurs, nous sommes régulièrement amenés à débattre de cet enjeu et des multiples questions qu'il soulève, notamment dans le domaine professionnel malgré plusieurs avancées significatives en la matière. Force est de constater que la situation des femmes reste plus fragile que celles des hommes travaillent à temps partiel, emplois à bas salaire plafond de verre carrières hachées inégalités salariales qui demeure une réalité en 2023. Ici même il y a quelques mois nous adoptions une proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle dans les entreprises aujourd'hui, c'est un texte qui concerne la fonction publique que nous examinons il y a 10 ans la loi Sauvadet marquer une évolution une évolution significative pour la fonction publique qui est, rappelons-le, le premier employeur de France avec 63% de femmes en son sein. Pour la première fois une loi imposer un taux minimal concernant les primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants de l'État mais également des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. 10 ans après, où en sommes-nous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes quant aux avancées permises par cette loi puisque nous constatons que le nombre de femmes a augmenté de manière significative et progressive et que les quotas de nominations ont été atteints dans les trois versants de la fonction publique, pour la première fois en 2020, la délégation aux droits des femmes, dont je salue ici le travail avait dressé l'an dernier, un bilan de cette loi et formuler des recommandations en vue d'accélérer la féminisation des emplois dans la fonction publique. Le texte que nous examinons on est le fruit grâce à l'initiative de la présidente de la délégation aux droits des femmes. Annick Billon ainsi que nos collègues Martine Filleul et Dominique Vérien. Je tiens également à remercier notre collègue rapporteur Françoise Dumont pour le travail mené son engagement depuis plusieurs semaines afin de parvenir à un travail et un texte équilibré applicable avec des objectifs également réaliste pour nos collectivités pour les primo-nomination un compromis a permis de retenir un taux de 45% au moins deux personnes de chaque sexe afin de laisser le temps aux administrations de s'adapter et de prendre en compte également des réalités et des difficultés de recrutement dans le même esprit, je partage l'avis de la rapporteure et de la Commission sur la nécessité de garder le seuil initial de population à 40.000 habitants afin de ne pas accentuer les difficultés des communes et des EPCI soumis à l'obligation de nomination. Sur le sujet majeur des questions salariales et de l'inégalité qui demeure une réalité dans notre pays, nous mesurons à quel point il est important d'objectiver les écarts de salaires qui perd 6 entre les femmes et les hommes. C'est l'objet de la mise en place de l'index de l'égalité professionnelle, telle qu'il existe déjà dans le privé depuis 2019. Je comprends et partage la nécessité. D'un tel outil. Attention cependant à mon sens à éviter l'utilisation en fait des index, on le voit bien au fur et à mesure des textes parce que ces index là doivent demeurer un outil au service d'une politique mais ne constitue pas en tant que telle la la politique les dispositions de ce texte sont autant d'avancées qui sont nécessaires et qui doivent être saluées en matière d'égalité dans le milieu professionnel. Un autre aspect, me paraît mériter toute notre attention et ça fera peut-être l'objet d'autres réflexions celui d'accompagner davantage les femmes dans le parcours de carrière et développer des méthodes de travail qui permettent de favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pareillement si nous souhaitons voir davantage de femmes prendre des responsabilités. Il me paraît important de développer des politiques pour les inciter et les encourager et également se sentir capable d'exercer des responsabilités et nous savons également à quel point l'interrogation sur la légitimité et malheureusement encore trop ancrée ancrée chez de nombreuses femmes enfin notre action doit également se porter sur la question de l'orientation professionnelle afin d'oeuvrer dès le plus jeune âge. Au niveau de l'école et de l'éducation nationale je finirai mon propos en soulignant que si la loi permet des avancées. On le voit bien. Nous avons également de belles initiatives sur nos territoires respectifs qui a un inside et qui plaide pour le changement et je tiens ici à saluer le travail notamment de l'association Femmes d'Alsace qui décerne chaque année des Marianne de la parité aux intercommunalités alsacienne les plus allantes en la matière et je salue et j'en profite. Les communautés de communes du riz de Marckolsheim et de Niederbronn les Bains et de Sélestat qui ont toutes les 3 été primé. C'est comme ça que nous arriverons tous ensemble de manière positive et concrète, a évolué sur le sujet. Merci cher collègue. La discussion. Générale est Close, nous passons la discussion du texte de la commission. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous indique que nous avons 29 amendements examiner. Et que s'agissant d'un espace réservé, d'une durée limitée à 4h je me verrais dans l'obligation de lever notre séance à 20h 35 que nous ayons ou non achevé l'examen du texte. Donc j'invite chacun chacune en tenir compte dans ses prises de parole, je vous remercie. À l'article 1er, deux amendements identiques, le l'amendement numéro de madame Vogel. Merci madame la présidente, je vais faire vite parce que je veux que la loi soit votée évidemment cet amendement il vise à supprimer le délai d'entrée en vigueur des dispositions de l'article qui a été fixée au 1er janvier 2029 sous proposition de la rapporteure. Voilà, tout simplement pour que. Ça soit appliqué plus rapidement. Je pense qu'on n'a pas autant d'années à attendre, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile et donc on veut que ce soit appliqué le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci le 15 même. La présidente de l'être. Oui le rapport de la délégation aux droits des femmes a relevé que les employeurs publics préféraient payer les pénalités financières plutôt que de nommer des femmes aux emplois direction cela est notamment le cas au sein de certains ministères aussi maintenir la possibilité d'une dispense de ces pénalités contribue à envoyer le signal selon lequel on ne peut s'exonérer de ses responsabilités en terme de parité. Le relèvement du taux de Primo nomination de chaque sexe de 40 à 45% à compter du 1er janvier 2025 et lors du prochain renouvellement des assemblées dans les communes et les. Il ne changera changera pas la donne. Comme je l'évoquais en discussion générale puisque pour 4 nominations, une unité d'un sexe est suffisante pour respecter cette obligation. Le présent amendement propose de revenir à la rédaction du texte initial et donc de supprimer la possibilité d'accorder une dispense de pénalité dès la promulgation de la présente, proposition de loi. Merci l'avis de la commission, madame la rapporteur. Un employeur à une pénalité financière dès lors que ces emplois relevant de sa gestion sont déjà occupés par à au moins 40% de femmes, d'une part et qu'aucune obligation légale n'impose un tel taux d'autre part, portant sur le stock d'emplois n'est pas entrée en vigueur, il n'est pas opportun de supprimer la dispense de pénalités financières offertes par l'article 132 tiré 8 du code général de la fonction publique, c'est donc un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Je le ferais très rapidement parce que je souhaite que le texte soit voté également madame la présidente. D'abord de raisons pour donner un avis défavorable à mon tour hein, de respecter les équilibres qui ont été ce et je le dis à ce stade du débat. Ça sera ma position assez constante. Vous, vous avez travaillé c'est trouver une position d'équilibre sur les dates sur les niveaux d'ambition fixée. Je trouve que ça se respecte. Ça c'est la position de de principes et ensuite. Le plus grosse avancée de ce texte au fond c'est d'introduire cette dispositif de stock d'emploi et je voudrais pas qu'on oppose cet objectif de stock Abdulatif. Temporel ou à un moment donné une année donnée de flux et donc je trouve que la position qui consiste à dire on privilégie le stock et l'exemption de sanctions, elle ne s'applique qu'aux administrations qui aurait déjà atteint le niveau de 40% me semble utile pour pas privilégier parfois des effets de rotation de turn-over au détriment du stock d'emplois féminisée donc pour cette raison là, je donne un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre, monsieur Marie. Question de quand même moi vous décidez comme vous voulez, bien entendu, vous avez. Tout votre temps moi ça nous dérange pas, j'arrêterais. 20h 30. Bien sûr, mais pas de prendre tout le temps, c'est simplement pour dire que nous allons voter ces deux amendements car nous considérons qu'effectivement reportée à 2029 la mise en oeuvre. De la suppression de ces distances n'est pas une bonne chose, donc nous allons voter. Merci. Alors je mets aux voix donc ces deux amendements identiques ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Donc il est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ne sont pas adoptés je mets aux voix l'article 1er qui est pour. Contraint qui s'abstient sont adoptés à l'article de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 17 mai, la présidente de la tante. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous proposons par cet amendement de rétablir le relèvement du taux de prime nominations à 50% comme cela a été proposé dans la version initiale de la proposition de loi, le taux de 45% retenu par la commission des lois appliquées en art et brandissant le résultat à l'unité inférieure, comme nous voulons de le dire ne frappe à passer un cap. Par rapport au droit actuel les considérations liées au sexe, encore trop souvent en raison de préjugés au détriment des femmes aussi. Seul l'établissement d'une parité stricte tout en maintenant la règle de l'arrondi inférieure permettra de garantir une certaine souplesse. L'amendement propose également de rétablir la possibilité de rattrapage initialement prévu tout en y apportant des modifications, il permet de retenir un quota de nomination de 50 à 60%, lorsque le taux de 40% n'est pas respectée sur le stock ou si l'objectif national de 40% sur le flux n'est pas respectée dans l'ensemble de la fonction publique. Cette disposition permettrait par ailleurs d'éviter de sanctionner les employeurs publics, dont la part de femmes dans les nominations réalisées au titre d'un cycle de référence serait considérée comme excessive, noter que l'amendement numéro 16 est un amendement de repli. Donc pour moi il est présenté. D'accord. Merci madame la présidente. L'avis de la commission, même la rapporteure. Ces amendements de la présidente de Lattre sont contraires à la position de la Commission, la commission a en effet estimé que l'augmentation du taux à 50% de personnes de chaque sexe dans les primo-nominations aux emplois supérieurs et de direction non seulement se heurterait à des difficultés d'application mais aussi aurait des effets contre-productifs pour les femmes elles-mêmes la 2ème disposition est quasiment satisfaite le relevé le relèvement à 45% du taux de personnes de chaque sexe que la commission a adopté rendrait tout à fait possible de nommer jusqu'à 55% de femmes ou d'hommes aux emplois visés d'ailleurs en l'état du droit, il est également possible de nommer jusqu'à 60% de femmes ou d'hommes, c'est donc eu un avis défavorable. Sur les deux amendements, nous sommes bien d'accord. Oui merci beaucoup. Il y avait du gouvernement, même avec le rapporteur, madame. Même avis merci je mets donc aux voix donc l'amendement 17 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Pour. Qui et contre. Qui. Tient n'est pas adopté l'amendement numéro 16 même vie même vote. Merci. Six amendement faisant l'objet d'une discussion commune le numéro 1 madame Vogel. Merci. Si madame la présidente. Donc cet amendement il a pour objet de rétablir le seuil des primo-nomination à 50% et non pas 45%. Je veux juste. Être éclairé sur, sur les 2 arguments qui ont été utilisées bon premièrement le fait que ce serait. Difficile à appliquer, notamment dans le le cas des nombres impairs. Alors il y a. Un article. Du code général de la fonction publique qui prévoit ça, donc c'est déjà prévu. C'est très simple, je vous lis l'article comme ça tout le monde sera peut être assuré. Qui dit le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommés en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure, c'est ce qu'on fait quand il y a un nombre impair donc la loi prévoit déjà ce cas en cas de nombres impairs. Il y a donc aucune difficulté à l'appliquer. Pour ce qui est du 2ème argument que ce serait contre-productif d'avoir 50% mais ce serait positif d'avoir 45% je veux dire franchement un peu de sérieux je sais cet argument qui consiste à raconter que la parité et le fait d'avoir vraiment une règle paritaire 50% c'est négatif pour les femmes mais par contre 45%, c'est positif. Je veux dire un peu sérieux, dites que vous voulez pas faire 50%

Le quota pour les primo-nomination d'abord fixée à 20% en 2013 et 2014 puis 30% en 2015 et 2016 a atteint son objectif de 40% en 2017. aucune augmentation et cela fait 6 ans que ce chiffre stagne alors que la logique voudrait que nous atteignons l'objectif final de parité soit 50%. C'est pour cela que je pense que les 40% ne suffisent pas, il faut ne pas insuffler un changement à la marge avec un passage à 45%, mais véritablement changer de braquet en inscrivant le taux des 50% tant attendue. le nombre de primo-nomination sera faible, la vitesse de renouvellement du stock sera faible. Également et le dispositif, on voit bien peinent à faire évoluer la féminisation des emplois donc inscrivons véritablement le principe de la parité et optons pour les 50% du taux de 1er primo nomination avec une application en 2020. Cette Et pour le sept. Madame la présidente, c'est un amendement de repli qui propose que les 50% du taux de Primo nominations hé bien vague en 2029. Merci l'amendement huit monsieur Marie. Merci madame la présidente. Dans sa rédaction actuelle. L'article 2 de cette proposition de loi exclut la fonction publique territoriale de l'entrée en vigueur dès 2025 du relèvement du taux de personnes de chaque sexe devant représenter 45% des nouvelles nominations. L'esprit de cette PPL, faut-il le rappeler, l'instauration de ces quotas repose pourtant sur un objectif. Primordial. Ils doivent être atteint dans les trois versants de la fonction publique. D'État, hospitalière et territoriale et et la loi Sauvadet avait déjà établi un calendrier échelonné donc ces obligations ne date pas d'hier. Donc, nous vous proposons de voter cet amendement qui vise à permettre une application harmonieuse de la loi dans les 3 volets de la fonction publique. Si l'amendement 26 monsieur le ministre. Un amendement du gouvernement le 26. Le par les, les débats s'agit de d'un d'un amendement qui est présenté par le gouvernement, effectivement, pour viser. Avoir un dispositif qui soit le plus effective possible pour des administrations parfois des collectivités qui partirait d'un niveau plus bas en matière d'équilibre de nomination et donc je porterai l'amendement identique pour la notion de flux et la notion de stock et je l'ai présente les 2 de façon cohérente. L'objectif c'est de pouvoir établir une première obligation, à partir de l'entrée en vigueur c'est-à-dire en en 2025 pour les administrations qui partirait de plus loin, d'avoir une obligation d'évolution de plus 3 points par rapport à la situation de départ sur la moyenne. Des primes aux nominations entre les années 2020 à 2022, ça permet de tenir compte de la réalité particulière, les administrations, je pense, pour prendre un exemple donné à des ministères sociaux. Les taux de féminisation sont beaucoup plus importants et donc en l'occurrence là où le sexe sous-représenté sont plutôt les hommes. Je prends l'exemple des ministères sociaux en 2020 sur 52 agents primo nommé 61% de femmes, 39% d'hommes. Et donc l'idée c'est d'introduire cette marche progressive 3 points par 3 points évidemment en ne remettant absolument pas en cause l'objectif d'arriver, c'est-à-dire 45% de prime aux nominations et 40% en stock. Je pense aussi à des plus petites collectivités, là où les viviers sont parfois moins important en matière de nomination et donc je pense qu'on aurait là un dispositif proportionnée donc efficaces. Merci le 21 madame Duranton. Merci madame la présidente, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l'article 2 prévoit que le nouveau taux applicable aux primo-nomination entrera en vigueur à l'issue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et des établissements de coopération intercommunale pour ce qui concerne les emplois supérieurs et de direction relevant de la fonction publique territoriale. Nous nous félicitons de l'adoption de ces dispositions qui laissera suffisamment de temps aux administrations communales pour s'adapter à la nouvelle exigence cependant nous constatons qu'aucune disposition n'est prévu pour les départements et les régions dont les assemblées délibérantes seront renouvelés en 2027 aussi, nous proposons de réparer cet oubli. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission, même la rapporteur sur ces amendements. Madame la présidente. Concernant les amendements ainsi c'est sept ils sont contraires à la position de la Commission. C'est donc un avis défavorable, ainsi que l'amendement huit de monsieur Marie l'amendement 21 de Madame Duranton. C'est un avis favorable. Il est en effet un complément utile. Et puis enfin l'amendement 26 du gouvernement. C'est un avis favorable aussi dans le sens où c'est une souplesse bienvenue que cette progression de 3 pour les employeurs qui nomme aujourd'hui moins de 40% de personnes de chaque sexe contre une obligation de 45% prévus par la loi. Merci. L'avis du gouvernement sur les autres amendements mais qui est le même que Madame la rapporteure sur l'ensemble des amendements qui ont été défendues. D'accord merci beaucoup. Alors je vais mettre aux voix donc l'amendement numéro 1 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est. Pour.

L'amendement numéro 8. Même avis même vote. L'amendement 26 du gouvernement qui a reçu un avis. Favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est donc. Adopté l'amendement 21 qui a reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est donc adopté l'amendement numéro 5 Monsieur Merci madame la présidente. Cet amendement vise à éviter que les villes les plus ambitieuses dans le recrutement des femmes fassent l'objet de sanctions ce qui est arrivé en effet les dispositions prévues par la présente, proposition de loi en son article 2 permettrait d'introduire une possibilité de rattrapage pour les employeurs qui présentent encore une situation déséquilibrée sur leur stock d'emplois fonctionnels, là où les plafonnement en vigueur actuellement sur le flux de nominations sont de nature à créer une inertie à cet égard, il apparaît toutefois utile d'aller au-delà de la condition tenant déséquilibre persistant sur le stock au sein de l'organisation et d'élargir le recours à cette faculté, même si l'employeur présente déjà un stock équilibré dès lors que l'objectif national de 40% de personnes de chaque sexe n'est pas atteint à l'échelle de la fonction publique dans son ensemble cet ajout aux dispositions prévues par la proposition de loi puis moins très d'en approfondir l'ambition mais aussi d'éviter toute pénalisation des employeurs les plus volontariste qui pourrait faire l'objet de pénalité au motif qu'ils ont nommé trop de femmes. Merci. L'avis de la commission, même la rapporteure. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur. Mes commentaires. Pour les amendements de Madame De Lattre numéro 17 SS. C'est donc une, un avis défavorable. Merci la vie de Monsieur le Ministre pour l'Auvergne. J'ai j'exprimais simplement un avis de sagesse puisque la nuance et la possibilité plutôt que l'obligation et donc en ça, j'émets un avis de de sagesse sur l'amendement. Merci Alors je mets aux voix donc l'amendement numéro 5 qui a reçu un avis défavorable de la commission. Un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. N'est pas adopté. L'amendement 25 du gouvernement, Monsieur le Ministre. madame la présidente. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, j'ai, j'ai pris l'engagement que pour les employes. Décision du gouvernement. S'agit des emplois de direction. Des emplois de cabinets ministériels sur lequel le vivier est plus important, 311 postes concernés. Le gouvernement se fixe l'objectif d'atteindre effectivement la parité ce n'est pas contradictoire avec la position du gouvernement sur les amendements précédents mais justement. À la fois dans un objectif d'exemplarité sur les emplois. Décision du gouvernement et parce que on sait que on bénéficie d'un vivier qui est plus important, il est plus facile de pouvoir se fixer cet objectif de parité et de ne pas tomber dans les travers qui conduisait une position défavorable sur les amendements précédents qui est parfois d'avoir des employes près fléché si je puis dire parce qu'on est sur un plus petit Vijay sur. Des emplois. Sur chacun des sexes et non pas sur les compétences et donc je vous propose de l'inscrire dans la loi. Cet engagement du gouvernement de fixer une parité parfaite des emplois à sa décision. Merci l'avis de la commission. Même le rapporteur. Je comprends l'intention du gouvernement de faire preuve de la plus parfaite exemplarité pour la parité des emplois qui sont à sa décision. Pour autant, je continue d'avoir des réserves, s'agissant du taux de 50% qui me semble comporter des difficultés inhérentes sera donc un avis de sagesse. Merci beaucoup. Alors je vais mettre aux voix donc l'amendement 25 du gouvernement qui a reçu un avis de sagesse de la commission qui est pour.

Qui est contre. Qui s'abstient. Ce n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour. Contre qui s'abstient. Il est donc adopté l'article 3 2 amendements identiques, le neuf monsieur Marie. Merci madame la présidente. Cet amendement vise à abandonner la référence à un seuil démographique et à exprimer ce seuil en nombre d'emplois fonctionnels en généralisant l'obligation de nomination équilibrées dès lors que la collectivité dispose d'un nombre d'emplois fonctionnels supérieure ou égale à trois, ce qui évitera toutes les discussions sur 40.000 ou 20.000 merci. Merci l'amendement 18, madame la présidente. D'accord. Alors la ville. La commission, madame la rapporteure. En effet, les autorités territoriales ne sont aujourd'hui pas obligés de déclarer la création d'emplois fonctionnels, faire des formes pendre l'application de l'obligation de nomination équilibrée de ce seul critère semble donc susceptible d'engendrer des difficultés de mise en oeuvre en outre ce critère ne permet pas de garantir que les employes fonctionnel en question sont occupés par des agents de catégorie A plus. Or l'obligation de nominations équilibrées a vocation à s'appliquer aux emplois supérieurs de direction occupé par de tels agents enfin il ne faudrait pas que, en conséquence d'une telle disposition que les collectivités territoriales soient réticentes à créer des emplois fonctionne fonctionnelle par crainte de se voir à appliquer l'obligation de nominations équilibrées. C'est pourquoi le système actuel qui combine les 2 critères de population et du nombre d'emplois fonctionnels me semble efficace. Ce sera donc un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. J'ai j'ai le même avis que le rapporteur, il me semble que c'est important d'appuyer le dispositif législatif sur des données parfaitement objectif qui en l'occurrence en ce qui concerne les données démographiques sont relevés par l'Insee et bon nombre de dispositions dans notre droit sont déjà appuyé sur ces dispositions qui sont relevés par l'Insee. Les données sur lequel vous proposez d'appuyer son effectivement sur la base déclarative. Donc il me semble que sur la robustesse. Juridique de ce que nous pourrions aujourd'hui produire il vaut mieux s'en tenir aux textes issus de la commission et donc un avis défavorable. Merci. Alors je vais mettre aux voix donc les amendements identiques ne fait 18 qui ont reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est. Pour.

Merci madame la présidente. Cet amendement propose d'opter pour l'arrondi supérieur à la place de la règle selon laquelle le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommé est arrondi à l'unité inférieure, je reprendrai l'exemple donné par ma collègue Delattre. Lors de la discussion générale, lorsqu'il y a 4 personnes concernées, là on dit inférieur, fait que ce sera une femme et pas de et donc systématiquement nous n'avançons pas en matière de parité. Merci. L'avis de la commission, madame la. Lors de Lors de l'examen du texte. Nous sommes effectivement demandé s'il était possible d'opter pour la règle de l'arrondi à l'unité supérieure. Les effets d'une telle règle combiné un taux de 45% 45% auraient été variable dans le versant territorial pour les collectivités territoriales pour lesquels l'obligation de nominations équilibrées s'applique sur un cycle de 4 nominations la combinaison du taux de 45% avec la règle de l'arrondi à l'unité supérieure. Équivaudrait à 50% les collectivités territoriales seraient ainsi contrainte de nommer strictement 2 hommes et de femmes sans aucune marge de manoeuvre possible dans les autres versants la combinaison du taux de 45% avec la règle de l'arrondi à l'unité supérieure aurait dans certains cas correspondu à un taux de 47 ou 48% mais d'autres cas, cela serait revenu à un taux de 50% également. Or la commission a estimé qu'un taux de 50% poserait de fortes difficultés d'application, pratiques et risquerait d'avoir des effets contre-productifs dans ces conditions l'alternative aurait pu être de conserver un taux de 40% tout en optant pour la règle de la ronde à l'unité supérieure. Nous avons toutefois considérer que le relèvement du taux à 45%, tout en gardant la règle à l'arrondi de l'unité inférieure constituée l'option la plus lisible et la plus efficace et donc un avis défavorable. Merci Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement. Écarterait pas d'un pouce de l'argumentation minutieuses et précises données par Madame la rapporteure et donc le travail de la commission et même avis que le rapporteur. Merci donc je mets aux voix l'amendement numéro 11 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. C'est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Pass adopté l'amendement 19, madame la présidente de l'être. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la création d'une commune nouvelle la fusion d'intercommunalité ou encore l'extension d'un périmètre intercommunal exige une réorganisation administrative laborieuses et impliquent bien souvent des recrutements au sein des services préexistants. Cette évolution périmètre peut soulever des difficultés d'application du quota de Primo nominations paritaire en cas de franchissement abrupt du seuil de 40.000 habitants. Ainsi, pour tenir compte de ce cas de figure bien précis. Le présent amendement propose de leur accorder un délai de 2 ans à compter de la date du transfert de compétences résultant de la création de la modification de périmètre pour se mettre en conformité. Si l'avis de la commission, même la rapporteure. Je comprends assurément la volonté d'éviter une situation une collectivité territoriale se voit soudainement appliqué l'obligation de nominations équilibrées parce qu'elle a franchi le seuil des 40.000 habitants. Pour autant, la disposition par madame de de Lattre, ne me paraît pas nécessaire. Tout d'abord je rappelle que la proposition de loi, telle qu'adoptée par la commission des lois ne modifie pas le seuil d'application de l'obligation de nominations équilibrées, celui-ci reste fixée à 40.000 habitants, comme il l'est depuis 2019. Par ailleurs le droit existant prévoit d'ores et déjà une souplesse dans l'application de l'obligation de nominations équilibrées en cas de fusion de collectivités territoriales ou EPCI ainsi la nomination dans les 6 mois à compter de cette fusion d'un agent qui a occupé un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est exempté de l'obligation de nominations équilibrées. S'agissant du cas de création de commune nouvelle il faut noter qu'à l'heure actuelle la population moyenne des communes nouvelles et de 3500 habitants et que seuls 36 communes nouvelles ont une population de plus de 10.000 habitants, vous le savez bien, ce sont essentiellement des communes de petite taille qui se regroupent pour former des communes nouvelles commune nouvelle dépasse les 40.000 habitants, c'est souvent parce qu'elle est issue d'un regroupement d'une ville de taille importante qui était déjà soumises à l'obligation de nominations équilibrées et d'une ou de plus petites villes, dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de prévoir une disposition transitoire à destination des communes nouvelles. C'est donc un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Peut-être une proposition de retrait puisque je trouve que l'argumentation de la rapporteure monte que le droit actuel satisfait. Cette souplesse telle qu'elle avait proposé et donc retrait ou avec des phares du gouvernement. Merci madame la présidente. On mets aux voix n'est retiré. Merci. Je me vois l'article 3 qui est pour. Contre qui s'abstient et donc adopté. Un article additionnel après l'article 3, Monsieur Marie. L'amendement 14. Merci madame la présidente. L'article L 132 8 du code général de la fonction publique, dispose qu'une contribution est du en cas de non respect de l'obligation de nominations équilibrées. Si cette contribution doit inciter à une mise en conformité. Elle est malheureusement parfois. Contournées et perdre alors de son intérêt. Notre groupe défend donc un renforcement de la sanction en proposant de la rendre publique car il serait inconcevable qu'un employeur public puisse persister à suivre. De mauvaises. Habitudes tout en bénéficiant d'une discrétion totale sur le non-respect de ses obligations paritaire le manque de transparence est à nos yeux un obstacle à lever pour s'assurer que le versement de cette contribution est systématiquement une finalité qui permettent de transformer la situation. Merci. L'avis de la commission, même la rapporteure. qui est dressée chaque année par la direction générale de la mine et de l'administration et de la fonction publique et publié sur le site internet du ministère de la transformation. Et de la fonction publique cette publicité découle de l'article IV du décret du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nomination équilibrée dans l'encadrement supérieur de la fonction publique, la publicité des sons des sanctions et donc déjà prévu par décret. Il n'est donc pas nécessaire de la prévoir par la loi, une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable mais il n'en reste pas moins qu'il conviendrait de réduire le décalage qui existe actuellement entre les nominations et le bilan qui, en effet, le dernier bilan de la mise en oeuvre de l'obligation de nominations équilibrées remonte à juillet 2021, pour la. Mais l'année 2019. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente. Même avis que la la rapporteure peut être là aussi plutôt une demande de retrait. Parce que le, le, la demande est satisfaite par la loi et la publication dans le rapport effectivement annuel. Peut être en y ajoutant un engagement de la part du gouvernement. Ça a été mentionné à la tribune. Aujourd'hui, le dispositif est pas suffisamment opérant parce qu'on publie, avec 2 ans de retard. Les données et donc on n'a pas ce suivi effectif. Qui serait nécessaire pour pouvoir faire bouger les lignes et donc moi je souhaite que nos droits soient réellement performatif et donc je prends ici l'engagement que à partir de l'année prochaine on publie systématiquement avec les données de l'année précédente et non pas avec les données de 2 ans. Antérieurement. Voilà l'engagement que j'ajoute peut-être pour justifier une demande de retraite. Merci, monsieur le Ministre, on prend acte de votre engagement. On vérifiera effectivement qu'ils soient tenus et donc nous retirons cet amendement. Merci. L'amendement 28, Monsieur le Ministre. L'amendement du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Il s'agit, je l'ai mentionné tout à l'heure d'harmoniser le dispositif de sanctions qui va reposer sur. Les différents dispositifs que nous mettons en oeuvre dans la loi pour avoir une harmonie entre l'objectif que nous nous fixons sur les flux de nomination des stocks de nomination et la non-. Publication de l'index. Aujourd'hui, tels que le texte est issu de la commission vous auriez. Des. Dispositifs de sanctions forfaitaire sur les flux de nomination de sanctions forfaitaire sur la non-. Publication de l'index, mais un objectif de sanctions qui irait jusqu'à 1% de la masse salariale sur le stock de nomination et donc ma proposition au nom du gouvernement est assez simple, c'est d'avoir un dispositif de sanctions harmoniser forfaitaire, 90.000 euros par unité manquante. Pour le stock de, de, le le jeudi de stock de nomination des objectifs de flux de nomination et la non-. Publication de l'index et donc c'est ceux-ci que je vous propose de modifier par amendements. Merci. L'avis de la commission, même la rapporteure. La commission a introduit un taux obligatoire de 40% de personnes de chaque sexe au sein des employes supérieurs et de direction et la sortie d'une sanction financière pouvant aller jusqu'à 1% de la rémunération brute globale annuelle de l'ensemble des personnels. Elle a précisé qu'il s'agissait là d'un plafond et que le montant précis de la pénalité pouvait être modulée en tenant compte notamment de la situation initiale de l'administration. S'agissant de la représentation des femmes au sein des employes visés le plafond de 1% de la rémunération brute annuelle globale des personnels correspond à un montant suffisamment dissuasif pour garantir le respect de l'obligation posée du reste il correspond au montant prévu dans le secteur privé par la loi Rixain de décembre 2021, à l'inverse, prévoir une sanction d'un montant forfaitaire qui serait fixé par décret ne semble pas suffisamment dissuasif. De surcroît, la rédaction de l'amendement du gouvernement laisse entendre que le montant forfaitaire ne serait lui-même qu'un plafond et pourrait être modulé, ce qui tend à affaiblir encore le caractère dissuasif de la sanction. Je pense qu'il faut être cohérent, si nous prévoyons une obligation, il faut également prévoir une sanction con conséquente. C'est donc un avis défavorable. Un instant sans sans rallonger les les débats pour que ce soit parfaitement clair sur ce qui est proposé par le gouvernement. Ce que nous proposons, c'est d'avoir un dispositif de sanctions sur l'index telle qui sera créé. Forfaitaire pour la non-. Publication de l'index me semble assez logique, soit on publie son publie pas et donc le dispositif de sanctions forfaitaire semble assez logique et que ensuite soit pas que laisser penser à la représentation nationale qu'on ne souhaite pas mettre en place une petite sanction ensuite sur une non-évolution à partir de à partir de situation de départ défaillante sur l'index nous prévoyons bien et c'est ce que prévoit l'amendement concernés de mettre en place un dispositif de sanctions pouvant aller lui jusqu'à 1% de la masse salariale comme cela s'applique pour le privé. Donc on aurait un dispositif qui serait symétrique entre ce qui serait proposée pour le privé et pour le public forfaitaire pour le stock forfaitaire pour le flux forfaitaire pour la non-. Publication de l'index, mais en revanche, si les administrations concernées n'évolue pas dans le bon sens à partir d'une situation de non satisfaisante pour l'index alors on irait un dispositif de sanctions pouvant effectivement aller jusqu'à 1%, la masse salariale. Voilà, je voulais qu'il y ait aucune ambiguïté dans le dispositif proposé et donc on n'a pas un dispositif qui amoindrit le dispositif de sanctions qui est prévu dans le cadre du privé. Merci. Alors je mets aux voix l'amendement. 28 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient donc pas adopté. Un amendement et un sous-amendement donc le 13 monsieur Marie. Merci madame la présidente. Notre groupe est particulièrement favorable à cette partie du dispositif qui permet d'agir véritablement sur le stock. Par l'instauration, donc d'un taux minimal de 40% de personnes de chaque sexe. Et donc ici aussi. Nous proposons de rendre publique la pénalité financière prévue en cas de non respect de l'obligation. Cette publication n'étant pas encore prévu à moins que monsieur le ministre s'engage là aussi à le faire. Merci madame Vogel pour l'abonnement, 30. leur amendement et le leur volonté dans public. Les les pénalités financières et ce sous-amendement il rajoute simplement une chose, c'est un délai dans lequel cette publication devrait intervenir pour éviter que ben si c'est publié vraiment longtemps après c'est complètement déconnecté de la situation qui a été sanctionné, hé bien ce sera sans doute moins utile. Voilà, c'est simplement ça. Encore merci à dos collègue socialiste. Merci. Alors même la rapporteure. L'avis de la Commission pour l'amendement et le sous-amendement. Le texte adopté par la commission prévoit un certain nombre de publications. L'article 4 prévoit la publication annuelle sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique des écarts de représentation entre les hommes et les femmes au sein des employes supérieurs et de direction. Il prévoit également l'application d'une sanction financière en cas de non-publication, prévoit quant à lui l'obligation de publication d'objectifs de progression par l'employeur public qui ne se conforment pas au taux de 40% sur le stock des emplois supérieurs et de direction la publicité du respect de l'obligation relative à la répartition serait donc assuré pour autant. Le texte ne prévoit pas pour l'heure, de façon expresse, la publicité des sanctions. L'amendement du groupe socialiste paraît donc bienvenu, c'est un avis favorable. S'agissant du sous-amendement 30 qui prévoit que la publication des sanctions infligées intervienne au plus tard trois mois après, je suis favorable à ce sous-amendement également. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis favorable que Madame la rapporteure. Vous m'avez demandé de prendre cet engagement. Il est évidemment pris mais ce ne fera pas de mal de l'inscrire dans la loi. Merci. Alors je mets aux voix l'amendement 30 qui a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement enfin le sous-amendement je mais on peut voir. C'est pour. Qui il est contraint qui s'abstient donc adopté je mets maintenant aux voix l'amendement 13 qui a reçu donc un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Contre qui s'abstient donc adopté ainsi sous-amendé. L'amendement 10 semaines filleuls. La présidente donc. Nous savons et nous avons déjà partagé sur la cible des primo-nominations pour dire qu'elle n'alimentait pas suffisamment le stock et donc avec mon groupe nous partageons la volonté d'aller jusqu'à 40% pour pour l'instauration d'un quota du du du stock je dis bien simplement, nous ne pouvons pas attendre 2029, comme il nous les proposer. Et pour rappel je vous je vous dis que dans le rapport de la délégation aux droits des femmes. Il a été proposé donc une application immédiate et je vous propose ce compromis donc d'une application à 2027. Merci. L'avis de la commission, madame la rapporteure. La commission a jugé pertinent de complique de compléter l'obligation portant sur les nominations d'une obligation portant sur la représentation des femmes et des hommes au sein des employes supérieurs et de direction mais nous sommes conscients que si la féminisation des nominations et progressive, celle des emplois effectivement, occupés l'est encore plus. C'est pourquoi nous avons par réalisme fixé à 2029 l'entrée en vigueur de l'obligation portant sur le stock afin de laisser le temps aux administrations de s'adapter et de mener la politique de ressources humaines permettant d'atteindre cette cible, la date de 2029 alors que nous sommes au printemps 2023. Et d'ailleurs déjà ambitieuse. Je rappelle que dans le secteur privé, plus de 7 ans ont été laissés aux entreprises de plus de 1000 salariés pour se conformer à l'obligation de 40% de femmes et d'hommes au sein des employes, dirigeant la loi adoptée en décembre 2021 a en effet prévu une entrée en vigueur au 1er mars 2029. C'est pourquoi avancer la date à 2027 ne me paraît pas pertinent. C'est un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, j'ai indiqué tout à l'heure je souhaitais respecter l'équilibre issu de la commission qui a permis l'adoption unanime du texte en commission et comme c'est vraiment l'objectif que je partage aujourd'hui j'aimais le même avis que Madame la rapporteure. Merci. Alors je mets aux voix l'amendement dit ce qu'il a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. C'est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement 27 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Je le défendrai extrêmement brièvement puisque je l'ai défendu tout à l'heure j'en ai défendu le font avec l'abondement 26 il s'agit de fixer des marches progressive sans rien renier à l'objectif d'arriver donc c'est le même amendement qui est présenté ici pour le stock de domination. Merci Monsieur le Ministre, l'avis de la commission, madame la rapporteure. L'amendement du gouvernement tente donc à donner un peu plus de temps aux employeurs publics dont les emplois supérieurs et de direction sont occupés aujourd'hui par moins de 37% de personnes de chaque sexe pour ses employeurs là l'obligation ne sera pas un taux de 40% de personnes de chaque sexe en 2029 mais l'obligation d'une progression de 3 tous les 3 ans jusqu'à ce que le taux de 40% soit atteint. Cette mesure me semble apporter une souplesse bienvenue c'est un avis favorable. Merci. Alors je mets aux voix donc l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient et donc adopté. Je me vois l'article 3 bis qui est pour. Contre qui s'abstient. Il était adopté, à l'article 4, j'ai trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. On commence par le 24. Monsieur le ministre à moment du gouvernement. Oui madame la présidente. D'un mot et sans rallonger la durée des débats. Ils en profitent pour saluer. L'introduction de l'index dans le texte de loi et je l'espère son son adoption ça sera, je l'ai dit tout à l'heure. Un pas important pour la fonction publique pour son efficacité pour son attractivité et pour son exemplarité. Et je crois que nous partageons assez unanimement et sur tous les bancs cet objectif cet amendement il vise à apporter 3 modifications ou précisions au dispositif adopté par la commission. La première serait de renommée, l'index en lui donnant les mots index d'égalité professionnelle permettrait d'avoir une approche assez large de ce que le gouvernement souhaiterait faire de l'index, c'est-à-dire un outil qui nous permettent de mesurer à la fois les inégalités salariales. C'est un des objectifs visés par l'index mais aussi qui nous permettent de mesurer les égalité en matière de nomination et le titre actuellement ne recouvre pas cette dimension-là et aussi la présence des femmes. postes les plus à plus forte influence ou à plus forte rémunération et donc il me semblait que l'intitulé d'index égalité professionnelle recouvrer l'ensemble de ses dimensions et c'est la raison pour laquelle je je proposais ce modification ensuite ce sont des modifications de précisions pour préciser à la fois la référence au CNDP. Dans la territoriale et puis d'inclure aussi dans le Champ de l'index les établissements de la fonction publique hospitalière. Je crois que nous partageons cet objectif-là enfin et c'est peut être l'essentiel. La proposition que je souhaiterais vous faire à travers cet amendement c'est d'accélérer la publication de l'index, pourquoi en le basant sur les données que l'administration est capable de fournir pour la fonction publique d'État, là aussi, prendre l'engagement que sur la base des données que nous publierons au printemps on puisse d'ici la fin de l'année, publié pour une première fois cet index étant donné que, après, je souhaiterais qu'soit publié à chaque fois en juin pour les trois versants. De la fonction publique et puis pour les collectivités et la fonction publique hospitalière. Sur la base, sur la base pardon des données fournies par les administrations, ces 2 versants. Sur le printemps 2024, permettre la publication. Au plus tard au 31 décembre 2 villes, 24. Je précise que ces dates que je soumets à votre vote sont l'issue des dialogues et des échanges que nous avons pu avoir avec l'ensemble des employeurs territoriaux les employeurs hospitaliers et nous semble raisonnable de permettre une accélération si vous en été. D'accord de la publication de cet index. Merci, monsieur le Ministre, l'amendement 29 de la commission des lois. Madame la rapporteure. Cet amendement vise à compléter la liste des employeurs publics redevable de la pénalité financière en cas de non-, publication des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il permet d'y intégrer les établissements publics de l'État ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, l'amendement précise que dans la fonction publique hospitalière. Chacun des établissements publics mentionnés à l'article 5 seraient redevable de la sanction et non le Centre national de gestion.

après. L'entrée en vigueur de la loi. Nous proposons simplement que l'index applique au moment où la loi entre ça paraît logique. J'avoue que je ne vois pas trop les raisons pour lesquelles s'appliquerait plus tard. Et voilà pour qu'il puisse être opérationnel au plus vite et efficace au plus vite. Je vous remercie. Merci la avis de la commission, même la rapporteur. Alors 4. L'amendement du gouvernement procède à de nombreuses modifications de l'article IV de portée inégale certaines modifications sont bienvenues et en procédant à des corrections. D'autres sont rédactionnels ou apporte des précisions qui ne sont pas indispensables, tel est le cas de la publicité des indicateurs prévus sur le site internet de l'employeur. D'autres portent sur l'articulation des articles au sein du code général de la fonction publique, le gouvernement propose de réserver la section créée par l'article à l'index relatif à l'égalité professionnelle et supprime donc les dispositions relatives aux écarts de représentation cette question peut être discutée en revanche certains points me ne me semble inopportun. Premièrement la suppression du non-cumul entre la sanction prévue pour non-. Publication de l'index et celles prévues pour non élaboration du plan en faveur de l'égalité professionnelle ne paraît pas justifié. Deuxièmement, les dates d'entrée en vigueur proposé semble moins opérationnel que les dates d'entrée en vigueur initial. C'est pourquoi je vous proposerai un avis défavorable à cet amendement et d'adopter à la place l'amendement que je vous ai présenté afin de compléter la liste des employeurs publics redevables d'une pénalité financière en cas de non-. Publication de l'index.

ne paraît pas adapté en effet la base de données sociales à partir de laquelle est élaboré le rapport social unique n'est disponible qu'au printemps de chaque année en outre dans les versants territorial et hospitalier. La base de données sociales ne sera mise en oeuvre pour la première fois seulement en 2024 au titre des données 2023 une entrée en vigueur différée et donc nécessaire. C'est donc un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Même avis que le rapporteur sur l'amendement numéro 4 et ensuite sur le principe de ce qui est contenue dans l'amendement madame la rapporteur l'amendement 29, je suis évidemment favorable puisque. Il vise un objectif convergents avec une des mesures que je propose dans l'amendement gouvernemental mais je maintiens. L'adoption ou la proposition d'adoption de l'amendement gouvernemental qui est plus complet, notamment sur l'accélération de la publication des dates. Voilà, je prends l'objectif ici très simple et opérationnelle que nous serons prêts à publier et. Cette issue aussi, je le répète du dialogue que nous avons eue avec les employeurs territoriaux et hospitaliers. Merci alors je mets aux voix donc l'amendement 24 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Et donc pas adoptée, je mets aux voix l'amendement 29 de la commission qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Contre ça. Tiens et donc adopté je mise aux voix l'amendement numéro 4 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre qui s'abstient. Pas adopté. Un moment vend même la présidente de être. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la création dans l'index de l'égalité professionnelle et cohérente par rapport aux obligations qui s'imposent désormais en la matière dans le secteur privé. Toutefois, il est nécessaire de tenir compte des difficultés d'application qui peuvent apparaître en cas d'évolution du périmètre d'une commune ou d'une intercommunalité lorsque le seuil de 40.000 habitants le présent amendement propose d'accorder un délai de 2 ans de ces collectivités pour se mettre en conformité avec les obligations relatives à cet index. L'amendement 20 de madame De Lattre vise comme son amendement 19 à l'article 3 à prévoir une disposition transitoire en cas de franchissement du seuil de 40.000 habitants. Je ne reprendrai pas là les arguments que j'ai exposées à l'occasion de l'article 19 je rappellerai en plus.

transitoire proposée par Madame De Lattre, ne me paraît pas nécessaire. C'est un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, même avec la portable. Merci. Alors je mets aux voix donc l'amendement numéro 20 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. je mets aux voix l'article 4 et pour. Les contraintes qui s'abstient. Il est adopté. Après l'article 4 à l'amendement 22 madame Duranton. Merci madame la présidente. Donc l'amendement numéro 24 du gouvernement ayant été rejeté. Donc je le, je retire mon amendement. Quand vous avez l'amendement 23. Merci madame la présidente. Donc la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique à instaurer l'obligation pour les collectivités territoriales de plus de 80.000 habitants et les EPCI à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants de publier chaque année sur leur site internet, la somme des 10 rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre et cela en précisant le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces mêmes rémunération donc dans un souci de cohérence d'harmonisation et de lisibilité, nous vous proposons de réduire à 40.000 habitants. Le seuil de population à partir duquel s'applique cette obligation. serait identique à celui applicable à l'obligation de nominations équilibrées et à l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et entre les femmes et les hommes. Si l'avis de la commission, madame la rapporteure.

est contraint qui s'abstient. Il est donc adopté monsieur Marie pour l'amendement numéro 12. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Nous allons dans un instant.

je sais que le Sénat n'est pas très friand des rapports mais. Au regard de l'ambition affichée des difficultés rencontrées. Jusqu'à présent pour atteindre les objectifs fixés, il nous semblerait nécessaire. Que le gouvernement nous présente à l'horizon 2028 un rapport. Exhaustif sur les avancées de telle sorte que nous puissions ensuite si nécessaire. De nouveaux légiférer pour atteindre la parité, le plus vite possible dans les 3 fonctions publiques. Merci. Merci l'avis de la commission, même la rapporteure. Il est bien sûr important de veiller à ce que les lois soient appliquées. Mais en l'espèce, il semble que les mesures de suivi soit déjà prévu pour les articles de la présente, proposition de loi ou des textes réglementaires. Il en est ainsi des écarts de rémunération et de représentation entre les femmes et les hommes qui doivent faire l'objet d'une publication par les employeurs publics. Il en est également ainsi de l'obligation de nomination équilibrée dont le bilan est assurée et publié chaque année par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. N'allons pas donc prévoir le suivi des instruments de suivi du reste, quand bien même le principe d'un tel rapport serait justifiée la date proposée ne sont pas pertinentes, pourquoi le 1er janvier 2028 alors que l'obligation du taux de 40% sur le stock d'emplois supérieurs et de direction n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2029 c'est donc un avis défavorable. Si l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, je. J'ai pris ce soir beaucoup d'engagement devant le sénateur auprès des sénateurs Marie et de l'ensemble la représentation nationale. Je partage exactement l'avis émis par madame la la rapporteure, effectivement il y a chaque année. Des documents qui sont transmis au Parlement et notamment le rapport relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique qui est déjà prévu dans la loi et donc, si je puis ajouter. Cet engagement-là supplémentaires. Je serais très heureux. Chaque année, de venir le présenter peut être devant la délégation du droit des femmes qui nous permettrait d'avoir un moment de rencontres. D'échanges, de dialogue et peut être avec une exigence accrue et convergentes pour continuer à faire bouger les lignes à moderniser notre fonction publique et a montré qu'elle sait aujourd'hui se rendra plus attractif et plus efficace. Donc même avis que Madame la rapporteure mais engagements pris si vous en êtes d'accord de venir présenter les rapports déjà prévu devant la chambre haute. Merci monsieur Marie. Simplement. Les amendements que nous déposons ne sont pas sans intérêt. La preuve c'est qu'ils obtiennent désengagement multiples de la part du ministre et donc nous en prenons acte et je retire mon amendement. Merci, merci beaucoup alors. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Donc. Madame la présidente, Lyon pour explication de vote. Merci madame la présidente. Tout d'abord je voudrais remercier la rapporteure Françoise Dumont. La commission des lois et le ministre pour le travail de coconstruction que nous avons eue avec les auteurs de la proposition Martine Filleul et Dominique Vérien. Je voudrais aussi dire que. Même si de nombreux sénateurs ou sénatrices ne sont pas favorables au quota au Seuil. Les quotas et les seuils sont nécessaires. Sinon on recule en terme d'égalité et donc c'est, c'est pour cette raison qu'il est important en permanence de cranté des des j'entends oui. Chers collègues, chers Matine la volonté d'un d'aller plus loin. Nous avons réussi à trouver un consensus avec la commission des lois, avec le Sénat et je crois que c'était important. Donc oui, on sera amené à errer sur c'est sur cette égalité dans la fonction publique parce que oui il y aura forcément des choses à faire mais nous pourrons d'ores et déjà tiré le bilan de ce qui a été fait, je me réjouis et je souhaite remercier à cet instant, aussi le groupe Union centriste pour avoir pris l'initiative d'inscrire cette proposition de loi dans sa niche puisqu'il y avait trois auteurs donc elle aurait pu être inscrite. Dans différentes niches et et le président Marseille nous a donné la possibilité de l'inscrire, donc c'était important. Je dois dire à monsieur le le ministre que nous avons entendu ses engagements donc nous le remercions pour les engagements qu'il a pris à la fois en terme. De rendu, mais aussi que vous serez bien entendu le bienvenu dans au sein de la délégation pour nous exposer. Tous ces éléments, donc c'est un pas supplémentaire, c'est pas, c'est ça ne s'arrête pas aujourd'hui le groupe Union centriste évidemment votera cette proposition de loi. Merci à Martine Filleul et Dominique Vérien qui avait fait un excellent travail sur le les 10 ans de la loi Sauvadet et que ce travail a forcément inspiré ce texte que nous dont nous avons débattu ce soir, merci. Merci monsieur Richard. un premier pour rendre hommage au travail d'amélioration du texte initial qui a été réalisé par la Commission et par le Sénat en débat de ce jour un 2ème mot pour vous dire que, malgré cela je ne voterais pas ce texte, je m'abstiendrai. Parce que je fais partie des personnes je ne sais pas si elles sont nombreuses, mais des personnes qui n'aime pas les quotas, je le dis depuis de longues années. Et je je suis malheureusement aujourd'hui cohérent. Je vous remercie. Merci. Alors je vais mettre aux voix, donc l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique Qui est contre. Qui s'abstient. Je vous remercie. Le texte est donc adopté. Mes chers Mes chers collègues. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observation. Je considère ces conclusions comme adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance jeudi 6 avril 2023 à 10h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie. La séance est levée et je vous remercie beaucoup d'avoir tenu les délais merci bonne soirée.